La séance est ouverte. Le compte-rendu intégral de la séance du jeudi 16 février, a été publié sur le site internet du Sénat. Nous n'avons pas reçu d'observation. y en a-t-il en séance. Je n'en vois point. Le procès verbal est donc adopté. La Première ministre, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, le port du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. Notre séance et retransmise. En Direct sur Public Sénat et notre site Internet. Chacun sera attentif au respect des uns et des autres et de celui du temps de parole. Je vais donner la parole tout de suite. À notre collègue. Thani Mohamed Soilihi. Pour le groupe du Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants. Vous avez la parole. Merci monsieur Merci monsieur le président, monsieur le garde des Sceaux. Le gouvernement a pris la mesure des enjeux liés à la justice dans notre pays puisqu'en 5 ans le budget qui lui est consacré, a augmenté de plus de 40%. Vous avez fait de la mise en oeuvre d'une politique de justice de proximité l'une de vos priorités et le groupe RDPI s'en réjouit. L'objectif poursuivi est d'apporter une réponse judiciaire concrètes et rapides aux petits actes de délinquance qui pèse lourdement sur le sentiment d'insécurité et le bien vivre-ensemble et dans le traitement jusqu'à présent entamer la confiance des citoyens envers l'institution judiciaire. Ce besoin de réassurance tout comme le redressement de notre justice passe par des mesures supplémentaires financier tout d'abord, et c'est avec satisfaction que nous observons de manière inédite et pour la 3ème année consécutive que le budget augmente de plus 8% humain également avec le lancement d'un vaste plan d'embauche de magistrats et de fonctionnaires le renfort qui a été apportée aux magistrats depuis 2020 de 2000 contractuels notamment a permis une réduction significative des affaires en attente de jugement. Ce dont nous nous félicitons lors d'un déplacement au tribunal judiciaire de Reims. Vous avez annoncé la CDI sation de ces contractuels. Cette mesure se participera à la lutte contre la précarité et l'emploi dans la fonction publique de l'emploi dans la fonction publique. Vous avez également signifier votre intention de poursuivre la consolidation de l'équipe pour les magistrats. Avec le recrutement de 300 juristes assistants supplémentaires et la création de la fonction d'attaché de justice monsieur le garde des Sceaux, pourriez-vous nous préciser quels seront les contours de cette nouvelle fonction d'attaché de justice, ainsi que le calendrier du déploiement du plan d'action pour la justice que vous avez présenté à l'issue des états généraux. On nous répond, la parole est comme monsieur Éric Dupond-Moretti Garde des Sceaux, ministre de la justice. Monsieur le garde des Sceaux, vous avez la parole. Merci monsieur le président, Mesdames, messieurs. Les sénateurs, Monsieur le Sénateur, Mohamed. Soihili grâce au budget que le Sénat a voté à chaque fois depuis 3 ans les 2000 contractuels dont les 900 juristes assistants que nous avons recruté ont apporté depuis 2017 une aide particulièrement précieux aux magistrats et aux greffiers de notre pays. D'ailleurs nous avons obtenu un déstockage des dossiers en attente, en matière civile de l'ordre de 30%. Grâce à madame, la Première ministre. J'ai annoncé dès lundi le recrutement de 300 juristes assistants supplémentaires cette année. Cependant, leur statut actuel, vous le savez est insatisfaisant trop précaire, il ne prévoit aucune formation, pas davantage que la définition des tâches qui sont les leurs. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de créer une fonction d'attaché de justice ouverte tant aux fonctionnaires qu'aux contractuels pour que partout dans nos territoires les attachés de justice soit présent l'émission seront définies les attachés de justice prêteront serment ils recevront une formation donnée par l'ENM. Ils formeront par ailleurs hein Villiers indispensable au recrutement massif de 1500 magistrats à venir. Une passerelle spécifique leur permettant l'accès à l'ENM sera envisagée et enfin tous les contractuels justice de proximité de catégorie A, B et C seront cédées Izé dans leur poste. Afin de concrétiser ses annonces. Je présenterai la nouvelle loi de programmation de justice et son volet organique au Sénat à la fin du mois de mai, elle sera une nouvelle étape du travail conjoint est constant que nous avons conduit depuis plusieurs années ensemble chancelleries et Sénat. Je vais en particulier monsieur le sénateur, je veux également rendre hommage à toute la commission des lois et à son président François Noël Buffet nous ferons tout cela. Pour renforcer les moyens dont notre justice a tellement besoin. Et donner la parole à notre collègue David Assouline pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Merci monsieur le président. Madame, la Première ministre, comme vous le savez, il y a une énorme attente du débat qui va commencer ici demain. Et ce d'autant plus que celui à l'Assemblée nationale. Qui n'a même pas été jusqu'au principal article a offert un spectacle parfois désolant. Pourtant, quand il a eu lieu, il a été éclairant sur les femmes qui, contrairement à vos affirmations sont les principales victimes de votre texte mais aussi quand vous nous parliez des prétendus 1,8 million de concernés par une retraite minimum à 1200 euros. Devenu 40.000 et finalement de 10 à 20.000 au Sénat. Nous la gauche, nous allons poursuivre ce travail de vérité, nous serons en écho avec une très grande majorité de nos concitoyens et avec des syndicats unis qui appelle à ce que notre pays s'arrête le 7 mars pour dire non à cette régression sociale nous débattrons cet article 7 qui est un impôt sur la vie des plus modestes et chacune et chacun ici devra prendre ses responsabilités. Par son vote pour ou contre 2 ans de plus pour celles et ceux qui ont déjà travaillé dur toute leur vie. Mais nous sommes ici attachée au débat de fond et le fond, comme la démocratie demande du temps, celui de l'argumentation et de l'écoute, celui de l'amendement et de l'explication de vote libre pour chacun qui sont des droits sacrés des parlementaires. Alors je vous le demande, allez-vous encore empêcher ce débat en le brutalisant en le menaçant d'interruption alors qu'il s'agit d'une loi qui touche à la vie de millions de nos concitoyens. Faute d'avoir recherché un accord acceptable avec les syndicats. Est-ce que cette limitation fait partie de l'accord des droites. Que vous auquel vous avez consacré tant d'énergie. Que vous avez négocié avec LR au Sénat pour faire passer, c'est un très fort injuste et inutile. et inutile. La parole est au ministre du Travail, du plein emploi, de l'insertion. Monsieur Olivier Dussopt. Vous avez la parole. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Assouline. Permettez-moi de vous répondre en 3 points. D'abord sur les conditions et la durée du débat. Le le gouvernement bien évidemment espère que le débat qui s'ouvre demain au Sénat, permettra d'examiner de débattre de discuter de chacune des dispositions du projet de loi et ainsi d'avoir un débat éclairé sur la totalité des articles la totalité des dispositions et la totalité du projet. Vous dites. À raison d'une certaine manière que le débat à l'Assemblée nationale n'a pas pu aller au bout. Mais ce n'est pas au gouvernement qu'il faut en faire le reproche. C'est à vos alliés se sont à vos alliés de la France insoumise qui avait que 18.000 amendements parfois quelques outrances ne nous qui n'ont pas permis d'aller au bout. Vous dites monsieur le sénateur. Qu'il veut qui que ce débat sera pour vous l'occasion de pointer des vérités. Permettez-moi d'en rappeler une et de confirmer un chiffre que vous avez donné avec cette réforme de retraites, nous prévoyons une pension minimale pour les assurés qui ont cotisé toute leur carrière au niveau du SMIC et je vous confirme de chiffres hein que vous avez cité grâce à cette pension parmi les 17 millions de retraités que compte aujourd'hui notre pays 1.800.000 bénéficieront d'une revalorisation et la moitié d'entre eux auront une revalorisation entre 70 et 100 euros. Peut-être que vous ne trouvez que c'est pas assez mais ça signifie si vous ne pouvez pas assez sympa ça je la passer si vous êtes assez déconnecté du niveau des petites pensions et de l'importance de la revalorisation Et puis cette réforme, elle va permettre à un nouveau retraité sur 4 200.000 parents d'avoir là aussi une pension meilleure avec la perspective puisque c'est notre objectif de garantir 85% du SMIC pour une carrière complète payés au niveau du SMIC. Enfin, monsieur le sénateur, vous dites, chacun devra prendre ses responsabilités. C'est une réalité. Nous travaillons avec tous les groupes qui le souhaitent et si nous pouvons avancer sur les droits familiaux avec la majorité sénatoriale, j'en serai le premier heureux mais prendre ses responsabilités c'est aussi assumer les positions de votre famille politique, j'ai entendu votre chef de parti monsieur Faure défendent la retraite à 60 ans avec 43 annuités. C'est une machine à des côtes, c'est une machine à pauvreté et c'est une machine à petites pensions.

ma question s'adresse à Madame la Ministre chargé des collectivités territoriales et de la ruralité. La France a a subit une sécheresse météorologique préoccupante avertissait mardi dernier météo France en confirmant que le pays venait de vivres 31 jours consécutifs sans pluie. Samedi matin, le président de la République a appelé les agriculteurs à la sobriété sur l'eau en plein coeur du salon de l'agriculture à Paris dans le bassin Adour-Garonne et qui couvre une grande partie du Sud-Ouest, le département des Hautes-Pyrénées, est un véritable château d'eau assurant l'irrigation des Terres jusque dans les Landes en traversant le Gers. Mais jusqu'à quand. Car on constate, année après année la baisse des nappes phréatiques. On va même jusqu'à manquer d'eau dans quelques villages de montagne riche pourtant de leur réseau hydrographique et c'est plus qu'inquiétant. Madame la Ministre. Je sais que vous prenez la mesure de l'ampleur de ce phénomène mais aujourd'hui nos agriculteurs et nous-mêmes. Nous avons besoin de réponses, car on ne peut pas uniquement imposer des mesures de restriction sans véritable politiques et ambitions quelle stratégie comptez-vous mettre en oeuvre pour accompagner notre agriculture dans cette adaptation indispensable face à la sécheresse. Quelles solutions au delà des économies d'eau nécessaires à leur apporterez-vous et que comptez-vous faire pour soutenir et faciliter la création de nouvelles réserves essentielles à la survie sur nos systèmes hydrographique pour nos besoins quotidiens. Ah non potable pour l'amène le maintien de la qualité des milieux et en terme de salubrité publique. D'une part et pour la préservation de notre agriculture garante de notre souveraineté alimentaire, d'autre part, je vous remercie. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Carrère. Je tiens tout d'abord excuser Christophe Béchu qui est actuellement au Gabon. Dans le cadre du One Forest mythe au sommet pour favoriser la préservation des forêts tropicales. La France métropolitaine connaît aujourd'hui vous l'avez dit, une sécheresse météorologique préoccupante cinq départements font déjà l'objet de restrictions les Pyrénées Orientales, le Var, l'Isère, l'Ain et les Bouches-du-Rhône. Dans les jours qui viennent d'autres départements feront l'objet d'arrêtés de restriction pris par les préfets. Le niveau de précipitations dans les 2 mois qui viennent, sera crucial pour déterminer la situation dans laquelle nous serons cet été. Le gouvernement en lien avec les opérateurs de l'État chargé du suivi hydrologique. Comme météo France, par exemple, suit avec attention l'évolution de la situation et les projections nous devons ensemble, État et collectivités territoriales, poursuivre notre travail d'anticipation et prendre dès maintenant si nécessaire des décisions de partage de l'eau. Le mot d'ordre et la sobriété des usages. Nous sommes tous concernés et tous les secteurs d'activité sont concernés. Concernant l'agriculture, il faut le rappeler sans eau. Il n'y a pas d'agriculture et sans agriculture. On ne se nourrit pas. Il faut donc réussir à trouver des compromis et discuter ensemble pour trouver des solutions avec Christophe Béchu. Nous sommes pleinement mobilisés les préfets qui coordonnent les sept grands bassins du pays ont été réunis le 27 février pour planifier les solutions liées aux problèmes de raréfaction d'eau auxquels nos territoires seront confrontés. La prochaine réunion aura lieu le 6 mars. À la demande de la Première ministre une cellule interministérielle de crise ouvrira au mois de mars. Enfin le plan sur l'eau, sur lequel nous travaillons depuis six mois, sera présenté dans les prochaines semaines suite au chantier sur la planification écologique sur l'eau. Il se penchera sur les questions de sobriété et de répartition des usages, notamment en matière d'agriculture. Merci madame. Si Madame Merci, madame la Ministre, malheureusement on ne pourra pas uniquement passer sur la sobriété et les efforts d'économies les déficits sont déjà trop important sur les bassins hydrographiques. Nous avons réellement besoin de stratégie. Et qu'en est-il aujourd'hui par exemple du du des propositions du Varenne, de l'eau qu'il y a eu il y a quelques années. de la simplification de l'accompagnement pour de nouvelles réserves. Merci. Merci monsieur le président. Ma question s'adresse aux minutes veulerie, culture. Alors Monsieur le Ministre. L'agriculture biologique traverse actuellement une très mauvaise passe. Une chute inédite de 4% de la vente. Faisant suite à des années de croissance à 2 chiffres. Madame, la Première ministre. Vous avez évoqué une aide de soutien à la filière via un fonds, un fonds d'urgence doté de 10 millions d'euros. Les acteurs concernés ont rapidement fait le calcul, 166 166 euros en moyenne par ferme juste le prix d'une paire de bottes pour aller Auchan. Monsieur le Ministre de l'Agriculture a déclaré que la bio. Ne souffrait pas seulement d'un manque de soutien mais d'un problème de demande. Alors quand la filière porc conventionnelle a connu en 2022 une crise de la demande à l'export. C'est un plan de sauf de sauvegarde doté de 270 millions d'euros qui a été mise en place et 15.000 euros d'aides directes en soutien à la trésorerie des exploitations porcines, le soutien à la demande. C'est aussi la communication quand de 20 millions d'euros permettent la communication en faveur des produits laitiers conventionnelle. L'Agence Bio doit faire avec 750.000 euros. Et quand on parle aussi de demandes en bio, rappelons la responsabilité de l'État pour permettre le respect des 20% bio dans la restauration collective, on est loin du compte. Et quant au chèque alimentation durable. Il a disparu de l'actualité. Alors Monsieur le Ministre, allez-vous enfin mettre en oeuvre un réel plan de soutien à l'agriculture biologique comme le demande l'ensemble de la profession agricole et aujourd'hui l'ensemble des syndicats agricoles. On vous réponde. La parole était monsieur Olivier Véran. Un porte-parole du gouvernement, n'en prenne ombrage Marc Fesneau, ministre en charge de l'agriculture et chacun peut le comprendre, actuellement au Salon international de l'agricole. Il m'a donc délégué la lourde tâche de représenter ce que je vais tâcher de faire de mon mieux. Nous avons conscience. Monsieur le sénateur, de que la toute la filière du bio traverse actuellement une crise, vous l'avez dit et c'est notamment une crise de la demande et c'est sur ce levier en particulier que nous voulons et devons agir. nous avons mis en place de nombreuses mesures pour soutenir déjà la production bio et encourager la consommation il y a et qu'au régime. Le crédit d'impôt, la participation de l'État au financement d'une nouvelle campagne bio réflexe à hauteur de 750.000 euros. Vous l'avez dit, comme nous l'avions fait en 2022, il y aura également une campagne assurée via le plan France 2030, à hauteur de 3 millions d'euros. Monsieur le sénateur. Nous avons également abonder le Fonds Avenir Bio de 15 millions au lieu des 8 initialement prévus dont 2 pour structurer la filière porc bio qui connaît des difficultés particulières. Lors des Assises de la bio. Le 6 décembre dernier, le ministre de l'Agriculture a demandé à l'Agence Bio d'engager un travail de structuration de la filière la consommation en restauration collective sera elle stimuler grâce à la campagne de communication que l'agence va lancer dès 2023 avec le financement du programme de promotion européen qu'elle a obtenu en 2022. Nous avons ouvert la possibilité aux régions qui le souhaitent d'heure exploiter des crédits fédère non utilisées. Le futur programme Ambition bio sera aussi l'occasion de construire une véritable filière renouvelé dans sa stratégie pour l'accompagnement et la structuration et puis pour apporter des réponses conjoncturelles, face à la situation actuelle du marché. La Première ministre a annoncé l'ouverture d'un fonds d'urgence doté doté de 10 millions d'euros qui va soutenir des exploitants des exploitations bio qui sont en difficulté immédiates, nous avons entendu la demande de la filière sur un risque que des exploitations bio s'écroule. L'État les soutiendra avec une aide de trésorerie qui sera versé dans les semaines qui viennent, nous encouragerons activement tous les acteurs, notamment la grande distribution, les collectivités locales à faire la promotion du bio sous la bannière du réflexe dès ce printemps et une réponse structurelle et pour autant nécessaire et il y aura donc. Des réponses qui seront apportées très prochainement je complèterait ma réponse tout à l'heure, il y a une autre question sur le Monsieur laver. Oui, Monsieur le Ministre ce vote vous donner quelques réponses, mais sur le Global c'est absolument insatisfaisant je voudrais ici insister sur l'avenir durable que représente l'agriculture biologique au regard des enjeux actuels, la préservation de la qualité de l'eau en qualité, mais aussi en quantité la la qualité du sol, la qualité de l'air, la préservation de l'environnement de la biodiversité des pollinisateurs la préservation aussi de la santé humaine. Alors toutes ces raisons font qu'on se doit de donner de véritables moyens à l'agriculture biologique pour qu'elle se développe. Merci. Merci. La parole est à notre collègue Pierre mais de miel pour le groupe les indépendants République et Territoires. En matière de produits phyto-Ford phytosanitaires nous respecterons désormais le cadre européen, et rien que le cadre européen. Tels sont les propos de la Première ministre lundi au salon de l'agriculture largement saluée par la profession. Nos agriculteurs ont besoin d'un cadre commun cohérent et réaliste au niveau européen sur les produits phytosanitaires. Stop aux technocrates qui veulent laver plus Vert que Vert. Nos agriculteurs ont surtout besoin que le cadre français ne soit pas la succession de sur-transpositions Made in France mortifère. Nous nous plaignons depuis des années de la pénalisation nos agriculteurs par rapport à leurs collègues européens. Il y a eu des progrès mais restons vigilants. L'agriculture est à la croisée des chemins. Face à des nécessités majeur et particulièrement la préservation de notre environnement de nos sols et d'autres biodiversité. L'équation plus de chaleur moins d'eau, plus d'aléas climatiques. Moins de phyto-. Tout en gardant le niveau de production suffisant est extrêmement compliqué à résoudre. Si rien n'est impossible. Nous allons devoir une agriculture de demain. Basée sur l'innovation, la technologie, la recherche et de formation. La liste des besoins longue mais en priorité. Je vois l'optimisation de leurs sources. Ah non bien sûr, l'utilisation de plan de nouvelle génération, l'accélération des délais d'obtention de l'autorisation de mise sur le marché de nouvelles maculent prometteuse. La profession se réjouit des annonces de nouveau plan Ecophyto 2030 qui doit aider à uniformiser les techniques agricoles au niveau européen et nous permettre d'être cohérent sur les marchés mondiaux. Comment pensez-vous que l'État peut accompagner concrètement la profession dans ce virage historique pour culture. Pour vous répondre. La parole est que le porte-parole du gouvernement, monsieur Olivier Véran. vous le savez, nous sommes confrontés à une réduction importante du nombre de substances actives au niveau européen et c'est un mouvement, on peut se le dire qu'il n'est pas terminé, loin s'en faut. C'est un sujet de souveraineté alimentaire et de transition écologique. Et c'est à travers la logique de planification que nous entendons concilier ces 2 impératifs. C'est dans cet esprit que la Première ministre a annoncé au salon de l'agriculture, élaboration d'un plan d'action stratégique pour renforcer le pilotage et l'adaptation des techniques de protection des cultures. Dans ce plan Ecophyto 2030. Nous devons assumer collectivement que le développement des alternatives est essentielle, y compris les alternatives non chimiques la voie à suivre. Elle passe nécessairement par plus d'agronomie, la mobilisation non pas d'un levier mais de plusieurs leviers et le renouvellement des pratiques agricoles et des systèmes de production. Cela passe aussi par des moyens importants pour accompagner les agriculteurs et massifier les solutions. C'est dans cet esprit que le ministre-travaille avec l'ambition que nous puissions collectivement de s'inscrire dans une nouvelle approche. D'abord avoir une stratégie de ne plus être sur une gestion au coup par coup ne plus être en réaction mais bien en anticipation, c'est ça qu'on appelle la planification ça passe notamment par une grande plus grande visibilité sur l'évolution des solutions en terme de protection des cultures. On veut aussi avancer avec les professionnels avec les filières avec les instituts techniques et de recherche. Faire en sorte que ce qui peut apparaître comme une impasse deviennent au fond une opportunité et donc il faut être et travailler étroitement ensemble, mobiliser nos capacités de recherche et de développement. L'État fera sa part bien sûr mais il faut aussi mobiliser les centres techniques des filières et les chambres d'agriculture. Troisièmement, on veut avoir une approche globale et donc ne pas négliger ce qui permet d'optimiser l'utilisation des produits phytosanitaires. Il y a sur ce point des innovations qui doivent être déployés le plus largement possible. Enfin on veut pouvoir s'appuyer sur ce qui a fonctionné élargir le travail fait dans le secteur des fruits et légumes comme exemple de notre méthode de planification écologique à l'ensemble des filières dans une approche mobilisatrice transversales et qu'on pourra décliner opérationnellement filière par filière.

de confiance et qu'on arrête les tabous sur une agriculture productiviste, parce que nous avons une besoin d'une agriculture qui produisait. La parole est à. Notre collègue Max Brisson. Pour le groupe Les Républicains. Maxime ce président, Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale. Mercredi dernier. Vous avez partagé l'émotion des élèves et des professeurs du lycée c'est au mois d'Aquin de Saint-Jean-de-Luz. Je vous en remercie. Ce drame absolu, n'a pas grand chose à voir avec la violence qui gangrène nos collèges et de lycées ou la difficile détection des situations de détresse des adolescents. De ces sujets nous reparlerons quand l'émotion sera passée. Pour l'heure, je voudrais vous narrer l'histoire d'un inspecteur d'académie venu dans un petit village de France, calculer le nombre d'élèves attendus pour la prochaine rentrée par la fenêtre d'école plusieurs maisons en construction doit accueillir dans 2 ou 3 ans. Des familles avec enfants. Mais ce qui se passera dans 2 ou 3 ans n'intéresse pas monsieur l'inspecteur d'académie l'école à la prochaine rentrée perdra 3 élèves, 3 élèves en moins, un professeur en moins une classe qui ferme télé le verdict de ce rituel immuable qui sont bons, la IVe République. La carte scolaire rituel qui conduit chaque année, les inspecteurs d'académie de France et de Navarre à sortir le règle à calcul pour compter les élèves et décider du sort des postes et des classes. Et pendant ce temps, l'État demande aux élus d'Esquire leur politique d'urbanisme dans les. Scott. Lui ou PLU imposant au maire de voir loin. Monsieur le Ministre, jusqu'à quand. Resterez-vous le seul de vos collègues qui adapte chaque année les postes au comptage à l'unité près de ses usagers. Monsieur le Ministre, à quand une procédure pluri-annuel de la carte scolaire adapté à notre époque. Monsieur le Ministre, au ministère de l'Éducation nationale. L'entrée dans la modernité, c'est pour quand. merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs le les sénateurs, monsieur le sénateur, Max Brisson. Je m'associe bien sûr l'hommage que vous venez de rendre. À Agnès Lassalle assassiné dans l'exercice de ses fonctions. Elle consacrait sa vie à ses élèves. Et mes pensées vont à sa famille, à ses collègues et à ses élèves. Toute atteinte contre un professeur porte atteinte à la République. C'est ce que j'ai dit sur place avec Stanislas Guerini, le ministre de la fonction publique avec vous-. Même avec la sénatrice Espagnac il avec le maire de Saint-Jean-de-Luz, Jean-François Hirigoyen. À propos de votre question, la carte scolaire. Tient compte bien sûr d'une manière générale de la baisse des effectifs scolaires qui sera j'ai eu l'occasion de le dire, dans cet hémicycle très importante. L'année prochaine, ce qui nous amène à fermer des classes ici à en ouvrir là dans votre département des Pyrénées-Atlantiques nous compterons environ 450 élèves de moins. L'année prochaine tout en veillant à ce que le taux d'encadrement particulièrement dans les régions rurales continue de s'améliorer, ce qui sera en effet le cas dans votre département des ajustements d'ici au mois de juin vont avoir lieu, en particulier sur quelques points sensibles. Éventuellement ce que vous connaissez tout en donnant priorité au RPI les regroupements pédagogiques intercommunaux donc aux zones rurales. À propos de pluri-annuel. Nous avons un regard pluri-annuel sur les évolutions démographiques qui nous est fournie par les statistiques. Du ministère de l'Éducation nationale ainsi que par les. Rectorats mais il faut aussi tenir compte des variations annuelles des migrations des familles qui s'installe des déménagements, ce qui oblige effectivement à construire annuellement une carte scolaire mais nous. Encore au stade des ajustements. Je vous remercie. Je vous ai parlé de procédure de la carte scolaire, je crois qu'il est grand temps que l'on travaille avec les assistants d'élus pour rentrer dans une démarche pluriannuelle les maires n'en peuvent plus d'avoir un comptable chaque année dans leurs écoles qui viennent calculer le nombre d'élèves alors qu'ils savent comme lotissement est en cours cours de préparation et que dans un an, dans 2 ans il y aura à nouveau des enfants c'est cette vision comptable qu'on vous demande d'abandonner pour une démarche pluriannuelle. La parole est à notre collègue Jean Michel Arnaud pour le groupe de l'Union centriste. Remercie monsieur le président, mes chers collègues. Alors que l'agriculture biologique a longtemps été favorisée par les pouvoirs publics au nom de l'impératif écologique. Elle est aujourd'hui à la marge des priorités gouvernementales. Le plan national stratégique dans le cas de la PAC supprime l'aide aux agriculteurs bio. L'Agence Bio et sous-financé et les dispositifs de soutien sont très insuffisants depuis quelques décennies, les pouvoirs publics promettait un soutien massif aux pratiques vertueuses une souveraineté alimentaire accrue de meilleurs débouchés pour nos agriculteurs. Quelle est la situation réelle aujourd'hui les modes de production sobre en énergie et respectueux de la biodiversité sont peu reconnus et nous constatons une baisse des ventes des produits bio, notamment depuis la crise sanitaire. Le contexte économique ne conforte en aucun cas, les conditions de travail de ce qui nous nourrissent hausse insupportable des coûts de production freinage des exportations signature de traités de libre-échange quand le Mercosur souvent synonyme de concurrence déloyale. Le marché bio est en situation de surproduction avec une demande toujours plus morose au regard de la de l'inflation actuelle. Ce déclin comme un ver dans la pomme, il ne faut pas laisser pourrir la situation. Que compte faire le gouvernement aujourd'hui pour contrer cette situation difficile est particulièrement difficile pour les 60.000 exploitants agricoles bio de ce pays merci. Pour vous répondre la parole être. Ministre porte-parole du gouvernement, monsieur Olivier Véran. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur Jean Michel Arnaud, j'ai, j'ai répondu tout à l'heure déjà à votre collègue sur sur le bio peut être commencer par dire qu'. On aime le bio on a besoin de nourrir l'ensemble des Françaises et des Français et on a aussi besoin de développer notre filière bio pour la consommation nationale et aussi pour l'export un des leviers. Je vais peut-être m'arrêter davantage sur celui-ci dans ma réponse, c'est la restauration collective. Pourquoi je dis ça parce que on a un objectif dans la loi Egalim. Vous le connaissez qui est 50% de produits de qualité et durable dans la restauration collective, dont 20% de bio, c'est un levier qui est majeure, et que nous souhaitons améliorer très fortement qu'il s'agisse des écoles, des collèges et lycées mais aussi des Ehpads et des entreprises, c'est aussi une manière de changer durablement les pratiques de consommation alimentaire que d'introduire massivement le bio dans ses restaurations collectives. Alors il se trouve que depuis 2018 on a fait face à plusieurs événements plusieurs vents contraires. D'abord la crise du Covid. Évidemment puisque la restauration collective a perdu transitoirement 40% de son chiffre d'affaires du fait des mesures sanitaires mais aussi actuellement le contexte d'inflation que nous connaissons depuis plusieurs mois, qui rend difficile un bilan précis depuis cette année mais on voit que les gestionnaires de restaurants collectifs doivent renseigner leurs résultats Egalim sur la plateforme ma cantine ça va nous permet de disposer prochainement de données plus détaillées qui seront naturellement communiqué au Parlement. Il y aura aussi besoin d'accompagner la filière car améliorer, améliorer la qualité des repas en restauration collective, ça passe aussi par la lutte contre le gaspillage alimentaire. Une réflexion sur les quantités qui sont servis ou encore les recettes utilisées. La Première ministre a pris une circulaire le 29 septembre dernier qui permet également d'aider tous les établissements publics à renégocier leur contrat et donc à acheter au juste prix. Il y a une réflexion qui est en cours avec les différents ministres concernés afin de rechercher des dispositifs adaptés à chaque segments de la filière de restauration collective. Atteindre l'objectif Egalim nous le voulons, ça représentera un potentiel d'augmentation d'environ 10% du chiffre d'affaires de la filière, ça viendra plus que compensé les baisses en vente bio constaté pour l'année 2022. Oui, Monsieur le Ministre, je crois qu'il nous faut une vraie politique de promotion de la filière bio et de soutien en faveur de cette agriculture biologique clarifier les labels actuellement existants ou encore inclure systématiquement comme vous l'avez rappelé, l'agriculture biologique dans les projets alimentaires. la souveraineté alimentaire doit aussi passer par une meilleure attractivité du métier d'agriculteur et je pense à cet instant particulièrement aux arboriculteurs alors que le groupe Carrefour met en tête de gondole des pommes polonaises. Nous avons culture ne s'en sortent pas, il leur manque 20 centimes de marge des marches qui effectivement ne sont pas aujourd'hui payer à la hauteur des coûts de production. L'agriculture biologique comme celle conventionnelles sont confrontés aussi à l'impossibilité de lutter contres les espèces invasives alors que nombre de traitements sont homologués au niveau européen la France par le biais de Lanxess maintiennent l'interdiction générale de plusieurs traitements y compris bio qui se cantonne à des dérogations successives en envoyant un message négatif aux clients, comme je l'ai sous-entendu dans les travées du du du salon international de l'agriculture il y a quelques heures maintenant en France, nous avons trop souvent le droit de manger ce que nous n'avons pas le droit de produire. La parole est à notre collègue Éric. Pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. Merci monsieur le président, madame, la Première ministre, mesdames et messieurs les ministres. Mes chers collègues, ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Agriculture, mais je sais monsieur Véran que c'est vous, aujourd'hui qui avait chaussé les bottes. L'association Terre de Liens publié hier un rapport très intéressant sur la propriété des surfaces des Terres ça agricole en France. En pleine semaine du salon de l'agriculture les constats présentés sont de nature à générer de grandes inquiétudes pour l'avenir de notre agriculture. Il y a en France 496.000 chefs d'exploitation agricole. Mais seuls 35% des Terres cultivées appartiennent aux agriculteurs. Le rapport présente un phénomène nouveau, on voit se développer des sociétés agricoles, dont certaines sont financiarisé celle-ci possédait 7% de la surface agricole il y a 20 ans ce chiffre atteint aujourd'hui 14%. On découvre ainsi que de grands groupes comme Auchan Chanel ou L'Oréal achètent des Terres agricoles. Les capacités de l'innovation financière sont décidément illimité, nous le savions, nous connaissions la finance des villes nous découvrons aujourd'hui la finance des champs. Ces sociétés possèdent aujourd'hui que 640.000 hectares ces pratiques font flamber le prix à l'hectare rendant par conséquent difficile l'accès de petits agriculteurs other et favorisant aussi les exploitations de très grande taille. Au cours des 40 dernières années 2 enquêtes statistiques pour étudier la structure de la propriété de Terres agricoles ont été menées par le service statistique du ministère de l'agriculture. Or depuis 30 ans. Le ministère ne recueille presque plus aucune donnée, Monsieur le Ministre. Ma question est double, tout d'abord n'est-il pas temps de procéder à un audit complet afin de prendre la mesure de ce phénomène nouveau. Et deuxièmement, nous pensons qu'il y a urgence à renforcer la régulation foncière agricole la future loi d'orientation agricole ne devrait-elle pas être l'occasion d'en lancer le chantier. Merci. Pour vous répondre. La parole est. Le ministre porte-parole du gouvernement, monsieur Véran. Monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur. Éric Bocquet. Vous m'interrogez sur la financiarisation des Terres agricoles et vous avez raison. Il y a de la concurrence sur l'usage du foncier et la préservation des Terres agricoles, c'est une priorité pour le gouvernement partageait donc. C'est un sujet de souveraineté agricole et de souveraineté alimentaire. il y a des outils de régulation qui ont été mis en oeuvre dans l'après-guerre le contrôle des structures les actions des affaires, le statut du fermage ont bénéficié ainsi en France du prix du foncier parmi les moins chers d'Europe. cela permet de maintenir la diversité des modèles. C'est un élément essentiel. Par ailleurs 2 avancées législatives importantes ont été réalisées cette fois-ci, lors de la précédente législature. C'est un peu plus récent et vous les connaissez, d'abord la zéro artificialisation nette sur lequel le Sénat est très engagé. Avec la disposition qui prévoit que les documents de planification régionale intègre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols. La mise en oeuvre également d'un contrôle renforcé des opérations sociétaire issu de la loi du 23 décembre 2001 dite la loi Sempastous. À instaure un dispositif d'autorisations administratives préalables en cas de cession de titres sociaux uniquement si l'opération confère le contrôle de la société cessionnaire et lorsque les surfaces ainsi contrôler dépasse un seuil d'agrandissement significatif, enfin vous le savez, nous avons lancé une grande concertation sur le pacte et la loi d'orientation. Et d'avenir agricole. L'objectif, nous voulons installer des agriculteurs en leur donnant les moyens de s'adapter aux conditions climatiques techniques et économiques de demain. Et question de foncier seront évoqués à cette occasion, comme vous le savez ou vous venez de l'appeler de vos voeux. Il s'agit pas que de leviers législatifs. Nous devons construire cela bien sûr avec les élus locaux et notre objectif commun, c'est donc de pouvoir agir rapidement avec des soucis opérationnel. Oui, monsieur le Ministre, je pense qu'il y a véritablement urgence à cette problématique, une ferme sur 10 est aujourd'hui une société financiarisé et je souhaiterais en conclusion, la première phrase du rapport de Terre de Liens je cite le jour où nos ancêtre s'ont fait de la terre une marchandise est un jour noir pour l'humanité. Merci la parole est à d'autres collègues Laurent Somon pour le groupe Les Républicains. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, on achète des oeufs venus de l'étranger pendu dans les cages, que nous avons vendu des cerises parce qu'on a arraché les cerisiers et bientôt pommier et noisetiers on va acheter le poisson déchargé de bateau battant pavillon étranger parce qu'on a détruit, on détruit notre flotte alors qu'on se targue d'avoir le 2ème domaine maritime mondial déjà les fruits et légumes, faute de main d'oeuvre peut être les endives laisser en terre faute à une énergie trop chère qu'on brade aux concurrents d'EDF le sucre ou les lentilles malgré le plan protéines importés de pays où sont autorisés des traitements interdits ici. Ajoutez à cela l'angoisse de règlements des contrôles des injonctions contradictoires des charges administratives et l'incertitude des revenus soumis aux négociations annuelles. Vous voyez le conte de fées ne fait pas rêver la profession agricole qui s'interroge sur la place réelle et l'avenir que vous lui réservez la ferme de France exposés à ces vents contraires s'expose cette semaine en lettres capitales pour proclamer la qualité des productions et l'engagement des hommes et des femmes pour des produits respectueux des exigences sanitaires et durable protéger les consommateurs et notre environnement. Croyez-vous que les agriculteurs refusent de mettre des 6 pourrait prendre plus de nitrates dont les coûts ont plus que triplé. Croyez-vous que les agriculteurs ou les industriels ont attendu les déclarations du président parlant de l'eau sur la fin de l'abondance pour l'économiser, alors que les entreprises comme Cristal-Union Union dans la Somme. Même des betteraves pour leur cycle de production de sucre et ne puisse rien dans les nappes pour gagner en compétitivité et répondre aux exigences environnementales. L'agriculture est soumise à la nature et en fait vous résigner le choix de son déclin ou d'une agriculture vitrifié et d'importation ou in vitro peut être la ferme France a a besoin de connaître le cap pour qu'elle adapte son évolution dépendant de la recherche technique génétique les moyens alloués et le pas de temps nécessaire ce pendant ce temps politique, c'est maintenant Monsieur le Ministre, quelle est votre ambition. Pour vous répondre. La parole est que le porte-parole du gouvernement de monsieur Véran. Oui, monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Laurence au monde. Alors d'abord je peux vous dire, pour le coup, a-t-il personnelle que je partage le constat que vous avez fait de dire que les agriculteurs ne nous ont pas attendus pour identifier des solutions. Il se trouve par exemple que vous citez l'entreprise Cristal Union d'usine de betteraves qui est capable de recycler totalement eau figurez-vous que je suis allée voir sur place dans l'usine pour constater avec eux qui avaient déjà mis la charrue avant les boeufs. Mais dans le bon sens du terme, puisqu'ils ont réduit énormément leur consommation énergétique et quasiment arrêté la consommation d'eau, ce qui veut dire que c'est possible mais ce que nous devons faire nous comme État. C'est ce qu'il a pas d'abord de colliger ces bonnes pratiques de les enregistrer de les reconnaît de les soutenir, mais aussi être capable d'essaimer dans l'ensemble des entreprises du secteur agricole et sur l'ensemble du territoire national. C'est ça qu'on appelle restaurer la compétitivité. La ferme France c'est aussi partir de ce qui fonctionne sur le terrain de l'exemple qui nous montré par celles et ceux qui aiment profondément la terre cultiver et nourrir les Français. que c'est vraiment notre ambition. Alors il y a un rapport du Sénat qui montrait que depuis 1990 il y avait eu un effritement progressif de la compétitivité de la ferme France et c'est pour ça qu'on veut vraiment identifier des solutions depuis 2017 il y a eu des choses qui ont été faites, on a mis, par exemple, le revenu agricole au coeur de notre politique je pense à la loi Egalim de que vous avez voté. Merci pour cela, pour que le juste prix ce soit plus seulement le prix bas mais c'est tout simplement celui qui permet à nos agriculteurs de vivre. C'est une vraie rupture avec la loi LME précédente et vous aurez prochainement l'occasion d'assurer la prolongation du SRP plus 10 qui est un des leviers d'Egalim. C'est également pour cela que nous avons initié des transitions ambitieuse avec le Varenne, de l'eau c'est important de pouvoir regrouper tout le monde, encore une fois de discuter ensemble et d'identifier des bonnes solutions. Je pense aussi à la réforme de l'assurance-récolte ou le travail mené sur la réutilisation des eaux usées. Parce que les agriculteurs qui sont bien souvent les premières victimes le savent parfaitement. L'adaptation au changement climatique, la souveraineté alimentaire c'est un même combat, c'est cela que nous appelons la logique de la planification écologique et ça va rejoindre à la logique de la planification agricole et c'est un projet porté à bras le corps par le ministre en charge de l'agriculture évidemment par la Première ministre. Monsieur le ministre, en 20 ans la France a vu son industrie décliner nous apportons désormais voiture médicaments jusqu'à notre électricité demain si vous ne remettait pas en cause vos choix nous perdrons nos agriculteurs les vocations et notre souveraineté alimentaire. Nous avons laissé notre industrie décliné, n'en faisons pas de même avec notre équipe à notre agriculture redonner confiance à nos agriculteurs que nous n'ayons pas à répéter au président ce que Fénelon écrivait en 1694 à Louis XIV. La France est devenue un grand hôpital désolé et sans provision.

Merci monsieur le président. Monsieur le Ministre. Hier, puissance agricole et 2ème exportatrice mondiale de produits agroalimentaires. La France est passée au 5ème rang en 20 ans ces importations ont suivi le sens inverse et représentent aujourd'hui près de la moitié des produits consommés par les Français. Chaque jour, nous ne sommes plus le grenier de l'Europe, nous sommes déficitaires en matière alimentaire depuis 2015, le nombre d'exploitations ne cesse de diminuer, tout comme les cheptels, et l'on observe un taux inquiétant de des conversions dans l'agriculture biologique. Après 5h et demi d'action gouvernementale, les situations, les agriculteurs ne s'est pas améliorée, loin de là. Le taux de suicide chez les exploitants agricoles et le plus élevé de toutes les catégories socioprofessionnelles. La transmission des exploitations reste un problème majeur en 25 ans le prix des Terres agricoles aura doublé dans 10 ans, 50% des chefs d'exploitation seront en droit de partir à la retraite la profonde crise des vocations s'explique avant tout par l'absence de revenu décent et par le coût de plus en plus élevé du foncier agricole. La proposition de loi pour lutter contre l'accaparement du foncier agricole déposée par votre majorité avant les présidentielles de 2022 n'a répondu en rien à la problématique de concentration du foncier et des outils de production à l'heure actuelle, l'État démontre manque total d'ambition. Or les crises se succèdent et vont se multiplier, très rapidement. Entré à quel point notre agriculture était fragile. La France est déjà depuis un mois en situation de sécheresse le véritable modèle agricole français que nous voulons déforme doit être pérenne familial respectueux des humains des animaux et des sols et c'est celui qu'il faut préserver à tout prix nos territoires et nos citoyens ont besoin de la polyculture élevage de la multiplication des circuits courts des relocalisations avec des chaînes d'approvisionnement alimentaire sur non soumise aux aléas climatiques. Et géopolitique préserver notre souveraineté et notre sécurité alimentaire, est un gage d'indépendance et de survie. À cet égard les intentions de l'État quant à la ratification des accords UE-Mercosur du CETA de l'Accord libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Autant de porte ouverte à une concurrence déloyale ne sont toujours pas claires, Monsieur le Ministre, nous avons besoin d'une trajectoire d'adaptation précise et cohérente face à tous ces enjeux et le temps presse. Quand allez-vous proposer une véritable politique agricole. Oui, monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, Monsieur le le sénateur Christian Rey dans sa Razi. Je vous écoute, on peut être. Que d'accord sur le constat que vous faites, vous avez raison de rappeler que d'ici une dizaine d'années près de la moitié des agriculteurs sera parti à la retraite et qu'il nous faut absolument rentrer dans une logique de renouvellement des générations. Vous avez raison aussi de souligner qu'il faut profiter de ce renouvellement des générations. Ça avait été le cas d'ailleurs dans les années, dans les années 60 lorsqu'il avait eu une, une planification agricole avec déjà un grand renouvellement générationnel dans le monde agricole. Il faut pouvoir accompagner les transitions c'est-à-dire à voir répondre à la demande des jeunes agriculteurs qui sont des gens qui aiment la terre qui aime cultiver qui veulent être propriétaires de leurs moyens de production et qui veulent pouvoir vivre de leur travail décemment ainsi la question du revenu est une question qui compte. Elle est pas unique mais c'est une question qui est central avec les loi Egalim hein. Et de nous avons mis fin à la spirale déflationniste et la destruction de valeur pour nos agriculteurs, ce sont des lois récentes nous devons travailler à leur pleine application au-delà, nous devons surtout assumer un discours clair, collectivement, nous voulons une alimentation saine, sûre, durable, respectueuse de l'environnement et de la biodiversité. Hé oui, monsieur le sénateur tout ça ça a un prix. Nous voulons garder un outil de production agricole en France ne pas dépendre des importations étrangères qui n'ont pas les mêmes standards. C'est ce qu'on appelle aussi la souveraineté alimentaire française. Hé oui, cela a un prix c'est la même logique que celle de la réciprocité des normes que nous avons ancrée dans le débat européen depuis la présidence française. Le revenu agricole c'est aussi une retraite digne et des avancées ont été adoptées en la matière je salue notamment les lois Chassaigne hein et deux mais aussi la loi dit que le Sénat vient d'adopter, qui prévoit que le gouvernement. Devra travailler aux conditions d'une pension calculée sur les 25 meilleures années à partir de 2026 et avec la réforme des retraites dont vous vous saisissez on va permettre concrètement d'améliorer revalorisé de 350.000. Retraite avec 100 euros en plus en moyenne pour une carrière complète enfin monsieur le sénateur, l'avenir de l'agriculture, c'est assumer accélérer les transitions, vous l'avez dit, je partage, je n'insiste pas. Merci la parole est à d'autres collègues Jean Sol pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président Madame la Ministre, mes chers collègues. Avec le réchauffement climatique. La question de l'eau et de plus en plus préoccupante. L'été 2022, marquée par une sécheresse record et généralisée. L'eau est L'eau est indispensable à une multitude d'activités comme elle était indispensable aux grands équilibres les milieux naturels. Notre pays s'est dotée d'une législation qui vise un équilibre entre les différents usages de l'eau. Il s'agit de répondre à nos besoins, tout en préservant la ressource à travers toute une série d'outils. Un de ces outils et le débit réservé la loi interdit de prélever dans un cours d'eau si cela conduit à réduire son débit en dessous d'un certain seuil, et ce pour préserver la faune et la flore aquatique. Si le principe est vertueux j'attire votre attention sur ces difficultés d'application et les dérives auxquelles nous assistons saisi par des associations de protection de l'environnement. Le juge administratif est amené à fixer les débits réservés bien au-dessus de ceux décidés par les préfectures, dans les Pyrénées-Orientales, des prises d'eau sur le fleuve côtier la tête qui servent alimenter les canaux d'irrigation aux ancestraux faisant revivre une agriculture maraîchère familiale sont condamnés à être inopérante et donc fermée par décision du juge qui a estimé que les calculs des services de la préfecture pourtant très compétent est erronée. Se basant sur d'anciennes études de volume près le VAB le par ailleurs contesté le juge fait une application maximale des textes en s'écartant de l'objectif d'équilibre entre les différents usages de l'eau, au risque de condamner les activités maraîchère locale et de faire disparaître le système des cadeaux qui contribuent pourtant à la biodiversité locale ailleurs à Sallanches en Haute-Savoie cette même interprétation maximaliste du débit réservé pour conduire à la destruction d'centrales hydroélectriques. Madame la ministre ma question est simple, envisagez-vous de modifier les modalités d'appréciation du débit réservé pour éviter de décimer les agriculteurs en les empêchant d'accéder à l'eau. On vous répond de la parole est à la ministre déléguée en charge des collectivités territoriales et de la ruralité. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur. Je vous demande à nouveau d'excuser Christophe Béchu et nous partageons le diagnostic que vous posez. L'année 2022 a déjà été marquée par une sécheresse prolongée intenses et étendues, départements ont été contraints d'adopter des restrictions d'eau et 75 départements ont subi des situations de crise. Les perspectives pour 2023 sont donc suivis avec attention, d'ores et déjà cinq départements font l'objet de restrictions en raison de la sécheresse de l'année dernière et du déficit de précipitations que nous connaissons actuellement, nous avons au niveau de nappe globalement dégradée par rapport à l'année dernière avec 2 mois de retard sur le niveau de recharge le niveau de précipitations dans les mois qui viennent, sera crucial pour déterminer la situation dans laquelle nous serons l'été prochain. Notre rôle est bien sûr d'anticiper la situation est d'encourager encore et toujours. La sobriété des usages avec Christophe Béchu. Nous sommes pleinement mobilisés. Nous poursuivons le travail d'anticipation absolument nécessaire dès décembre. Je l'ai déjà dit à Madame, la sénatrice Carrère tout à l'heure, les préfets ont été chargés d'identifier les collectivités fragile en matière d'alimentation en eau potable pour les accompagner prioritairement les agences de l'eau pourront mobiliser. En 2023, 100 millions d'euros d'aides supplémentaires en faveur des projets de résilience très territoriaux les préfets coordonnateurs de bassin ont également été réuni le 27 février pour planifier des solutions liées aux problèmes de raréfaction de l'eau. La prochaine réunion aura lieu le 6 mars, un plan sur l'eau sera présenté dans les prochaines semaines, dans le cas de la planification écologique, portée par la Première ministre. Nous nous engageons à travailler sur les sujets que vous nous avez pas reporté dans votre question. Merci monsieur le sénateur Les acteurs de terrain de la politique de l'eau Madame la Ministre ne peuvent plus se contenter de réponses dilatoires. Il y a urgence à modifier les textes sur l'eau pour prendre en compte les besoins légitimes de nos territoires. Sinon les prochaines saisons s'annonce explosive. Je vous invite aussi à vous emparer des propositions du rapport récent de notre délégation à la prospective pour éviter une panne sèche généralisée. Je vous remercie. Merci la parole est à notre collègue Alain Dufour. Le groupe de l'Union centriste. Il y avait la parole. Monsieur le président, madame, la Première ministre Madame messieurs les ministres, mes chers collègues. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'. Bon, il n'est pas là mais je pense que Madame Dominique Faure va me répondre sur ce sujet, nous avons connu. En 2022, une sécheresse importante et au début de cette année 2023. La question a été posée à monsieur le président de la République dans le cadre du Salon de l'agriculture, il a répondu qu'il fallait. Prendre des arrêtés de restriction au niveau des préfets mais également. Dans le cadre d'infrastructures, le développement et la mise en place de retenues collinaires. C'est dans le sujet qui vous est proposé aujourd'hui. J'avais déposé une proposition de loi faisant état de la mise en place de retenue collinaires, de petite taille pour des superficies de moins de 150.000 m3.

les territoires être entendu. Le Salon de l'agriculture pour vous poser véritablement cette question qui me paraît tout à fait pertinente car effectivement leurs agriculteurs, les éleveurs, les vignerons de ce pays entame de de votre part une réponse particulièrement précise et efficace pour. Les rassurer définitivement merci. Madame Dominique Faure ministre délégué en charge des collectivités territoriales. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur du four. Je renouvelle toutes mes excuses. Pour l'absence de Christophe Béchu et je passe brièvement sur les réponses. Sur les réponses que j'ai déjà porté sur le diagnostic que vous posez. Sur ces sécheresses estivales et qui nécessite nécessite toute anticipation que je viens de citer et je viens. À la question des retenues collinaires. En fait, pour vous dire qu'il n'y a pas, monsieur le sénateur de dogmatisme. Il faut les apprécier au cas par cas, chaque projet qui respectera les critères exigeants que nous fixons pourra être validé le stockage hivernal lorsque les expertises techniques, le juge soutenables pour les milieux lorsqu'il s'inscrit dans un projet territorial largement concertée et lorsqu'ils participent d'un meilleur partage de la ressource peut être une solution. Les stockages hivernaux font partie du panel des solutions a mobilisé par contre ce n'est pas l'unique solution est sur beaucoup de territoires, cette solution ne sera pas techniquement techniquement possible. Soyez assuré que nous serons particulièrement vigilants sur les taux de remplissage de ses ouvrages dans le contexte actuel particulièrement tendu. Je vous remercie. Monsieur Dufour. Madame la Ministre, nous serons vigilants, les agriculteurs seront vigilants dans la mise en place de ce dispositif, car aujourd'hui il faut être dans l'action et non pas dans l'incantation. Les Français entame de d'une manière générale des résultats tangibles et vérifiés et vérifiables. Voilà la réalité. Merci. Merci. La parole est à notre collègue Catherine Bell Ricky pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président Madame la Ministre de la Transition énergétique chers collègues la crise actuelle a mis en évidence la dépendance énergétique de la France, tant financières que quantitative. indispensable de consolider à la fois nos filières de production énergétique et de développement durable sans y sacrifier notre indépendance aujourd'hui la Moselle nous en fournit les moyens et je vous ai écrit à ce sujet il y a déjà plusieurs mois. mois. 3 forages de recherche ont permis d'identifier un immense volume du gaz certifié de paix le gisement du gaz lorrain représente au total un volume de 190 milliards de mètres cubes de gaz, soit environ 5 années de consommation de gaz pour la France d'un point de vue technique, son exploitation présente l'Avantage décisif de ne pas recourir aux techniques de fracturation hydraulique ou d'autres procédés polluant. À la différence notable du gaz de schiste. De sorte que l'utilisation de ce gisement réduirait de 10 fois l'empreinte carbone de la fourniture de gaz. Aujourd'hui une entreprise française se tient prête à assurer l'exploitation de ce gaz à investir près de 20 millions d'euros et à créer de nouveaux emplois. Pour ce faire, il serait même possible après extraction du gaz de réaliser des enfouissements de CO2 dans le sous- sol ainsi libéré le temps de l'action est donc venu. Il est suspendu à l'accord du gouvernement concernant l'attribution d'une concession d'exploitation à l'entreprise qui se fait attendre depuis maintenant 3 ans. Cet accord renforcerait notre souveraineté énergétique au regard de nos relations extérieures avec d'autres pays et d'un contexte global imprévisible. Il contribuerait à stabiliser notre situation économique, marquée par une hausse du prix du gaz et du coup supporté par les entreprises et les ménages. Il sera durée enfin notre engagement sur le plan écologique et envoyé rendent mental si vous partagez ses objectifs Madame la Ministre l'exploitation du gaz lorrain peut-elle compter sur votre soutien. Pour vous répondre. La parole est au ministre de la transition énergétique. Madame Pannier-Runacher. Je mène au nom du gouvernement, une politique énergétique qui vise à sortir notre pays de sa dépendance aux énergies fossiles. Cette dépendance qui pèsent encore pour 2 tiers dans notre consommation énergétique finale d'autres stratégies, vous le savez, elle repose sur 3 piliers la sobriété, l'efficacité énergétique, puisqu'il faudra réduire notre consommation de de 40% d'ici 2050. Si nous voulons tenir notre objectif de neutralité carbone. C'est tout le sens du plan de sobriété que j'ai présenté avec la Première ministre en octobre dernier qui a permis de réduire notre consommation d'énergie de 10% cet hiver nous avons finalement fait en 3 mois ce que nous n'avions pas réussi à faire en 30 ans le 2ème pilier, c'est la production massive d'énergie renouvelable. C'est tout l'objet du projet de loi qui a été largement adopté sur ces bancs au mois de février, le 3ème pilier enfin c'est celui d'une relance historique de notre filière nucléaire là encore un projet de loi que vous avez adoptée et qui sera examiné ce soir. À l'Assemblée nationale dans cette stratégie, madame la sénatrice, nous devons mobiliser toutes les ressources de production disponible sur notre territoire en privilégiant les moins carbonée. C'est dans ce contexte que les services de l'État instruisent le projet d'exploitation de gaz dessous de couches en Lorraine, de la société française de l'énergie sur lequel vous m'interrogez ce projet, ce à extraire du méthane contenu dans les veines de charbon. Il a fait l'objet d'une enquête publique qui a mobilisé la population avec plus de 500 observation. En majorité défavorables au projet, les assurances, les associations environnementales locales se sont également exprimés contre ce projet, car vous le savez contrairement au gaz demi-de mines qui lui s'échappe de manière. Et qu'il est donc important de valoriser puisqu'il va directement dans l'atmosphère. Je porte la plus grande vigilance sur ses projets de gaz de couche qui consiste à investir dans une énergie fossile. L'instruction de ce projet est en cours de finalisation confirmant conformément au code minier et je serai amené à me prononcer dessus d'ici quelques semaines, je vous remercie. Madame belle Rithi. Alors l'étude qui avait été fait et les questions qui ont été posées ce ça s'est situé avant la crise que nous connaissons aujourd'hui et aujourd'hui je pense que les gens seraient favorables. À plutôt exploité un gaz mosellan plutôt que d'apporter un gaz de schiste des États-Unis. Merci madame. La parole est à notre collègue Annie. Le héros pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Monsieur le. Malgré les moyens du Ségur de la santé et ses promesses d'attractivité pour l'hôpital public. L'hôpital public continue de faire face à un absentéisme important et pallier au nombre postes Si l'intérim médical est nécessaire pour répondre aux difficultés temporaires de recrutement l'usage abusif qui en effet conduit je vous cite a un intérim cannibales qui rémunère injustement le nomadisme professionnel détruit la cohésion des ici des Certains professionnels sont devenus de véritables mercenaires de la santé font monter les enchères hebdomadaire du marché de l'intérim à 2003 1000 euros par jour, voire plus sur certaines périodes tendues en comparaison un jeune praticien à l'hôpital perçoit un salaire mensuel d'environ 4500 euros pour un engagement sans limite auprès de ses patients. Pour répondre à cette injustice. La loi de 2021, à encadrer les tarifs de l'intérim médical avec un plafond fixé par décret à 1170 euros brut pour une mission de 24h son application prévue en octobre 2021, a été décalé afin de prévenir les dysfonctionnements à un mois de la mise en oeuvre de la nouvelle échéance fixée au premier avril nous sommes alertés par les praticiens hospitaliers, notamment dans les services d'urgence qui peinent à boucler les plannings faute d'intérimaires acceptant les nouveaux tarifs. Avez-vous envisagé la réquisition de ceux qui profitent du système au mépris du serment d'Hippocrate pour éviter des fermetures de lits ou d'urgence, quelles mesures avez-vous prises pour éviter un nouveau recul dans le respect du temps de travail des praticiens hospitaliers titulaires et des patients qui ne doivent pas être les victimes collatérales de cette guerre de tranchées entre le ministère et ses mercenaires.

La régulation de l'intérêt médical est une constante et une préoccupation du législateur depuis au moins 2 mandatures et vous avez rappelé récemment une loi la loi Rist 2021 s'est aussi attaché à ce sujet. Je suis aussi. Très attentif au fait que votre assemblée, le Sénat surveille de près la mise en application des lois, c'est pour cela que je me suis engagé à mettre les décrets d'application de cet article sur l'intérim médical en action dès début avril. Bien entendu et vous l'avez dit, cela ne vise pas l'intérêt médical habituel, mais bien les dérives de l'intérim médical ces dérives qui fort heureusement ne sont que minorité dans l'ensemble de l'intérim médical. C'est d'abord une question d'éthique, mais même au-delà de cette question éthique. Il faut rappeler quelques chiffres, vous l'avez fait. 359 millions d'euros, c'est le coût pour les hôpitaux de l'intérim médical en 2021. Vous parliez de chiffre jusqu'à 3000 euros ça va même jusqu'à 5000 euros les 24h, là où le cadre et vous l'avez rappelé, 2170 euros. Au delà du côté financier, c'est aussi un véritable outil à détruire les équipes hospitalières et l'engagement des praticiens là où vous avez de médecins qui font le même travail et la payer 3 fois, 4 fois, 5 fois plus que l'autre pour la même période. Alors depuis plus d'un mois, j'ai demandé aux ARS d'animer des concertations locales, territoire par territoire, avec les préfets avec les élus pour affiner les diagnostics, établissement par établissement. je leur est également demandé de construire des solutions avec les professionnels de santé du territoire, mais également avec les CHU les établissements siège de j'ai acheté, dont c'est la responsabilité. J'en appelle également aux acteurs du privé des cliniques privées qui se sont engagés envers moi à suivre le même sens dans la rémunération. De ces périodes d'intérim médical. Je suis bien sûr avec une attention très particulière, l'ensemble des établissements et des établissements qui sont en fragilité et je peux vous assurer qu'aucun territoire ne restera sans solution. du plafonnement du prix de l'intérim qui démontrerait une fois de plus l'échec de votre politique de santé qui nécessite d'être revu de fond en comble avec la profession. Je crains que le respect du nouveau tarif ne soit un poisson d'avril au mépris de ceux qui s'engagent pour l'intérêt général auprès des patients et sans reconnaissance. La parole est à notre collègue Jean-Claude Amblard. Pour le groupe Les Républicains, vous avez la parole. Merci monsieur le président, ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Transition énergétique. Madame la ministre, alors que la France dispose du part hydroélectrique. Le plus important de l'Union européenne que ce par produit 12% de la production nationale d'électricité et qu'il est essentiel pour le mix énergétique, sa situation est aujourd'hui fragilisée par des années d'indécision. Les 340 ouvrages exploités sous le régime de la concession de services publics. Font face à l'absence de renouvellement des concessions échues dans de nombreux ouvrages dans la vallée de la trouille hier et du Lot, Aveyron. La situation du parc hydroélectrique nécessite une action urgente et déterminée en raison des conditions de renouvellement des concessions échues. Exploité un délai glissant et du contexte juridique modifiée par la règle. Européenne. Après la privatisation et le démantèlement d'EDF prévu dans le projet. Sur lequel je vous avez déjà interrogé ici-même, il y a 2 ans et qui aura provoqué de nombreuses oppositions contre lui. Le gouvernement est resté dans l'expectative en ce sens, la Cour des comptes a adressé une véritable mise en garde au gouvernement le 6 février dernier en soulignant la nécessité de sortir rapidement de cette situation, afin d'éviter que la situation ne se dégrade plus encore Oui, madame la ministre, il est urgent de vous intéresser à ce problème. Dernièrement l'hydroélectricité n'a pas été abordé dans le projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, ni dans celui visant à accélérer la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. Vous pouvez toujours vous abriter derrière l'annonce d'un prochain grand texte sur le sujet mais un. En attendant, les faits sont là. Alors Madame la Ministre pourrez vous pouvez-vous nous dire si vous partagez le constat sévère de la Cour des comptes sur l'inaction du gouvernement. Pouvez-vous nous dire si vous partagez la solution consistant à ce que les concessions soient fondés sur un ensemble de considérations économiques et juridiques. Madame la Ministre dites-nous vos difficultés sur le sujet et nous pourrons vous aider comme la Cour des comptes vient de le faire. Je vous remercie. Pour vous répondre. La parole est au ministre de la transition énergétique. Madame Pannier-Runacher. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur angles. Le gouvernement porte une grande attention à l'énergie hydroélectrique et à son développement, cette énergie renouvelable et pilotable est essentiel vous le savez à l'atteinte de nos objectifs climatiques, mais également à la sécurité d'approvisionnement des Français, ainsi qu'à la bonne gestion de la ressource en eau. Aujourd'hui la France compte plus de 2600 installations hydroélectriques qui ont représenté près de 11% de la production électrique française en 2022. Le secteur hydraulique. Vous l'avez rappelé contribue aussi à l'économie locale au travers des emplois créés dans les vallées. Vous avez cité, celle du Lot des de la crue hier mais également de la Dordogne ou des Pyrénées. La Commission européenne a engagé un précontentieux vis-à-vis de la France portant notamment sur l'absence de renouvellement par mise en concurrence des concessions hydrauliques échu comme vous l'avez évoqué, la Cour des comptes a présenté un rapport sur ce sujet le 6 février dernier en réponse à la Cour des comptes, le gouvernement a indiqué qu'il explorait plusieurs scénarios pour le renouvellement des concessions qui doivent satisfaire 5 objectifs clairs relancer rapidement des projets de développement, actuellement bloqué par le contentieux européens dont des projets de step garder la pleine maîtrise de notre parc hydraulique que pourrait fragiliser des remises en concurrence favoriser les synergies dans les usages de l'eau et faire en sorte que l'ensemble des bénéfices générés par l'exploitation des concessions bénéficient in fine et à la collectivité et. En fin de contrat souple avec des possibilités de modification assez vaste pour adapter ces dernières aux évolutions des besoins à court terme et peut-être cela vous a échappé. Le projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables. Adopté le 7 février dernier permet désormais de réaliser les investissements assurant la pérennité des ouvrages ouvrages hydroélectriques dont la concession est échu, quelle que soit la solution retenue, le gouvernement sera très attentif à la préservation du potentiel énergique techniques et humains des sociétés hydroélectriques hydroélectrique et à leur ancrage territorial. Merci la parole est à notre collègue Cyrille va pour le groupe Les Républicains. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre, mes chers collègues, ma question est le fruit d'une concertation transpartisane. Je la pose au nom des sénateurs membres du groupe développement économique de la montagne que j'ai l'honneur de présider. Nous sommes tous vivement inquiet par la situation économique des stations de ski et particulièrement les plus petites qui se trouve aujourd'hui dans une situation intenable d'asphyxie financière du fait de la hausse des coûts de l'énergie. L'ensemble des activités économiques et industriels sont bien évidemment touché mais certaines sont plus pénalisés que d'autres, ce qui nécessite un accompagnement complémentaire de la part de l'État. C'est le cas des domaines skiables qui subissent actuellement une double peine. Tout d'abord les domaines skiables subissent de la, de par leur activité une discrimination tarifaire au regard du mois d'attribution de la reine prévue par les textes, d'avril à octobre, alors que les plus gros pics de consommation des domaines skiables ont essentiellement lieu durant la période hivernale. De plus, malgré la mise en oeuvre d'aide appréciée et attendue des acteurs économiques de la montagne. Le dispositif d'écrêtement de la reine vient sensiblement réduire l'effet amortisseur de prix. Ce qui fragilise les structures et notamment les plus petites comme les régies de remontées mécaniques. Actuellement, plus de 40% des domaines ce qui a français ont récemment dû renégocier leur contrat d'électricité avec des prix vous ne pouvant être multiplié par 10 et des pénalités exorbitantes, en cas de rupture anticipée. De nombreux petits domaines se trouve donc aujourd'hui au bord de la faillite et pourrait déposer le bilan. Si le gouvernement n'agit pas. Pour les collectivités support de stations qui serait défaillante. La prochaine étape laisse peu de doute, la mise sous tutelle par la chambre régionale des comptes, ce qui serait dramatique pour tout l'écosystème montagnard, madame la Ministre j'avais alerté le ministre Bruno Lemaire au mois d'août du risque qui pesait sur les stations sur les stations il y a maintenant urgence. Comment peuvent-elles absorber une hausse des coûts de l'énergie qui passe de 3 à 20% d'un chiffre d'affaires. Ainsi, j'ai plusieurs questions. Comment comptez-vous adapter les dispositifs d'aide pour que les traitements ne viennent plus annuler le bénéfice des aides et ce, notamment pour les régies de remontées mécaniques. Comment comptez-vous prendre en compte les spécificités du domaine skiable pour la future réforme de la Qu'en est-il de la possibilité de renégocier les contrats. Maintenant que les prix se stabilisent des annonces ont été faites il y a quelques semaines. Qu'en est-il aujourd'hui. Merci. Merci monsieur le président, Monsieur le Sénateur. Votre question porte sur les effets de la hausse des prix de l'énergie sur les stations de ski. Vous le savez. Le gouvernement a mis en place plusieurs dispositifs d'aide et assez tôt d'ailleurs, les sénateurs, vous l'avez mentionné mais aussi les députés. Élus de la montagne ont échangé avec tout à la fois Bruno Lemaire et moi même et vous le savez très bien. Les régies. Par exemple sont. Absolument intégrer aux aides que nous avons déployé autant pour moi, je vous cherchais je vous remercie. Que nous avons déployés que nous continuons à déployer. Ça n'est pas une annonce anodine. Il est donc bien prévue. Ça va mieux en le répétant que les régies qui ont une taille équivalente à nos PME. Dans l'acception européenne jusqu'à 250 salariés soient couverts par l'amortisseur électricité soit parce qu'elles ont une personnalité morale soit parce qu'elles sont collectivité qu'elles ont rattaché une collectivité territoriale elles-mêmes bénéficiaires du dispositif. Il vous a pas échappé qu'ayant l'honneur d'être à la fois en charge des PME et du tourisme. Monsieur le sénateur, d'abord je suis proche des élus de la montagne aussi des acteurs économiques. J'étais encore au salon de la montagne il y a pas si longtemps, je veille avec beaucoup d'attention pour que l'ensemble des régies soient accompagnés et je vous le dis comme je l'ai dit à l'ensemble des élus de la montagne. Si vous avez des exemples spécifiques de régie qui ne rentreraient pas dans la grille que je viens de de vous dire, n'hésitez pas à me saisir au moment où on se parle je n'ai pas vu à date ça veut pas dire que demain il y en ait pas de remonter. Dramatique concernant des régies par ailleurs, je tiens quand même. Dans ce tableau un peu noir mais c'est le charme de l'échange que ce faudrait pas oublier non plus les fantastiques. Résultat, des acteurs de la montagne qui les chiffres sont sortis hier font des résultats remarquables. 42% de nos compatriotes ont l'intention d'aller au ski au cours de l'hiver 2023. En janvier 2023, on a un taux d'occupation qui est en hausse de 17% par rapport à janvier 2022 et pour février on enregistre une hausse de quasiment 12 points du taux de réservations par rapport à la même période il y a un an et perspectives sont belles, le gouvernement est là et pour ma part je reste à votre disposition si vous avez des sujets spécifiques, je vous remercie. Nous en avons terminé, merci madame, la Première ministre, mesdames et messieurs les Ministres. Avec les questions d'actualité au gouvernement. Les prochaines auront lieu le mercredi 8 mars à 15h. Je vais suspendre la séance elle sera reprise à 16h 30. Pour le débat d'actualité sur le thème des conséquences de l'inflation sur le pouvoir d'achat des Français. La séance est suspendue.

La séance est reprise. Madame la Ministre, mes chers collègues j'informe le Sénat que des candidatures pour siéger au sein de la CMP chargée d'élaborer un texte sur la proposition de loi visant à ouvrir le tiers-financement à l'état à ces établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique ont été publiés ces candidatures seront ratifiées si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure prévue par notre règlement. J'informe le Sénat qu'une candidature pour siéger au sein de la commission des Affaires européennes a été publiée, cette candidature sera ratifié si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure prévue par notre règlement. L'ordre du jour appelle la désignation des 19 membres de la commission d'enquête sur l'utilisation du réseau social TikTok son exploitation des données sa stratégie d'influence en application de l'article 8. Alinéa 5 de notre règlement. Les listes des candidats présentés par les groupes ont été publiés ces candidatures seront ratifiées si la présidence ne reçoit pas d'opposition dans le délai d'une heure prévue par notre règlement. L'ordre du jour appelle le débat d'actualité dont le thème sur la proposition du président du Sénat après concertation avec les groupes et le suivant les conséquences de l'inflation sur le pouvoir d'achat des Français. Dans ce débat. Le gouvernement aura la faculté s'il le juge nécessaire de prendre la parole immédiatement après chaque orateur pour une durée de deux minutes orateur disposera alors à son tour du droit d'répartis pour une minute. Le temps de réponse du gouvernement à l'issue du débat est limité à 5 minutes. Madame la Ministre vous pourrez donc si vous le souhaitez répondre après chaque orateur. Une fois que celui-ci ou à retrouver une place dans l'hémicycle. Dans le débat. La parole est à monsieur Stéphane Ravier pour les non inscrits pour 3 minutes.

Monsieur le Président Madame la Ministre, mes chers collègues. Depuis janvier 2021, les Français font face à une hausse de prix généralisée est inédite depuis 40 ans. Elle est principalement due aux restrictions d'activité de la période Covid combinée à de forte dépendance en matières premières et produits manufacturés en provenance de pays étrangers. En vérité, la guerre en Ukraine n'a fait que renforcer un phénomène d'inflation déjà bien installé. Les Français ont désormais une certitude, l'affaiblissement de l'État stratège et souverain voulue par votre gouvernement nous conduit à l'appauvrissement actuel. Selon l'Insee, l'inflation accélère à 6,2% en février sur les 12 derniers mois, avec plus 14,5% dans l'alimentation et plus 14% des prix de l'énergie de plus en plus de stations service affiche le prix des carburants, quel qu'il soit à plus de deux euros le litre, aujourd'hui un kilo de pommes de terre noisette surgelés coûte 2 euros 19 en février 2000, il coûtait 1 euros 0 5, soit une augmentation de 108% le prix de la crème fraîche fouettée a augmenté de 40% en rayon. 210 grammes des mental ramper coûter un euros 65 en février 2022, il coûte 2 euros 19 aujourd'hui, soit une hausse de 33%. Le chariot des courses et des classes populaires et de plus en plus réduit aux Restos du coeur a augmenté de 12% cette année, les banques alimentaires révèle et des 2.400.000 personnes, soit 3 fois plus qu'en 2011 dans la 6ème puissance économique du monde qu'est la France des millions de personnes ne mangent plus à leur faim ne se chauffe le plus ne se soigner plus. C'est le grand effondrement des classes populaires qu'une fiscalité toujours très importante accompagne dans l'affaissement de la classe moyenne française. La fiscalité est un vrai sujet pour le pouvoir d'achat des Français. Quand on sait que 60% du prix de l'essence ne sont que des taxes qui alimentent les caisses percée de l'état d'urgence et de remettre à produire en France pour permettre la création d'emplois et donc de salaire une fiscalité scène pour in fine et retrouver la croissance. Mais même, même après avoir éteint la lumière de leur domicile baisser voire couper le chauffage sacrifier le renouvellement de leur garde-robe et une partie du contenu de leur réfrigérateur. Les ménages, les retraités, les étudiants ne voit toujours pas le bout du tunnel inflationniste. Vos annonces et prévisions sont toutes se sont toutes révélées fausses. Le ministre de l'Économie avait promis l'effondrement à venir de l'économie russe suite aux sanctions au printemps 2022. Résultat, en 2023, le FMI révèle la très bonne santé économique de la Russie. Pendant que la nôtre, prend l'eau de toutes parts. Monsieur Véran véritable boussole qui indique le Sud avancée au mois d'août dernier que nous avions atteint le pic de l'inflation alors que les prix n'ont cessé d'augmenter depuis. Madame la Ministre, qu'entendez-vous donc pour sortir du marché européen de l'électricité et de la reine revenu Cléa risée relocaliser baisser la fiscalité, les cotisations patronales sur les salaires. Merci. Hein la ministre. Non. Non. La parole est maintenant au président Jean-Claude Requier pour le groupe RDSE pour cinq minutes. Monsieur Monsieur le président de la la ministre, mes chers collègues. À dans mes préoccupations de nos concitoyens dans les territoires ou celle des professionnels. Présents en ce moment au Salon de l'agriculture, ce débat sur les conséquences de l'inflation et peut être encore plus d'actualité, qui est celui des retraites. Le retour d'une forte hausse des prix à la consommation courante pour aller alimentaire pour dire entretien matériaux divers équipements de construction pour de l'énergie est un tournant majeur de l'après-Covid si le choc de la guerre en Ukraine et les sanctions contre la Russie. En yuans un effet indéniable sur les prix de l'énergie. La remontée des prix. Ah oui la réalité commencé dès 2021 au moment des premiers des confidences. Elle s'explique en particulier par l'augmentation du coût des matières premières et les transports notamment du fret maritime avec des marchandises en grande partie importés de l'étranger soit hors d'Europe. Nous commençons peut-être à payer le prix de la désindustrialisation et de la petite et la perte de souveraineté écolo.

Et l'inflation observé ou ressentie par les consommateurs qui n'est pas de son niveau de revenu de son lieu de résidence de ses préférences et de ses contraintes personnelles. Par ailleurs, l'indice des prix à la consommation ne donne pas une mesure complète. Du coup la du coût de la vie d'autres données lourde pèse lourdement sur le budget des ménages comme le prix. Je vois que les statisticiens intérieure de l'indice pondéré des loyers de façon générale les les prix des actifs mobiliers ou immobiliers ont beaucoup augmenté ces dernières années, qui ont massives de liquidités par les banques centrales. A entraîné une forte inflation des valeurs mobilières sur une longue période, mais qui n'avait pas eu d'impact sur les prix alors consommation. Le taux d'inflation courant était lui aussi resté faible voire nulle. Pendant des décennies à peine atteignait à peine atteignait il l'objectif de 2% fixé par la Banque centrale européenne, l'inflation est longtemps resté un souvenir remontant aux années son Soit le fait des pays en développement comme la Turquie l'Iran le Venezuela ou l'Argentine. Aujourd'hui elle touche à nouveau l'ensemble des pays développés peut-être à calculé sur à quelques exceptions près comme le Japon. Les conséquences de cette inflation sont à la fois massive et inégal. Une baisse du pouvoir d'achat des ménages, une érosion de l'épargne. Mais qui dépendent beaucoup de la part de chaque poste de dépense dans le budget individuel déménage.

Face à la complicité de calculer l'inflation et du pouvoir d'achat des indices Lyon alternative plus ont été élaborées. D'abord l'indice Big Mac aux États-Unis suite à l'indice jambon-beurre plus français. l'économie seulement un quatre de lui élaboré la mise inflation perçue qui intègre des paramètres plus individuels et subjectifs dernièrement. L'agence Bloomberg a créé un indice Coco un Qui intègre le prix des ingrédients nécessaires à la préparation de ce plat traditionnel sur Alain il y aura augmenté non pas de 6% comme l'indice synthétique et les prix mais de près de 15%. Si les prix de l'ensemble des produits de consommation semble maintenant se stabiliser ceux des produits alimentaires, hors eux fortement augmenté depuis l'été 2022. C'est dans ce contexte tendu que devrait aboutir au plus tard aujourd'hui, les négociations commerciales entre fournisseurs et distributeurs de produits de grande consommation à propos desquels le Sénat a adopté une importance une importante, proposition de loi, il y a 2 semaines. Des questions, voilà le ministre en conclusion de mon propos. Face à ce défi de l'inflation, le gouvernement prévoit-t-il des mesures supplémentaires. En faveur du pouvoir d'achat en plus des nombreuses initiatives qu'il a déjà prise depuis un an et demi et qui connaissent des fortunes diverses. Même si elles contribuent plus qu'ailleurs à atténuer les DVD inflation sur les ménages et Anzin dans son panier devient anti-inflation. Le gouvernement envisage-t-il aussi de mettre à contribution les entreprises, en particulier celles qui ont largement bénéficié d'aides publiques ces dernières années. Merci monsieur le président, madame la ministre. Merci. Bien sûr, monsieur le sénateur. Merci monsieur le. Président, Monsieur le Sénateur. Je m'attelle arrête. Répondre à vos questions, parce que j'ai pas grand chose à remettre en question dans vos propos ni d'ailleurs sur l'indice un peu. Maquereau. Qui est porté par l'Insee ni sur ce que vous avez dit sur la l'inflation ressentie. Qui me semble être la boussole, la plus importante à suivre. Vous dire quand même que la progression en matière d'inflation. Elle est réelle et je ne la renie en rien le gouvernement non plus. On est à 6,2% sur un an. Et on est très clairement avec une accélération de la poussée inflationniste en matière alimentaire, vous l'avez vu hier, les chiffres sont sortis plus 14 5 % d'inflation en février, après plus 13% en janvier. Pour autant, si cette inflation et demeure soutenu l'Insee constate aussi que la croissance a été positive au 4ème trimestre et que malgré tout, fruits aussi des mesures prises par le gouvernement, le pouvoir d'achat au 4ème trimestre. Pouvoir d'achat de nos concitoyens n'a pas chuté, n'a pas été morcelé, n'a pas sombré pourquoi parce que les prélèvements obligatoires et notamment fiscaux, continuer à diminuer. C'est l'effet aussi de la suppression de la redevance télé. C'est l'effet de la 3ème tranche de la suppression de taxe d'habitation mais aussi grâce à une politique très volontaire en matière d'emploi, vous le savez et au versement particulièrement élevé, dixit les l'Insee. De la prime. Partage de la valeur. C'est plus d'un milliard d'euros pour aller vite, qui ont été distribué à un million de salariés en moyenne 1000 euros par salarié. Donc le pouvoir d'achat se maintient malgré cette inflation soutenue. Vous m'avez posé une question très très clair, j'y réponds aussi clairement, le gouvernement a beaucoup fait. Le gouvernement continue à faire en sorte que nous partagions les efforts. L'État a fait beaucoup les Français font beaucoup. Nous demandons le président de la République en chef. La Première ministre et Bruno Lemaire aussi et votre modeste serviteur à ce qu'aujourd'hui les distributeurs notamment essaye de contribuer à l'effort en essayant de faire des opérations qui puisse permettre en prenant sur leur marge et non pas sur celles de nos producteurs. Qui puisse permettre de limiter l'inflation alimentaire le plus possible aux caisses, nous sommes donc toujours en poursuite de négociations sur ce sujet par mer. Si Madame la Ministre, Monsieur le Président. OK pas de réponse. La parole est maintenant au président Serge Babary pour 7 minutes pour le groupe Les Républicains.

Monsieur le Président Madame la Ministre, mes chers collègues. La guerre en Ukraine depuis le 24 février 2022. Ses conséquences sur les prix des matières premières a servi de catalyseur à de profonds bouleversements économiques. Le 1er d'entre eux et le retour de l'inflation qui avait pratiquement disparu depuis plus de 20 ans. La crise de la Covid depuis l'apparition de nombreux goulot d'étranglement au niveau des chaînes de production. Avait déjà entamé les vertus d'un commerce mondial libéral fonctionnant en grande partie sur la base d'une énergie à bas coût. Même si certains économistes envisager en 2022 une reprise modérée de l'inflation. Le retour de cette dernière, à des niveaux jamais vus depuis 50 ans a surpris tous les spécialistes en effet. L'affaiblissement croissant de la conjoncture mondiale une mondialisation permettant de baisser les coûts de production, notamment en Asie et l'abondance des matières premières énergétiques bon marché ont fixé durablement l'inflation sous la barre des 2%. La sortie de la crise sanitaire de 2020 a généré une demande soutenue de la part des ménages désireux de pouvoir enfin consommer après des semaines de confinement. Les prix de nombreux produits ont ainsi augmenté face à une production insuffisante désorganisé. Il y a des difficultés de transport mais c'est surtout la guerre en Europe de l'Est qui a perturbé l'acheminement de matières premières énergétiques industrielle et alimentaire. En réponse aux sanctions occidentales. Les Russes ont sensiblement réduit leur exportations de gaz en direction des Européens jusqu'à les arrêter, ils sont un suivi une forte hausse des cours du pétrole et surtout du gaz européen qui a généré une flambée de l'inflation. Cette dernière a ainsi atteint plus de 10% en zone euro, mettant sous pression le pouvoir d'achat des ménages entraînant logiquement une baisse de la consommation. La guerre en Ukraine n'a pas provoqué l'inflation elle renforcer et accélérer. Paradoxalement, l'inflation à doper la croissance du chiffre d'affaires des principaux groupes français du CAC 40 qui affiche plus de 140 milliards d'euros de résultats nets cumulés. Ces résultats s'expliquent par des montées en gamme des plans d'économies mais aussi et surtout par le fait que la très grande majorité a pu répercuter dans ses prix. La flambée des coûts. Tels n'a en revanche pas été le cas de très nombreuses ETI et PME. Consommatrice d'énergie dans le domaine industriel agricole et artisanale. Le cas bien concret des nombreuses fermetures de boulangerie. On est le meilleur exemple. Madame la Ministre pourquoi ne pas avoir supprimé le critère lié à la puissance installée. Permettant de bénéficier des tarifs réglementés de vente d'électricité des fameux 36 qui En début de semaine, les ministres européens de l'énergie se sont retrouvés à Stockholm. Madame la Ministre où en est la réforme du marché européen de l'énergie qui avait été annoncé pour la fin de l'année 2022. A-t-on enfin obtenu le découplage du prix de l'électricité et du gaz. Combiné à l'augmentation du prix de l'énergie, l'inflation des prix des produits de grande consommation en Puccini. Significativement, le pouvoir d'achat des Français. De 5% l'été dernier, l'inflation des prix à la consommation sur un an s'établit aujourd'hui à 6,2%. À cette crise du pouvoir d'achat s'ajoute une crise sociale voire sociétal. Selon une étude publiée ce lundi de 4 millions de personnes bénéficier de l'aide alimentaire. Fin 2022, soit 3 fois plus qu'il y a 10 ans. En ce début d'année plus d'un tiers des personnes accueillies sont des nouveaux bénéficiaires. Dès juillet 2022, notre collègue, présidente de la commission des affaires économiques. Sophie Primas. Vous enjoignait de cesser cette politique de chèques dispendieuse. Éphémère. Et d'engager une politique ferme de revalorisation du travail et notamment de la défiscalisation et désocialisation des heures supplémentaires. L'exercice était certes difficile mais faute d'anticipation et d'évaluation suffisante la loi pouvoir d'achat n'a eu qu'un effet pansement moyennant un coût non négligeable pour nos finances publiques. Les prix des produits alimentaires ont bondi de 14. 5 % sur un an. La confiance des ménages est dégradée. Mais le taux d'épargne qui s'établit à 16,6% du revenu brut. Selon France Stratégie. Les conséquences de la crise varie selon le profil des ménages. Les personnes âgées éloignées des centre-ville étant particulièrement exposés. Alors que les négociations commerciales entre eux industrielle et les enseignes de la grande distribution s'achève aujourd'hui. On nous annonce un mars rouge. Hier devant nos collègues députés. Bruno Lemaire a écarté cette idée et affirmé que des solutions applicables aux produits alimentaires étaient à l'étude plus encore. Des mesures efficaces et crédibles devrait nous être présenté dans quelques jours. Pourtant, la Fédération du commerce et de la distribution évoque une augmentation à venir de l'ordre de 10%. Et ce matin même en plein Salon de l'agriculture, la présidente de la FNSEA accuse une partie des distributeurs de refuser de payer l'intégralité de la part des agriculteurs. Les causes de la crise inflationniste. On l'a vu sont multiples. Cette crise appelle une stratégie claire des mesures ciblées et des investissements long. Madame la Ministre quel sera le plan du gouvernement pour aider les Français à traverser cette nouvelle crise. Je vous remercie. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre je vous en prie. Merci monsieur le président. Monsieur le Président Babary je ne reviens en rien sur les causes et merci d'avoir appelé aussi la le retour de la demande post-Covid qui a contribué a boosté l'inflation avant même la guerre en Ukraine. D'abord j'ai à coeur de vous répondre sur le bout. Qui est. Tarifaire et la question précise sur les 36. Kilovoltampères. Vous parlez dans votre conclusion de la nécessité de cibler les aides et je connais la sensibilité de la chambre haute et la vôtre et la mienne à la dépense publique. Nous avions face à ce choix de problématique, nous aurions été amenés à accompagner des entreprises qui n'aurait pas eu besoin d'être sous un bouclier. Et donc prise en charge et ça aurait entraîné des dépenses publiques massives. Ça se compte ici en milliards. Et et ça n'aurait pas été idoine on aurait accompagné des entreprises, en un mot qui n'en aurait pas forcément eu besoin par ailleurs je voudrais pas qu'on oublie. Si ça, si c'était si simple ça aurait peut-être été fait mais que pour installer des compteurs, ça ne se fait pas du jour au lendemain et que ça aurait été de l'. Par des énergéticiens. mais c'est important et je connais votre sérieux donc en termes de logistique n'était pas si facile que ça et ça n'aurait pas été fait, du jour au lendemain, donc nous avons choisi de cibler un amortisseur plus un guichet qui est assez facile impôts Point gouv Point FR tout est disponible et pour les TPE un tarif à 280 euros le mégawattheure lissé sur l'année 2023. Vous. Parlez de pansement, en matière de soutien au pouvoir d'achat. Je voudrais quand même rappeler l'ampleur du pansement. Le bouclier tarifaire qui protège nos concitoyens de la hausse des prix de l'énergie, c'est 110 milliards d'euros. de présence de l'État entre octobre 21 et décembre 2023, 110 milliards d'euros. C'est un plan de relance de la consommation à lui tout seul, je voudrais pas qu'on oublie non plus le paquet pouvoir d'achat. Avec la revalorisation des APL des minima sociaux. La prime de rentrée exceptionnelle. L'adoption du chèque énergie exceptionnel. Mais aussi, et je le disais, la prime partage de la valeur. Je connais votre sensibilité aux entreprises 300.000 entrepreneurs de nos TPE ont versé plus d'un milliard d'euros à un million de salariés pour justement accompagner les salariés dans cette poussée inflationniste. J'ai pas assez de temps pour les autres questions, j'y répondrai par écrit je vous remercie. Merci, madame la Ministre, la parole est maintenant Madame Vanina Paoli-Gagin pour le groupe les indépendants pour cinq minutes. Monsieur le Président Madame la Ministre, mes chers collègues. Avec les conséquences économiques de la pandémie, les sécheresses. Le dérèglement climatique 2021 réunissait bon nombre de conditions propices et une inflation record. L'invasion de l'Ukraine par Poutine encore aggravé cette situation, les prix de l'énergie ont bondi la crise alimentaire est devenue plus menaçante. Lorsque les Russes ont délibérément choisi de bloquer les exportations ukrainiennes blé. Nous craignons que la fin du quoi qu'il en coûte apporte son lot de faillite et le retour de la guerre en Europe dans des économies déjà très éprouvée par les confinements. De présager rien de bon. Au cours de la difficile année 2022, les prix ont augmenté en France de 6,2%. J'espère ne choquer personne en disant que ce n'est pas si mal. Sur la même année. À titre de comparaison, l'Argentine a battu son propre record avec 95% d'inflation et plus proche de nous, le Royaume-Uni Global Britain ont enregistré une inflation de 11%, devant les États-Unis avec quant à eux 7 pour au sein de l'Union, l'inflation moyenne constatée sur 2022 a été de 10 pour %. Avec une guerre à nos portes avec la raréfaction notre approvisionnement en gaz l'envolée du prix des hydrocarbures avec nombre de nos centrales à l'arrêt. Je crois pouvoir dire que nous en sommes plutôt plutôt pas trop mal tiré. Bien que quand on se compare on se console. Quand on se regarde, on se désole quand même. L'inflation frappe plus fortement les plus des nos concitoyens, ceux dont le pouvoir d'achat est fortement contraint par les dépenses obligatoires les dépenses courantes, ceux-là sont en grande difficulté. Les prix alimentaires ont bondi de 14,5%. Cela pèse très lourd dans le budget des ménages français. C'est aussi le cas, tout le monde le sait, des prix de l'électricité avec un mégawattheure qui est passé de 220 euros en décembre 2021 à 700 euros au cours de l'année 2022 il est heureusement redescendu depuis mais malgré le bouclier énergétique, la facture de nos concitoyens a néanmoins augmenté de près de 15%. Les prix des carburants ont également atteint des sommets grevant l'activité de tous ceux qui travaillent, les artisans, les chauffeurs, les livreurs et plus généralement de tous les Français, particulièrement ceux qui vivent en milieu rural. Face à ces augmentations frappant plus violemment les plus vulnérables d'entre nous. La tentation est grande de recourir à l'argent public. Entre la crise de la Covid et les difficultés économiques que nous rencontrons actuellement notre dette publique elle aussi cette envolée. De 1300 milliards en 2019. Elle avoisine aujourd'hui 3000 milliards avec la remontée des taux d'intérêt cet état de fait est alarmant. Il est urgent de renverser la vapeur et de commencer à réduire notre dette publique. Mais alors, quelles solutions pour améliorer le pouvoir d'achat de nos concitoyens. J'envoie de principalement tout d'abord et au risque de choquer. La sobriété. En 2022 années de grande tension énergétique, la consommation électrique de notre pays a nettement baissé par rapport à 2021 grâce notamment aux efforts consentis par nos entreprises et par nos concitoyens à travers nos écogestes. Nous avons même réussi à diminuer notre consommation par rapport à l'année 2020 qui était quand même marqué par les confinements et où les gens sont beaucoup rester chez eux. Les prix délirants, de l'énergie rendre ainsi bien plus rentable. Les travaux d'isolation et les énergies renouvelables. La sobriété présente en outre l'Avantage de ne pas participer à la spirale inflationniste. La 2ème solution pour le pouvoir d'achat. Ben c'est le travail. Les aides gouvernementales sont toujours prélevées sur nos concitoyens, que ce soit par l'impôt ou par la dette. Nous ne devons jamais l'oublier. Nous saluons donc l'effort du gouvernement, madame la ministre, depuis 2017 pour s'efforcer de réduire le des contributions sont nos entreprises, nos concitoyens, nous souhaitons que cet effort soit poursuivi notamment sur les impôts de production. Il nous faut favoriser les investissements dans nos territoires pendant les infrastructures que dans l'appareil productif. Le dérèglement climatique, nous exhortait depuis bien longtemps à changer nos modes de production. La crise que nous traversons peut être l'accélérateur de ce changement. Les Chinois désigne par un même mot crise et opportunités. Il y a longtemps que les Français le savent. À défaut d'avoir du pétrole. Nous nous devons d'avoir encore des idées et cette fois-ci des bonnes je vous remercie. La parole est donc maintenant Monsieur Paul Toussaint Parigi pour le groupe écologiste pour cinq minutes. Monsieur Monsieur le Président Madame la Ministre, mes chers collègues. Les chiffres sont historiques. 6,2% d'augmentation des prix à la consommation sur un an. Sur les six derniers mois, les structures alimentaires partenaires du réseau des banques. Alimentaires ont recueilli un tiers de personnes en plus. La hausse des prix creuse dramatiquement l'écart entre les Français qui, vous le savez, selon leurs revenus, mais aussi leur lieu de et conditions de vie subissent plus ou moins fortement les conséquences de la crise qui marginalise et précarise à vitesse accrue. Une grande partie de nos concitoyens. À titre d'exemple. Et selon les récente étude de l'OFCE et de France Stratégie le choc varie fortement en fonction du profil des ménages. Les personnes âgées pauvre éloignées des centre-ville étant plus impactées. Si l'inflation moyenne. Sur l'année 2022 se situait à 5,2%. Elle était de 8,5% pour les ménages étaient plus exposées, et de 3 4 % pour les moins touchées, soit un écart de 5 points en défaveur des plus précaires. Cela je le constate. De chaque jour en Corse sur mon territoire majoritairement rural dont 18% de la population vit sous le seul de pauvreté. Contre 15% sur le plan national. Chaque jour, je constate aussi les ravages de la crise qui accentue la précarité et creuse les inégalités car aux conséquences de la crise, s'ajoute pour notre territoire, le surcoût induit par l'importation de nouveaux produits et matières premières. Face à ce constat, force est de constater que des mesures apportées par le gouvernement sont à ce stade insuffisante et trop ponctuelles face à une crise qui sa racine. Face à une précarisation structurelle qui a hélas contribuer à aggraver en actant de nombreuses régressions sociales. Réforme de l'assurance chômage, baisse des APL. Quant aux mesures temporaires comme la revalorisation anticipée des minima sociaux en deçà de l'inflation n'apporte aucune solution durable. Pire. Le gouvernement agite et se vante de mesurettes à effet d'un moulinet par temps de canicule. La création d'un panier anti-inflation sur une cinquantaine de produits basés sur le volontariat. Nous pouvons que remercier d'action ambitieuse de ce gouvernement, à la, à la hauteur de ces enjeux En 2021, une étude de l'Insee ce aide alimenter a montré que 64% des personnes interrogées expriment de la honte à se rendre à l'aide alimentaire. La création d'une prime d'alimentation aurait limiter tout effet de stigmatisation et laisserait les personnes actrice de leur alimentation. Au cours des derniers mois notre groupe. Avait porté plusieurs propositions afin d'aider les Français face à l'envolée des prix. Nous avions proposé dès juillet dernier, de protéger les plus précaires en établissant des mesures visant à limiter un pour de la hausse des prix des loyers. Pour les locataires. L'Espagne, elle a suivi cette voie en limitant la hausse à 2%. Nous avons défendu l'augmentation des salaires, notamment du salaire minimum porté à 1500 euros Net. Aujourd'hui nous défendons une augmentation substantielle des minima sociaux. Au-delà du seuil de pauvreté comme l'instauration d'un revenu minimum garanti. Aucune de ces propositions pourtant efficaces immédiatement et sur le long terme n'ont trouvé écho du côté du gouvernement, nous ne pouvons que le regretter. Enfin, j'ajouterais que si l'inflation actuelle a des origines conjoncturelles, notamment du fait de la guerre en Ukraine et ses conséquences. Quant à l'acheminement des produits agricoles énergétiques. Nous serions tous coupables. Si nous en mettons un facteur structurel, celui de la réaffectation des ressources. En effet, nombreuses sont les études scientifiques qui ont directement liées. La baisse des rendements agricoles ou encore de la production industrielle avec la hausse des températures. Le réchauffement climatique impacte donc de manière durable le coût et les volumes de production, entraînant une hausse inexorable des prix. La Banque centrale européenne a déjà averti à plusieurs reprises sur le sujet. La dégradation de l'environnement, associé à l'arrêt, vérification des ressources nous expose donc à une inflation de fond qui touchera plus durement les Français les plus modestes. C'est pourquoi nous ne cesserons de le rappeler, il est aujourd'hui urgent de donner des moyens à la France de réussir sa transition écologique et de mettre en place une économie au service de la construction de la sobriété. Aujourd'hui nous sommes au regret Madame la Ministre de constater que le gouvernement n'apporte aucune solution durable à cette crise sans précédent qui. Merci,

Merci monsieur le président, Monsieur le Sénateur par Heidi. Chacun qualifie comme il le veut. Les mesures mises en place par le gouvernement mais je ne peux pas. Ne pas réagir à l'esprit de à l'entendent surtout de mesurettes, comme vous l'avez mentionné. Quand on parle de ce que nous faisons maintenant depuis 2 ans et demi. D'abord, vous aurez remarqué que je ne me suis pas. J'ai pas commencé par rappeler. Les chiffres de l'inflation et surtout le fait que, effectivement, par rapport à nombre de nos voisins européens, on peut peindre le tableau comme on veut. Mais la France s'en sort quand même. Mieux que l'ensemble de ses voisins européens et ça n'est pas le fruit du hasard auquel je ne crois pas. C'est le fruit aussi d'une politique économique, c'est le fruit d'un combat pour l'emploi, c'est le fruit d'un travail de fond pour faire baisser les prélèvements obligatoires et les impôts que payent nos Français et augmenter leur pouvoir d'achat. Vous dites mesurettes je le redirai autant de fois qu'il faudra le dire 110 milliards d'euros de soutien à la demande par le truchement du bouclier tarifaire pour nos compatriotes. Si ça c'est une mesurette. Alors il faut m'expliquer comment on forme un budget pour ce qui est juste de vous fixer une comparaison l'ensemble des Français payent en matière d'impôt sur le revenu, 86 milliards d'euros. Nous avons mis plus pour accompagner les Français durant cette période que ce que nous récoltons en matière d'impôt sur le revenu. Nous avons. Augmenté les minima sociaux vous considérez Monsieur pas Reljic c'est assez. Nul ce que nous avons fait en un mot, chacun pense ce qu'il veut. J'ai quand même à coeur de partager ce que ça donne, ça donne pour un certain nombre de nos compatriotes. Des aides allant de 202 377 à 416 euros selon les âges et les enfants par famille pour l'allocation de rentrée scolaire, ça donne aussi un accompagnement de 687 euros nets annuels pour une secrétaire de mairie avec 15 ans d'ancienneté. Grâce à l'augmentation du point d'indice, mais aussi un gain de 543 euros nets annuels pour un agent d'accueil en début de carrière par exemple. Dire que ce sont des mesurettes je ne disant je suis pas d'accord, dire que vous auriez fait autrement. C'est le charme de nos échanges dans la chambre haute. Je vous remercie. Si Monsieur Paris dit. Non. La parole est maintenant madame Nadège avait pour le groupe RDPI pour six minutes. Monsieur le Président Madame la Ministre, mes chers collègues. Pendant plus de 30 ans, la hausse durable des prix leur hausse généralisée à la fois sur les biens et les services a été contenue en France la rupture intervenue à l'été 2021 fûts soudaine, avec des conséquences négatives sur le pouvoir d'achat des Françaises et des Français sur le fonctionnement de nos services publics de nos entreprises et de nos collectivités. Cette rupture fut violente et en particulier pour les plus modestes car le renchérissement du coût de la vie touche avant tout les produits alimentaires et l'énergie. Ils touchent aux fondamentaux de notre vie quotidienne et c'est par conséquent pour les responsables publics. Public pardon que nous sommes une préoccupation majeure. D'où la tenue de débats réguliers et d'où notre débat de cet après-midi. Les causes sont multiples et de nature différente. Certains, certaines d'ordre conjoncturel, d'autres plus structurelle. Un effet cocktail en somme. Cette inflation est la conséquence de la sortie de crise pandémique, avec une demande qui a pu nettement augmenté plus fortement que l'offre restait fragile sur certains produits. Elle est la résultante de l'agression militaire russe en Ukraine qui a occasionné une baisse des exportations et une montée des prix des matières premières. Elle est aussi alimentée par la baisse de l'euro qui a renchéri les prix des importations. Les prix de l'énergie ont aussi été mis sous pression. l'explication ne réside pas que dans le contexte international, elle réside aussi dans un fait durable l'épuisement des sources d'énergie fossiles couples couplé avec l'impérative transition écologique qu'il nous faut nécessairement mener de front. Cette rupture fut et de mort demeure pendant ce cependant moins appuyé en France qu'ailleurs. Avec un taux à 6,2% sur un an selon la dernière note de l'Insee publiée hier, la France reste en dessous de la moyenne de la zone euro et le pic. Inflationniste. Cela a été dit, devrait être atteint cette année. Les explications sont à trouver dans les politiques mises en oeuvre depuis maintenant plus d'un an fièvre l'inflation. L'État a agi il agit et agira encore nous soutenons toutes vos actions en effet afin de soutenir le pouvoir d'achat, de nombreuses mesures ont été adoptées. Avec la revalorisation des minima sociaux des prestations sociales et familiales, de même que des pensions de retraite de base. Globalement, les dispositifs de soutien ont porté sur l'encadrement des prix de l'énergie, 12 millions de ménages les plus modestes ont été destinataire d'un chèque de 100 ou 200 euros en décembre dernier, un chèque exceptionnel a été attribué à se se chauffant au fioul ou principalement au bois. Une action résolue sur le travail aussi, revalorisation du point d'indice des agents publics, la prime Macron devenue prime pour le partage de la valeur. Un dispositif pérenne que les entreprises peuvent mettre en place chaque année. Il a bénéficié à 5,5 millions de salariés en 2022, une augmentation de 50% par rapport à 2021 et avant tout au sein des petites entreprises. Une prime moyenne de 739 euros pour un total de 4 4 milliards d'euros. Elle a contribué à préserver le pouvoir d'achat des ménages en 2022 en dépit de la hausse des prix l'Insee le rappelle également par ailleurs j'en profite pour saluer l'accord intersyndical validé par la CFE-CGC, la CFDT, FO et la CFTC. Son objectif généralisée largement des dispositifs tels que l'intéressement, la participation et la prime de partage de la valeur à toutes les entreprises de plus de 11 employés, on avance sur ce point essentiel. Je forme le voeu que nous continuer à que nous continuions pardon a avancé lors de l'examen du texte plein emploi je pense enfin au projet de loi énergie adoptées ou en cours de discussion au Je citais les derniers chiffres de l'Insee. Quel est le constat dans le détail une baisse sur les coûts de l'énergie 14% sur un an, contre 16 3 en janvier. Mais une persistance d'une hausse sur les prix de l'alimentation et des services, alors que les négociations annuelles entre distributeurs et industries agroalimentaires s'achève, les prix dans les rayons des supermarchés pourrait encore grimper. Il est par conséquent nécessaire Madame la Ministre qu'une vigilance particulière soit portée en ce domaine afin de maîtriser ce que j'appellerais la fellation de l'assiette en visite au Salon de l'agriculture samedi le président de la République s'est exprimé à destination des pêcheurs en donnant de la visibilité sur les aides mais aussi sur la hausse des prix dans les supermarchés en appelant les distributeurs à faire un effort sur leurs marges. Il y a la détermination des nouvelles mesures adaptées ciblée et puis il y a je dirais l'optimisation du recours au dispositif existant, un exemple pour aider les Français modestes à faire face à la flambée des prix du carburant, le gouvernement a mis en place une indemnité de 100 euros parce que plusieurs millions de conducteurs. Ne s'était pas encore manifestée, vous avez on a annoncé la prolongation du délai de demandes jusqu'à la fin du mois de mars sur les aides, nous devons le faire savoir dans nos territoires respectifs. Je voudrais conclure en soulignant la situation en Outre-mer le ministre Jean-François Carenco, a présenté en décembre un plan pour préserver le pouvoir d'achat des ultramarins fruit d'intenses négociations ce plan traite essentiellement de l'élargissement des bouclier qualité/prix adaptées à chaque territoire, où en est-on de 7 ou 10 non du pouvoir d'achat à la carte alors qu'au-delà de cette période inflationniste. La vie chère est un problème structurel en outre-mer je vous remercie. Merci monsieur le président, madame la sénatrice. a déjà vu, je suggère. Si vous l'autorisez parce que le sujet est trop important pour que je l'ai lu de répondre sur la question Oudinot. Outre-mer. Par écrit, après la séance dans cet hémicycle pour que je sois parfaitement complètes vous m'avez aussi et en même temps. Interrogé sur la prise de parole du président de la République au Salon international de l'agriculture samedi matin et. Les actions qui vont arriver et que nous appelons de nos voeux. Pour continuer à juguler ensemble la poussée inflationniste qui même si elle est moins forte en France qu'ailleurs reste assez soutenue en matière alimentaire. Et comme l'on dit. Nombre d'entre vous frappe en réalité très diversement nos concitoyens à commencer par les plus fragiles C'est donc un, un sujet sur lequel nous continuons à travailler. L'idée est assez simple, au même titre que je l'ai dit. D'abord les Français nos compatriotes contribue. Et pour certains voient la hausse des prix et la paye. L'État a pris sa part. Je ne vais pas refaire. Le point sur le bouclier tarifaire et l'ensemble des aides, je l'ai fait juste avant mais juge sur 2023. Ces 46 milliards d'euros. Pour vous donner une idée, c'est plus que le budget du ministère de la Défense. Hé oui effectivement au même titre que les énergéticiens ont fait un effort, si nous arrivons à un prix à 280 euros le mégawattheure sur les TPE et à réussir à faire avancer le sujet avec les PME, c'est parce qu'ils ont contribué total aussi. Le président de la République a effectivement avec Bruno Lemaire demander aux distributeurs de faire un effort et d'y contribuer en prenant sur leur marge nous attend donc nous attendons donc des propositions dans les prochains jours, un objectif, une solution collective tous ensemble juste ou les distributeurs prendraient sur leurs marges et non pas sur la marge de notre producteur ou de l'amont de la chaîne et surtout une solution rapide qui soit efficiente et surtout opérationnel pour les Français dans les supermarchés. Dès l'arrivée du printemps qui vous le savez arrive à la fin mars. Nous sommes en train d'échanger et nous continuerons à le faire dans les prochains jours pour trouver une solution qui accompagne nos compatriotes durant les prochains mois. Merci. La parole est maintenant Madame Viviane Artigalas pour le groupe socialiste pour 4 minutes.

Merci monsieur le président, mes chers collègues. Madame la Ministre Bruno Lemaire, a dit la semaine dernière qu'il ne croyait pas aux prévisions des économistes, qui estiment qu'il faut s'attendre à un mois de mars rouge et à une inflation qui dépasserait les 10% sur les produits alimentaires. Il a dit je le cite, ce n'est pas la réalité. Alors j'aimerais vous rappeler ce qu'est la réalité quotidienne de plus en plus de nos concitoyens depuis près d'un an, les prix à la consommation ont augmenté de 6% à cause de l'inflation, le nombre de bénéficiaires de l'aide alimentaire a augmenté de 10% en 2022, les retraités et les étudiants sont touchés mais aussi les personnes qui ont un emploi. Les prix de l'énergie ont augmenté de 16%, malgré le bouclier écrit faire et la remise à la pompe. Dans les outre-mer l'inflation et la forte dépendance de ces territoires aux importations via l'aviation est le fruit maritime se répercute particulièrement sur le prix des produits alimentaires dans ces territoires également les mêmes mécanismes entraîne les mêmes conséquences sur les populations les plus précaires. Il renforce le sentiment prégnant d'une vie encore plus cher à raison d'un coût de la vie déjà supérieur à celui de la métropole et ça aussi c'est la réalité, cette hausse globale les des dépenses contraintes à un aime pas directe sur la capacité des plus modestes à se loger. Le nombre de ménages en retard de paiement de loyer de plus de 3 mois a augmenté de plus de 10% en 2 ans et la précarité dans le logement, c'est aussi la précarité énergétique. 5,6 millions de Français sont dans cette situation et le chiffre ne baisse pas avec la loi climat et résilience, le gouvernement s'est fixé un objet pour objectif d'éradiquer les logements énergivores d'ici 2028. Or, avec 37% de passoires technique thermique occupés par des ménages vivant en dessous du seuil de preuves pauvreté. Avec un reste à charge extrêmement important pour les familles modestes avec une réelle de difficultés d'accès aux droits et aux aides auxquelles elles ont droit, faute d'un accompagnement adéquat. Comment réussir à atteindre une telle objectif nous formulons elle fasse elle inlassablement des propositions Madame la Ministre dans le cas de de loi de finances successifs, par le biais de propositions de loi dernièrement avec mon collègue Rémi Cardon. Nous avons déposé une PPL qui propose de recentrer l'effort budgétaire du pays sur l'éradication des passoires thermiques thermiques de mettre en place un reste à charge zéro pour les personnes les plus précaires et d'assurer un égal accès aux dispositifs d'accompagnement sur tous les territoires, y compris dans les zones peu denses. Vos mesures, vous les avez cités, elles contiennent certes l'inflation et limite des hausses des prix de l'énergie mais elles ne sont ni pérennes ni structurel et ne cible pas les classes moyennes et populaires, les plus en difficulté. Elles sont donc incapables de répondre à nos enjeux sur le long terme. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y aura pas de mars rouge. Les Français sont déjà dans le rouge. Or, pour lutter contre les conséquences de l'inflation. Il faut de la cohérence et une véritable justice sociale, le forfait charge des aides au logement doit être réévaluée. Le chèque énergie doit attendre atteindre sa cible les personnes chauffées en collectif comme les locataires du parc social et les copropriétaires ne peuvent y recourir pour payer leurs factures. Même constat pour les personnes hébergées en foyer ou en résidence sociale. Toutes ces personnes sont éligibles mais ne peuvent pas utiliser le chèque énergie, comment expliquez-vous cette inégalité quand on demande aux 5,6 millions de ménages en situation de précarité énergétique dans les plus exposés aux aléas climatiques et à le hausse des prix de l'énergie d'agir pour la sobriété énergétique dans un but de transition écologique. On ne peut pas leur reprocher d'éprouver un fort sentiment d'injustice car ce sont eux les moins favorisés qui sont les premiers à payer la facture et il en faut peu madame la Ministre, pour que ce sentiment ne se transforme en colère. Merci cher collègue. Madame la Ministre non. La parole est maintenant monsieur Éric Bocquet pour le groupe CRCE pour cinq minutes. C'est le président Madame la Ministre, mes chers collègues. Dès le mois de décembre 2020, les prix de l'énergie ont massivement augmenté, plus 41% pour le gaz entre décembre 2020 et 2 octobre 2021, plus 21% pour le carburant. Plus 4% pour l'électricité et la tendance, c'est bien sûr confirmé en 2022, l'envolée des prix de l'énergie, nous y entraîner dans une spirale inflationniste, atteignant des niveaux record que nous n'avions pas connue depuis les années 80. En janvier 2023, les prix de l'énergie ont ainsi crû de 16,3% en glissement annuel, tandis que ceux de l'alimentation. Eux ont connu une hausse de 13,3%. Concrètement pour les ménages, c'est plus 20% pour les pâtes. Plus 29% pour le steak haché, plus 34% pour les légumes frais et jusqu'à 120% pour l'huile de tournesol, chacun s'en souvient, le passage en caisse devient une épreuve. Pour beaucoup, il faut choisir, manger, se chauffer ou se déplacer plus de 10 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, dont un enfant sur 5, 7 millions de personnes vivent dans une situation de précarité alimentaire et doivent, cela a été rappelé par beaucoup de nos collègues recourir à l'aide alimentaire La fréquentation des Restos du Coeur a augmenté de 12% en 6 mois. Situation inédite. Six mois avant le Russie le conflit russo-ukrainien le 6 octobre 2021. Le journal Les Échos s'inquiéter et titré sur ses je cite trader pris dans la folie spéculative du prix du gaz. Et pour cause, sur un mois, l'activité sur les options, c'est-à-dire les produits dérivés spéculatifs sur la matière première avait bondi de 158% dans la même veine, si l'invasion de l'Ukraine par la Russie a bouleversé les chaînes de distribution. Certains, dans certaines entreprises profitant de leur position dominante sur les marchés ont spéculé sur les prix des denrées alimentaires ou augmenter leur marges dans certains cas, mais tout cela n'est pas vraiment nouveau. Cela fait près de 3 ans que nous vous alertons que les associations vous alerte sur la paupérisation croissante d'une partie toujours plus importante de la population. Du côté des PME, même son de cloche pour les entreprises du secteur agroalimentaire, c'est plus 29% pour le coût des matières premières agricoles par rapport à 2021, plus 26% pour le coup des emballages cartons et plastiques, plus 57 pour les coûts de l'énergie. Et ce n'est pas fini. La facture d'électricité et de gaz va être multiplié par 3. Dès 2023, par rapport à 2022 et par 5 par rapport à 2021, voire davantage en ce sens ce débat d'actualité n'en est pas vraiment hein c'est un, d'un bilan des mesures prises par le gouvernement pour tenter d'enrayer l'inflation, la spéculation et la perte de pouvoir d'achat qui s'ensuit dont nous avons besoin ou est le chèque alimentaire promis dès 2020 par le président de la République. Comment expliquer que 50% des personnes ayant droit à l'indemnité carburant d'un montant de 100 euros ne la demande pas. Idem pour le chèque énergie côté aide aux entreprises. Le bouclier tarifaire exclu de nombreuses entreprises qui en raison des équipements nécessaires à leur activité possède un compteur électrique dont la puissance est supérieure à 36. L'amortisseur. Se révèle également insuffisant au regard de l'explosion cumulée des prix des matières premières et des produits énergétiques de plus la complexité des différents dispositifs ne permet pas aux bénéficiaires de s'en saisir massivement. Alors oui, comme le soulignent de nombreux consommateurs, le prix des biens de première nécessité a moins augmenté que dans d'autres pays en France mais il a tout de même augmenté dans des proportions sensible alors que de nombreux États ont mis en place des mesures de revalorisation des salaires. Vous avez préféré des mesures ponctuelles sans portée générale, vous continuez de ménager le capital au détriment du travail et pourtant la relégation de la question des salaires en marge du débat politique explique pour l'essentiel la baisse de la qualité de vie de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Ainsi, selon l'OCDE, la France est le pays qui a subi la plus forte baisse des revenus réels au 2ème trimestre 2022 là où la majorité des autres pays ont progressé et paradoxalement, alors que les dividendes battent des records, tous les jours. Notre pays connaît une hausse de la pauvreté inédite depuis de très nombreuses années, selon les mots d'Olivier De Schutter, rapporteur spécial de l'ONU. Manger à sa faim se chauffer, se soigner, devrait être un droit fondamental et une pris une priorité politique c'est la pauvreté qu'il vous faudrait combattre cela vient un véritable blocage des prix alimentaires via une augmentation des salaires et des minima sociaux via un tarif réglementé du gaz et de l'électricité pour tous et la sortie du marché européen de l'énergie. Autant de mesures que nous portons dans cet hémicycle de manière constante, merci. Merci cher collègue. Madame la Ministre je vous en prie. 2 3 choses déjà, effectivement, on ne sera pas d'accord sur une chose. Quand on est à 7,2% de taux de chômage après 6 ans d'action résolue. Quand on a un taux de chômage de nos jeunes qui est. Le plus bas ou parmi les plus bas en réalité le plus bas depuis qu'on le mesure. Quand on a. Une réindustrialisation de la France qui est en cours. Ça prend du temps parce qu'on part de loin, oui. Quand on a 1725 décisions d'investissements étrangers sur la seule année 2022, permettant de créer ou de maintenir plus de 58.000 emplois industriels sur notre pays alors même que ses employes depuis 15 ans, 20 ans, quitter le pays. Oui, je vous répondrais d'abord et avant tout mais j'ai à coeur de parler des associations aussi que la meilleure façon de faire en sorte qu'on ait du pouvoir d'achat et qu'on puisse en sortir d'ailleurs pas que pour des raisons pécuniaires mais aussi pour des raisons d'épanouissement personnel et je sais que nous ne serons sûrement pas d'accord. C'est le travail. Le travail c'est vers ça que qu'on jouait verges toute notre politique et notamment notre politique fiscale l'allégement des prélèvements sociaux. Nous n'avons pas oublié, j'imagine que vous non plus. La baisse des cotisations sur les fiches de paye qui à augmenter les salaires nets en 2018 et ça aussi ça fait 6 ans qu'on se bat pour que le travail paye mieux. Est-ce à dire que nous ne faisons rien et j'ai été en charge de l'économie sociale et solidaire et j'ai trop de respect pour les acteurs associatifs pour laisser dire que nous ne faisons rien. Dans le PLFR 2022 qui a été votée, c'est quasiment 60 millions d'euros pour les associations. Hier encore, le ministre-Combe, annonce 60 millions pour 2023 pour l'aide alimentaire de qualité. Je passe les 27 appel à projets du plan de relance dont j'ai eu l'honneur de parler aux banques alimentaires pour que l'État tout au long de l'année 2020 et 2021, continuer à les soutenir financièrement. Oui, on se bat pour que les gens travaillent et que le travail paye mieux. Hé oui on a trompé en même temps celles ou ceux qui n'ayant pas de travail, ont besoin de la solidarité nationale. J'avais à coeur de le rappeler, je vous remercie. Merci. Monsieur Bocquet. La parole est maintenant monsieur le questeur Vincent Capo Canellas. Pour le groupe Union centriste pour huit minutes. Monsieur le président, madame la mes chers collègues. Rarement un débat sera autant tomber à point. Si nous devions nous interroger sur l'intérêt des débats d'actualité. Nous aurions sans doute la réponse aujourd'hui. À quelques heures de la fin des négociations commerciales. La grande distribution les agriculteurs. Les industriels. Le gouvernement se renvoient la balle sur une hausse à venir de 10% des prix alimentaires. Des chiffres filtre 25% d'augmentation éventuelle pour les boîtes de Nesquik 10% aurait dit Coca-Cola 17% pardon. Si l'inflation ralentit et si nous avons jusque-là évité c'est fort bien la boucle prix-salaires la hausse des prix alimentaires et elle plus alarmante. Et même si nous essayons de faire la part des choses, on ne peut qu'être inquiet bien sûr 6,2% d'inflation en France, c'est mieux que huit et demi dans l'ensemble de l'Union européenne. Bien sûr, le gouvernement a su mettre en place un certain nombre de mesures. Ça a été rappelé pour soutenir le pouvoir d'achat telles que la remise carburant l'indemnité inflation le chèque énergie, le bouclier tarifaire sur le gaz, l'électricité ou encore des aides ciblées pour les ménages et bien sûr les entreprises. Mais hier, mardi, nous avons connu l'inflation alimentaire de février sur un an. À savoir 14 et demi pour 100. Et le constat est simple, les prix des denrées alimentaires évoluent de manière beaucoup plus forte que l'inflation. Et ce qui filtre des discussions en cours laissent entrevoir des hausses élevé sans doute de même niveau. Le président de Système U à parler 10 pour %. Le président de Carrefour a été plus alarmant encore. L'addition des 14,4% déjà constaté avec la hausse attendue disons de leur de 10% si elle devait se confirmer. Fait froid dans le dos. Il y a bien sûr une part le bras de fer dans ce face-à-face annuel. Entre. Chacun des acteurs de la distribution. quand même pose question. Les distributeurs accueilli des transformateurs qui désigne du doigt les hausses des prix des matières premières. Voir les agriculteurs. Le gouvernement demande de grandes surfaces de réduire leurs marges. Il évoque un panier un chariot de prix alimentaires. Qui devrait être maintenus sous contrôle et vous nous direz peut-être mal analyse tout à l'heure où vous en êtes de ces discussions avec quel dispositif vous pensez pouvoir mettre en oeuvre. On peine à expliquer totalement ces augmentations. L'année dernière. La guerre en Ukraine, les prix de l'énergie et des matières premières, ceux des transports ceux des produits. Facturé pouvait expliquer l'inflation alimentaire mais en 2023, ces chiffres sont bien moindres. Bien sûr, le niveau des prix de production. Relais peu à peu l'inflation déjà constaté et se diffuse. L'inflation des prix de production serait 17 pour ce chiffre au demeurant élevé est inférieur à celui qui existe dans le reste de l'Union européenne. Faut-il y voir. L'une des causes et augmentation attendue quoi qu'il en soit. Si le pouvoir d'achat a pu être préservée en 2020 et 21. Il a baissé. De 0 2 % en 2022 et nous risquons de perdre cet acquis en 2023. Il est vrai qu'en 2022, les salaires ont augmenté de 4,2% en moyenne et l'inflation de 6, le niveau des prix va être dans son évolution au niveau des salaires. Les aides de l'État et les primes ne pouvant rester élevé. Le moral des ménages est à un niveau qui devient plus faible. Le sujet et que les salaires augmentent moins vite que l'inflation et que la consommation s'en trouver affectée. Alors que c'était jusque-là un des moteurs de notre économie. Sur ce point, il nous faut peut être voir comment l'avenir peut être construit. La soutenabilité notre budget nous appelle bien sûr à la plus grande vigilance et c'est toute la quadrature du cercle. Elle suppose cette soutenabilité un effort collectif reposant sur la maîtrise de la dépense, qui doit être couplée à la recherche d'une plus grande efficacité de celle-ci. Il y a bien sûr une consacra. Une contradiction dans dont il ne faut essayer de sortir la croissance, la maîtrise de l'inflation sont de ce point de vue là des nécessités. Peut être. Vous nous direz-vous comment vous voyez les choses sur ce plan là. D'ici là, il faut sans doute répondre de manière. Segmenté à un certain nombre d'urgence. L'Observatoire français des conjonctures économiques. Il a publié une étude, certains l'ont rappelé sur les mesures budgétaires importantes qui ont été mises en place et sur leur effet sur le pouvoir d'achat, les Français en 2022 et 2023. Il estime qu'en 2023 le pouvoir d'achat pourrait revenir à son niveau d'avant la crise sanitaire fin 2019 et se réduire de 1,2% à 2%. Entre la fin 2021 et la fin 2023. Bien sûr, sans les mesures prises l'Observatoire estime que la baisse du pouvoir d'achat entre fin 2021 et fin 2023 toujours aurait pu atteindre 5% tout l'efficacité des mesures qui ont été mises en oeuvre. il est vrai que le bouclier tarifaire, la remise carburants ont semble-t-il permis de soutenir le pouvoir d'achat en moyenne à hauteur de 790 euros en 2022. Et. Aussi de soutenir le niveau de vie des ménages les plus modestes de 5,1%. Et j'ai noté que pour les ménages les plus aisés. C'était de 2,2%. C'est l'impact de l'inflation sur les ménages touchent les Français. Il le fait de façon inégale en fonction de leurs revenus de leur situation personnelle et de leur lieu de vie. Selon les travaux de l'OSCE encore les ménages ruraux se éloignées des centres urbains et les plus modestes seraient les plus touchés par ce phénomène inflationniste. Ah la la ministre ça ne nous invite peut être à réfléchir à des mesures différenciées qui pourrait voir le jour afin de prendre en compte l'impact disparates de l'inflation. Alors évidemment c'est très difficile d'avoir des mesures très catégoriels. Mais tout de même, on voit bien qu'elles touchent de manière différenciée selon les situations. Selon. Les âges même et selon les territoires concernés. Selon une étude des banques. Le nombre de personnes bénéficiant de l'aide alimentaire a triplé en 10 ans, avec une hausse de 10% en 2022. 2,4% millions de nos compatriotes ont été accueillis par ces structures pour bénéficier d'une nourriture gratuite ou très peu cher. Disons cela je n'oublie pas et vous l'avez rappelé vous-même Madame la Ministre. L'effort qui a été fait sur l'emploi mais sur un certain nombre de mesures de soutien mais je ne veux pas non plus nier les difficultés. Avant de conclure, je voudrais rajouter un élément. L'envolée des taux d'intérêt affectent la capacité des ménages, notamment les primo-accédants à devenir propriétaires. C'est je crois une grande difficulté. Beaucoup de. Primo-accédants potentiels sortent du marché. Et on a là un point d'alarme. Tant pour. Le secteur immobilier et la construction que bien sûr et avant tout pour ceux qui veulent accéder à la propriété. Pour les accidents, je crois que protéger. Proroger le PTZ, dispositif coeur du soutien à la propriété. Serait particulièrement utile dans un contexte de hausse des taux. Et. Peut-être faut-il réfléchir aussi à développer massivement le bail réel solidaire, notamment pour les jeunes ménages ça serait me semble-t-il des mesures utiles et en tout cas il y a un sujet sur la cherté. Du logement et la difficulté d'accession. Comme le logement pèse dans le budget des ménages pour une part importante aussi pour les locataires ou futurs locataires du parc social. Il y a sans doute aussi une réflexion à conduire pour pas mettre parfois des loyers plus adapté. Nous mesurons Madame la Ministre l'ampleur des difficultés l'effort qui a déjà été réalisé. Nous avons ici une pleine conscience des contraintes budgétaires. Mais les mesures que le gouvernement doit semble-t-il annoncé sont pour beaucoup une question de vie quotidienne et même d'urgence. Je vous remercie. Merci monsieur le questeur Madame la Ministre. Merci monsieur le président. Monsieur le questeur. D'abord merci de la précision étayé de vos chiffres et de vos sources. C'est vrai que dans ces débats et vous avez été nombreux à le dire d'ailleurs, peu importe les, les bancs. Le débat mais je ne suis pas étonné tomba à point nommé. Il vous a pas échappé mais comme vous l'avez mentionné, je vais le préciser que je ne me suis pas. Caché derrière des chiffres. Macro et que je reconnais. La réalité de l'inflation et de l'inflation alimentaire ressenti par nos compatriotes et ayant en charge les PME mais aussi la consommation. C'est à l'aune de cette inflation ressentie que je raisonne, je voulais juste pour corroborer vos propos. Rappeler que l'Insee. Pas plus tard qu'hier, a rappelé qu'au total sur l'année 2022 le pouvoir d'achat et globalement préservés. Il ne faudrait pas oublier de prendre en compte ce que vous avez fait l'ensemble des mesures et notamment les chèques. Énergie ainsi le pouvoir d'achat dit ajusté progresse même de 1,2% en 2022. J'en profite aussi pour répondre indirectement aux sénateurs Babary les bonnes nouvelles sont rares. Le taux de marge de nos entreprises progresse aussi sur le 4ème trimestre et s'établit en moyenne à 32% en 2022. Il baisse un peu par rapport à 2021 qui était une année particulière mais il est quand même au-dessus de son niveau de 2018, 2 0,5 point, c'est-à-dire qu'on sort après la crise sanitaire. On est aujourd'hui dans une crise inflationniste et nous avons des entreprises dont. Le taux de marge quoi qu'il advienne, est en augmentation. Vous m'avez demandé. En un mot aussi où nous en étions côté grande distribution et à la suite des travaux que nous menons, je le redis le suite à l'annonce à la demande du président de la République nous travaillons. D'arrache-pied avec Bruno Lemaire pour en marquer les distributeurs à nos côtés, mettre en place une solution collective rapide juste j'ai proposé une idée, c'est une sorte de mise de jeu, je n'ai jamais dit que c'était la seule solution et j'ai encore moins dit qu'elle était parfaite. Elle a le mérite d'exister, de pouvoir être critiqué de pouvoir être soutenu j'attends et Bruno Le Maire de contrecoup propositions dans les jours qui viennent. Hé bien, j'exagère qu'on paye moins cher à la caisse, vous. Merci monsieur le président. Pas de réponse. Dernier orateur inscrit, Monsieur le Président, Patrick Kanner pour le groupe socialiste pour cinq minutes. Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues. Ce matin, je, j'écoutais une chaîne de télévision continue et qui est titré. Inflation mars le mois de tous les dangers. Je vous ai aussi écouter madame sur une une grande chaîne publique. Ce matin, vous voyez. C'est important, c'est le ça se met de bonne humeur. En novembre. Dernier. Lors d'une audition par la commission des affaires économiques. Monsieur le Ministre de l'Économie avait confirmé ses déclarations précédentes et a indiqué que l'inflation que nous subissions n'était que transitoire avec une baisse des prix interviendrait à partir de fin 2022. Nous sommes dans le 1er trimestres 2023 et cette baisse des prix n'est pas intervenue. Alors oui, pour certains ce trois mois. C'est peu de chose. Mais pour ceux qui éprouvent des difficultés financières, c'est une éternité, on le sait aujourd'hui, cette inflation sera pérenne. Les estimations portent plutôt sur une stabilisation d'ici 2025. Mais de quoi parlons-nous. Finalement en 2025. Inflation nulle. Inflation de 3%. Comment vont évoluer les taux d'intérêt. Quelle politique sera menée par la BCE. Personne ne peut le dire, au vu de la vitesse à laquelle évolue l'économie mondiale et je crois qu'on a intérêt à se méfier des estimations de et la sagesse qui commanderait à relativiser toutes les prévisions que nous pourrions faire. Il faut donc avoir en tête que malheureusement les épisodes de choc économique que nous avons connu, notamment avec la Covid seront amenés à se répéter à devenir de plus en plus fréquent. Les prévisions donc peuvent être faussées. Mes chers collègues. L'objet du débat d'aujourd'hui porte sur les conséquences de cette inflation sur le pouvoir d'achat des Français et en particulier des plus modestes de nos concitoyens. Or malgré le courrier que madame, la Première ministre a pu m'envoyer. Il y a quelques semaines. Je reste persuadé que les difficultés éprouvées par les foyers français sont prégnantes. je reste mobilisée pour lutter contre la précarisation avec mes collègues du groupe socialiste, écologiste et républicain contre la fin. Des mois difficiles contre toutes ces trappes à pauvreté que ce gouvernement Madame la Ministre continue de ne pas voir, c'est d'ailleurs pour cela que notre groupe a proposé la tenue de ce débat. me je suis heureux de voir que Monsieur Larchet et pu le retenir dans ce. Voilà. Dans ce contexte qu'on appelle maintenant les débats d'actualité du 1er mercredi de chaque mois. Il est important de continuer à porter ces sujets au sein du débat national. Il est important de continuer à être les porte-voix des concitoyens les plus modestes. Madame la Ministre aucune prime. Aucun chèque. Ne remplacera une hausse juste et durable des revenus pour maintenir et seulement maintenir le pouvoir d'achat. Car non Madame la Ministre l'augmentation du SMIC de 8% et les aides ponctuelles mises en place par votre gouvernement ne suffisent pas à compenser la véritable déflagration économique que certains foyers ont pu subir et continuent à subir. Par ailleurs, l'obsession du dogmatisme. Moins d'impôts que vous vous vous évertué à ériger comme solution à tous les problèmes ne semble pas approprié à ce contexte. En fait en termes de ruissellement, c'est celui de la précarité que nous connaissons de plus en plus Madame la Ministre. Les mesures que vous avez pu prendre en faveur du pouvoir d'achat existe nous le reconnaissons. Pour autant, les coupes budgétaires que vous avez pu opérer pèse également sur le budget des Français les plus modestes. Je pense bien sûr symboliquement à cette baisse de 5 euros décidée au début du quinquennat précédent sur les aides au logement. Ce qu'il faut aux Français, ce ne sont pas des chèques énergie des chèque carburant ou d'chèques de rentrer. Ce qu'il leur faut c'est une revalorisation des salaires. Le groupe socialiste, écologiste républicain d'ailleurs rédigé une proposition de résolution demandant que soit tenu un Grenelle des salaires en France à l'initiative de notre collègue Thierry Cozic ce qu'il leur faut, c'est mettre fin au désarmement fiscal Pour rappel la politique mise en oeuvre par votre gouvernement entraînera une perte de 500 milliards d'euros de recettes fiscales entre 2017 et 2027. Ce qu'il leur faut français c'est une répartition des richesses dans les entreprises prospères qui soit juste. Nous vous avons proposé de taxer les superprofits. Nous avons été soutenus par des millions de Français. y compris même par des collègues parlementaires issus du centre. Vous ne nous avez pas là non plus entendu il y a quelques jours était confirmé des dividendes qui atteignent des records, 140 milliards. Cette situation n'est pas juste et devient insupportable. Il est demandé à tous les Français de fournir un effort et on va y venir dans quelques heures sur le débat concernant les retraites, la décence serait de demander le même effort à tous nos à tous nos concitoyens y compris ceux qui ont le plus bénéficié de l'hyper bouclier fiscal depuis maintenant bientôt 6 ans, nos concitoyens que nous voulons aider Madame la Ministre, ce ne sont pas. Les plus riches, vous l'avez compris mais ceux qui aujourd'hui font exploser les chiffres des restaurants du corps du coeur de notre pays. Madame la Ministre, ce qu'il faut aux Français je termine là-dessus. Monsieur le président je ne sont pas des mesures ponctuelles, ce qu'il leur faut c'est une réelle redistribution sinon, attention danger le désespoir est source de toutes les colères, je vous remercie. Merci monsieur le président. Monsieur le Président. Kanner. Décembre noir. Juillet vers Mars rouge. Dieu sait si j'aime la peinture. Mais je ne crois pas qu'il relève d'un membre d'une équipe du gouvernement. De choisir le Pantone. Des difficultés qui sont devant nous et on ça je comprends tout à fait la position que je partage si tenté vous en doutiez de mon ministre de tutelle Bruno Lemaire. Sur le fait que l'inflation va demeurer soutenue est soutenu et va demeurer soutenue sur le fait et nous serons d'accord là-dessus. Monsieur le Président, canard, vous avez parlé de choc. Qu'effectivement nous sommes face à un choc inflationniste et sur le fait qu'il était indispensable qu'en plus, que de ce que nous faisons depuis maintenant 6 ans. Nous continuons à essayer de faire plus. C'est bien pour ça que nous demandons en responsabilité aux acteurs économiques aujourd'hui de faire un effort sur le choc inflationniste, d'ailleurs là aussi. Je serais plutôt d'accord avec vous, je ne suis pas devant, je ne saurais. Mentionné d'ailleurs ni précisément son début et encore moins ça enfin ce que je sais mentionné, c'est ce que j'essaye modestement de faire au nom du gouvernement pour accompagner les Français, vous dites-nous je dire on nous sommes les les porte-voix des plus modestes. Je ne vais pas revenir. J'ai peu de temps mais, à défaut de de je sais pas si c'est des porte-parole ou des porte-voix en tout cas c'est des portes actions que vous avez au sein du gouvernement. Nous n'avons pas tremblé quand il a fallu augmenter les minima sociaux, nous n'avons pas trompé je l'ai dit tout à l'heure pour les 5,7 millions de fonctionnaires dont le point d'indice a été revalorisé dès juillet avec la plus forte hausse depuis 37 ans, j'ai donné un exemple mais je voudrais en donner un autre c'est pour l'illustrer un gain de plus de 1093 euros nets annuels pour un infirmier anesthésiste avec 8 ans d'ancienneté. Nous avons effectivement revaloriser aussi la prime d'activité à plus de 4%. Vous appelez de vos voeux. Une conférence sur les salaires. Je l'entends bien, je rappellerai mais je sais que vous le savez puisque je vous respecte. Monsieur le Président canard que jusqu'à preuve du contraire, l'État ne fixe pas les salaires et c'est très bien comme ça. Je vous remercie. Merci madame la ministre. Monsieur le Président Kader non. Madame la Ministre. Il vous revient de conclure si vous le souhaitez pour cinq minutes. Merci

Messieurs les sénateurs. D'abord, merci pour ce débat, cet échange qui, malgré nos divergences pointe je pense le sujet de préoccupation de nos compatriotes et en ça, un débat qui me semble. Absolument indispensable à avoir ensemble. De mon côté, j'ai essayé de vous faire part du fait qu'indépendamment du choc inflationniste, nous menons depuis maintenant 6 ans une action résolue pour accompagner le pouvoir d'achat des Français pour revaloriser le travail. J'entends aussi avec beaucoup d'humilité que toutes ces solutions, en tout cas pour certains vous paraissent largement insuffisante. On se les dit mais je pense important de le rappeler même si c'est compliqué et que le ressenti. Est majeur, il faudrait quand même pas oublier. Que nous demeurons très en deçà de l'inflation que subissent nos voisins européens et que là encore. Le hasard est un. Concept mais c'est aussi possiblement le fruit de politiques économiques résolus depuis 6 ans après, j'ai envie d'être assez clair et dans le cadre du respect que je porte à la chambre haute évidemment. Est-ce à dire que nous en faisons assez. Non parce qu'en réalité on n'en fera jamais assez pour revaloriser le pouvoir d'achat de nos concitoyens. On n'en fera jamais assez contre l'inflation et notamment l'inflation alimentaire pour les plus fragiles et donc. On doit on humilité continuer à proposer des solutions. On doit aussi faire attention j'ai bien entendu notamment du président Kader dont je connais l'expérience les propositions en matière de salaire. Attention à l'alimentation de la spirale inflationniste à laquelle certains pays européens ont cédé qui conduirait. Par exemple, possiblement comme l'ont fait les belges. à une indexation de tous les salaires sur l'inflation. Je n'oublie pas que les belges ont une indexation des salaires sur l'inflation mais n'ont pas de bouclier tarifaire. Et je sais que vous êtes nombreux à raisonner dans le contexte contraint que connaissent nos finances publiques, avec des taux d'intérêt qui désormais dépasse les 3 14 %, puisque l'inflation a aussi la Bourse de Paris hier l'a démontré des conséquences directes sur la crédibilité financière de la signature française. À côté des mesures financières que nous avons prises. Je veux aussi vous dire que nous prenons des mesures qui peuvent paraître pas ici mais parfois dans les débats secondaires pour certains mais qui ne le sont pas. Je veux aussi vous rappeler avec la loi pouvoir d'achat et notamment les abords des sénateurs que nous avons aussi améliorer le pouvoir du choix de nos compatriotes quand ils veulent se dégager d'un abonnement quand ils veulent arrêter de payer des abonnements et qui souhaitait résilier facilement. C'est le cas aussi au-delà du gaz, de l'électricité des magazines et d'Internet pour les assurances et les mutuelles et d'ici 3 mois au plus tard au 1er juin 2023. L'ensemble des vendeurs et assureurs devront prévoir un bouton résiliation en ligne facile d'accès, la résiliation des abonnements la facilitation et le dégagement par les consommateurs de ces engagements peut aussi permettent plus facilement de retrouver un peu de respiration financière vous dire aussi. Pour terminer. Que j'ai d'abord à coeur la mission que j'ai eu pendant quasiment 2 ans au service de l'économie sociale et solidaire que vous avez été nombreux, notamment sur la gauche de l'hémicycle. A rappelé la situation d'un certain nombre de nos compatriotes très fragilisée par la crise. Vous dire que, au même titre que nous avons été là avec des montants historique dans une situation très compliquée et notamment via le plan de relance, aux côtés des banques alimentaires le ministre-Combe a aussi annoncé hier une mobilisation de 60 millions d'euros à l'endroit des banques alimentaires Pour être très Direct que la Première ministre n'hésitera pas s'il faut faire plus pour accompagner nos associations qui accompagnent les plus fragiles. Pour ce qui est de ce débat, je vous en remercie et j'espère que j'aurai prochainement le plaisir d'de échanger avec vous sur ces sujets. Pour se battre ensemble pour faire baisser et contenir l'inflation que subissent nos compatriotes inflation forte mais inflation qu'il convient quand même de rappeler qu'il est bien moins forte que celle de nos voisins européens. Je ne sais pas si quand on sera pas on se compare on se rassure, où on se désole en tout cas, comme le disait Michelet c'est quand on se résigne que tout est perdu et compter sur moi je suis pas prête de me résigner, je vous remercie. Merci, madame la Ministre. Le 1er débat est donc clos avant de passer au 2ème point à l'ordre du jour. Je vais donner la parole à monsieur le questeur Vincent Capo Canellas pour une mise au point. Merci monsieur le président. Je fais de procéder à une rectification concernant le vote de mon collègue Hervé Maurey sur le scrutin, numéro 134 du 14 février 2023. Ce vote concerné, l'amendement 5 rectifier bis présenté par Monsieur Stéphane. Sautarel tendant à insérer un article additionnel après l'article IV. Cette. Il s'agissait d'une proposition de loi portant amélioration de l'accès aux soins. Par la confiance aux professionnels de santé. Monsieur Maurer souhaiter voter pour et non contre. Donc pour l'adoption de cet amendement, je vous remercie. Changement d'équipe. Bonjour, madame la Ministre. Ah bah oui, ah oui il faut partir même d'ici je sais. Oui. Ainsi va la vie. Selon Madame la Ministre. L'ordre du jour appelle l'examen de la proposition de résolution appelant à faire de la lutte contre les violences pornographique une priorité de politique publique présentée en application de l'article 34 1 de la Constitution par madame Annick Billon Alexandra Borchio-Fontimp, Laurence Cohen, Laurence Rossignol et plusieurs de leurs collègues demande du groupe Union centriste. Dans la discussion générale. La parole est immédiatement à madame la présidente Annick Billon, auteur de la proposition de résolution pour 3 minutes. Merci monsieur Monsieur le Président Madame la Ministre, mes chers collègues porno l'enfer du décor ou comment résumer en 5 mots. Le rapport choc que notre délégation aux droits des femmes a publié en septembre dernier mot d'une industrie licencieuses qui prospère en irriguant la toile de contenus illicites. Avec mes 3 collègues corapporteur Alexandra Borchio-Fontimp. Laurence Cohen, Laurence Rossignol. Nous avons pour la première fois dans l'histoire parlementaire enquêté pendant 6 mois sur la réalité des pratiques de l'industrie pornographique. Nous avons entendu toutes les parties prenantes dont à huis clos des victimes de l'affaire French Bukkake et cette affaire a permis de mettre au grand jour les pratiques de producteurs de barbares qui ont détruit la vie de dizaines de femmes. Nous avons analysé les principaux contenus disponibles sur les sites pornographiques. Ces plateformes en ligne les tubes qui propose gratuitement et sans aucun contrôle, des millions de vidéos. Il faut sortir de toute vision datée. Édulcoré du porno Le porno aujourd'hui ce sont des contenus violents et dégradants humiliants. Les scènes dans lesquelles un homme ou plus souvent des hommes infligent des violences physiques et sexuelles à des femmes sont devenus la norme. La pornographie n'est pas du cinéma. Les pleurs, les cris, les viols le sang il n'y a pas d'effets spéciaux, tout est vrai. Ce sont ces violences et leur banalisation qui nous ont amenés à prendre des positions fortes. Notre rapport a eu un écho médiatique considérable en France et à l'international, suscitant une onde de choc dans l'opinion. Le nombre de co-, signataire de cette proposition de résolution 255 exactement

Ce chiffre témoigne d'une prise de conscience collective. Plus que d'inviter il engage le gouvernement à mettre en oeuvre les recommandations que nous avons formulées la ministre à qui nous avons présenté le rapport nous ont assuré vouloir avancer sur ce sujet je pense bien sûr à la su lotion de contrôle d'âge annoncé récemment par Jean-Noël Barrot et Charlotte Caubel, ainsi qu'à toutes les mesures de politique pénale qui permettront de poursuivent les auteurs et diffuseurs. La massification de la production et de la consommation nous oblige. Je sais pouvoir compter sur vous, madame la ministre, vous partagez notre détermination nos propositions sont sur la table. Le gouvernement doit s'en saisir, je vous remercie. Merci. Madame la présidente. La parole est maintenant madame la présidente Laurence Rossignol, auteur de la proposition de résolution pour 3 minutes. Monsieur le président. Madame la ministre. Madame la présidente de la délégation aux droits des femmes. Chers collègues, je vais pour ma part évoqué le de la dimension industrielle du pour nous, nous avons effectivement voulu que notre rapport s'intéresse à l'industrie pornographique, pas simplement à l'effet du porno à qui en consomment toute la chaîne qui part du recrutement des méthodes de tournage des méthodes de diffusion, puis de l'influence sur les cerveaux et la société sur les jeunes, comme sur les adultes car le porno c'est d'abord une industrie mondialisée qui génère plusieurs milliards d'euros de profits chaque année concentré dans les mains de quelques grandes multinationales souvent basées dans des paradis fiscaux, la production massive de contenus pornographiques et de plus en plus. Violentes ces contenus sont violents sont extrêmes et la production et de plus en plus volumineuses, elle alimente ce monde ce business mondiale et génère un trafic vidéo prépondérance sur Internet les vidéos pornographiques hébergés sur des plateformes de streaming constitue ainsi plus d'un quart de tout le trafic vidéo en ligne du monde. La demande de contenus pornos sur Internet correspond quant à elle à une à une recherche sur huit quand il s'agit d'un ordinateur et une recherche sur cinq quand il s'agit d'un mobile et ne nous voilons pas la face. Mes chers collègues. Nos recherches statistiques ont montré que la France est un des pays les plus consommateurs de pornographie au monde le porno c'est aussi une industrie qui, par sa nature même est génératrice de violence systémique envers les femmes. N'oublions pas la définition de la pornographie. Il s'agit de l'exploitation commerciale de la représentation explicite d'actes sexuels non simulés. Or d'après les chiffres publiés notre rapport 90% des scènes pornographiques porte des violences sexuelles physiques ou verbales, ces violences ne sont pas simuler mais sont bien réelles pour les femmes filmées. Nous avons également constaté au cours de nos travaux une grande porosité entre l'univers pornographique et l'univers de la prostitution. Ce sont 2 mondes entrent lesquels les passerelles sont nombreuses et qui utilise des méthodes de recrutement similaire pour exploiter sexuellement les mêmes femmes vulnérables économiquement, socialement et souvent psychologiquement. Enfin le porno est une industrie qui fait maintenant l'objet de poursuites pénales. Enfin il était temps. Pour la première fois en France des violences commises dans un contexte de pornographie sur des femmes victimes de graves maltraitances sexuelles physiques et psychologiques font l'objet d'un traitement pénal. Les auteurs de ces violences sont poursuivis pour viol viols aggravés, complicité de viol avec actes de torture et de barbarie traite des être s'humains enfin de viols, proxénétisme. Voilà la réalité de cette industrie aujourd'hui. C'est pourquoi nous appelons à faire de la lutte contre les violences pornographique une priorité de politique publique. L'omerta qui pèse sur ces violences doit cesser. Il est temps de mettre un terme au déni à la complaisance dont bénéficie cette industrie depuis trop longtemps et pour cela nous avons Madame la Ministre besoin de votre engagement à nos côtés, nous savons que déjà ce sujet vous. Et nous espérons beaucoup de l'ensemble du gouvernement, enfin ma collègue parlera dans quelques instants de l'influence du porno sur les jeunes cerveaux. Je voulais dire que le porno n'est pas toxique que pour les adolescents. Le porno est toxique pour l'ensemble des consommateurs de porno, y compris pour les adultes. Pour ces hommes qui sont devenus addict au porno et ne sont plus capables d'avoir une sexualité réelle tant ils sont motivés et excité exclusivement par les scènes violentes qu'ils voient sur internet. Merci madame la présidente. Là. La parole est maintenant à madame Alexandra Borchio-Fontimp, auteur de la proposition de résolution pour 3 minutes.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues co-rapporteurs chers collègues. Porno l'enfer du décor. Un jeu de mots pour arrêter de jouer avec les plus fragiles et pour dénoncer les conséquences de la massification des contenus pornographiques des consommateurs toujours plus nombreux, de plus en plus jeunes en demande de contenus de plus en plus violents extrême et dégradant. Ce sont aussi les conséquences de l'accoutumance. Mais jusqu'où ira cette surenchère malsaine une escalade infernale pour tenter d'assouvir une curiosité qui finalement n'est jamais comblé et ce, sans considération pour les conditions dans lesquelles ces contenus sont produits. 2 tiers des moins de 15 ans et un tiers des enfants de moins de 12 ans ont déjà eu accès à des images pornographiques triste réalité lorsqu'on sait que l'Exposition des mineurs à ce type de contenus s'inscrit en parfaite violation du code pénal car comme vous le savez depuis la loi du 30 juillet 2020 à l'initiative de notre collègue Marie Mercier que je veux saluer pour ses travaux sur ce sujet précis les sites pornographiques ont l'obligation de s'assurer de la majorité de l'internaute qui les consultent et pourtant tous les sites pornos demeure accessible en un clic, sans aucune vérification d'âge tout comme les réseaux sociaux, devenu aujourd'hui le support social de référence des nouvelles générations sur lesquels de nombreux comptes affichent des contenus pornographiques violents, bien loin de la réalité et qui ont pour conséquence de banaliser ces pratiques sexuelles comme si elles étaient la norme se poser des questions sur la sexualité. Quand on est à l'école primaire est une curiosité finalement naturelle qui fait partie de son développement. En revanche, aller chercher des réponses sur les plateformes numériques qui proposent des contenus inadapté avec leur maturité et absolument pas représentative de la réalité pose un sérieux problème là aussi il y a un effort à fournir en matière de prévention afin de sensibiliser les enfants et les parents aux dangers de la pornographie et de la marchandisation du corps. Les conséquences sur la jeunesse de cette Exposition massive au porno sont plus que préoccupante et elle ne se limite pas qu'aux mineurs bien sûr le porno peut également avoir un impact dangereux sur les adultes sur leur représentation de même des femmes et de la sexualité. Face à ce constat alarmant. Il est donc urgent d'agir dans notre rapport, nous avons proposé notamment la mise en place d'un dispositif d'attestations de majorité reposant sur un principe de double anonymat. Plus que des annonces. Nous attendons maintenant des actes forts Madame la Ministre, mes chers collègues avec Annick Billon Laurence Cohen et Laurence Rossignol. Nous avons abordé ce sujet tabou, parce qu'il nous a semblé. Nous avons entendu à huis clos des témoignages glaçants surréaliste de victimes de violence mais aussi d'adolescents dans un collège à quelques encablures d'ici qui considère que le corps peut être une monnaie d'échange. Il est temps d'ouvrir les yeux et d'agir pour que notre pays ne soit plus complice de cette triste réalité avant qu'il ne soit trop tard pour rectifier. Merci cher collègue. Là. Par les maintenant madame Laurence Cohen, auteur de la proposition de résolution pour 3 minutes. Monsieur le Président Madame la Ministre, mes chers collègues porno l'enfer du décor. La délégation aux droits des femmes du Sénat et aujourd'hui le Sénat tout entier peuvent être fiers de ce rapport. Un véritable pavé dans la mare lancé il y a quelques mois, y aura notamment permis de mettre à l'agenda du gouvernement. Le sujet des pratiques de l'industrie pornographique et de ces violences. Il aura aussi contribué à sensibiliser l'opinion publique à ces violences et à les mettre au coeur du débat public. De ce point de vue, nous pouvons considérer que notre rapport pionniers à beaucoup d'égards est une réussite en soi. Au delà de cet écho médiatique et populaire, nous attendons aujourd'hui des avancées concrètes suite au 23 recommandations formulées dans notre rapport. Je rappelle rapidement les 4 grands axes de ces recommandations, Premièrement, faire de la lutte contre les violences pornographique une priorité de politique publique et pénal. Deuxièmement, faciliter la suppression de contenus pornos pornographique illicite et l'exercice du droit à l'oubli. Troisièmement, bloquer l'accès des mineurs au contenu pornographique à cet égard nous nous félicitons des récentes annonces du gouvernement concernant la mise en place dès le mois de mars d'un dispositif technique opérationnel de vérification d'âge reposant sur le principe du double anonymat tels que celui que nous avions proposé dans notre rapport. Et que vient de rappeler notre collègue Alexandra à bord Kyo Fontin. Enfin 4ème et dernier axe de nos recommandations. L'éducation des jeunes à la sexualité et la sensibilisation des parents, des équipes pédagogiques et des professionnels de santé aux dangers de l'Exposition à la pornographie des enfants et adolescents. Globalement, nous pensons qu'il est nécessaire de mettre en oeuvre un plan interministériel de lutte contre les violences pornographiques avec des mesures fortes dans les 4 domaines que je viens de citer. Pour mettre en oeuvre un tel plan. Il faudra bien sûr des moyens importants adapté et nouveau notamment un renforcement de l'arsenal pénal des effectifs et des moyens matériels, mis à disposition des services enquêteurs et des magistrats. À traiter des violences commises dans un contexte de pornographie. Nous sommes également favorables à l'exploration de toutes les mesures fiscales permettant de taxer l'activité de l'industrie pornographique, marché extrêmement rentable qui génère des milliards d'euros de profits chaque année. Bref, nous revendiquons sans détour un pouvoir de nuisance à l'encontre de cette industrie aussi puissante que néfastes. Unissons nos forces dans ce combat pour que ces son sein les violences systémique induite par les pratiques de cette industrie, c'est l'une des conditions pour bah. Une société d'égalité entre les femmes et les hommes. Nous sommes toutes et tous concernés et nous pouvons être fiers d'examiner aujourd'hui cette proposition au Sénat, je vous remercie. Merci cher collègue là dans la suite de la discussion générale. La parole est maintenant Madame Véronique Guillotin pour le groupe RDSE pour cinq minutes. Monsieur le président, madame la ministre, madame la présidente de la délégation aux droits des femmes cher Annick. Mesdames les auteurs de la proposition de résolution, mes chers collègues, pour reprendre un constat évident du rapport d'information de mes collègues Annick Billon Alexandra Borchio-Fontimp Laurence Cohen et Laurence Rossignol. Le milieu de la pornographie est aujourd'hui est avant tout un Business et un Business qui peut rapporter gros. À l'instar de secteurs qui situe souvent au-delà de la légalité. Qu'on pense à la prostitution aux trafics en tout genre, il est difficile d'obtenir des statistiques précises sur l'ampleur et les caractéristiques du phénomène. On sait toutefois que les volumes d'affaires se chiffrent en milliards d'euros. aujourd'hui d'un secteur concentré dans les mains de quelques plateformes de diffusion à l'échelle mondiale, ça a été dit souvent d'origine nord-américaine mais dont les sièges sociaux peuvent être établies dans des paradis fiscaux et qui se caractérise souvent par une certaine opacité financière. La diffusion et la et la consommation de contenus pornographiques et massive représentant le quart de la bande passante d'Internet les plateformes dites pour adultes font partie des sites les plus consultés comparable aux grands moteur de recherche aux réseaux sociaux aux grands médias et La France occupe je dirais hélas la 4ème place mondiale dans la consommation de contenus pour adultes. Les critiques sur l'évolution de l'industrie pornographique ne sont pas nouvelles en ce qui concerne ses effets sur le consommateur, notamment les plus jeunes mais pas que, qu'il soit volontaire ou accidentelle mais ces critiques ont pris plus récemment un tour dramatique avec la révélation d'abus particulièrement grave en France même sur des jeunes femmes lors de réalisation de tournage dit des tournages amateur. La massification et la banalisation de la pornographie peuvent entraîner la recherche de contenus toujours plus inventifs et par conséquent des pratiques de plus en plus extrême, voire violente sans le consentement réel des personnes. Nous devons donc nous interroger davantage sur les conditions de production des contenus pour adultes et sur les règles qui devrait encadrer ces productions par exemple en imposant des médiateurs du consentement ou des dispositifs comparables. Il ressort des travaux de la délégation aux droits des femmes que ces abus touchent particulièrement l'industrie dite amateur réalité qui cache en fait l'absence totale de garantie pour les jeunes femmes car ce sont elles, le plus souvent les victimes et une organisation digne des labels les plus établis la pornographie dites professionnelle n'est pas pour autant, exempt de critiques, on sait de longue date que les conditions de travail hein. Lors des tournages et les conditions sanitaires les plus élémentaires ne sont pas respectées. C'est un point important qui ressort des auditions menées l'année dernière, les actrices qui refusent d'être assimilés à des prostituées demande à être reconnus en tant qu'actrice, et à ce que leur profession puisse s'organiser de façon à mieux défendre leurs droits au moyen par exemple de syndicat interprofessionnel d'agence au même titre que pour les acteurs classiques en tant que co-, signataire de la proposition de résolution qui fait l'objet d'un consensus transpartisan. Je me permets d'attirer l'attention sur ce point. J'en viens maintenant au 2ème axe de la problématique, l'effet de la pornographie sur le public qu'on le veuille ou non, la pornographie, la pornographie, occupe aujourd'hui une place importante sans pour autant qu'il faille la considéré comme un produit de consommation classique en ce qui concerne les mineurs. L'accès à la pornographie est problématique dans la mesure où ces contenus leur sont interdits par la loi. Le contrôle de l'âge est une difficulté réelle, un dispositif de certification de l'âge est en cours d'élaboration pour une mise en oeuvre cette année je rappellerai pour ma part la loi du 2 mars 2022, visant à renforcer le contrôle parental sur les moyens d'accès à Internet adopté adopté avec succès il y a un an, est ce que l'on sait si d'ores et déjà, cette loi a produit ses effets. L'accès des adultes à la pornographie est quant à lui autorisé en France et plus largement dans les pays occidentaux mais souvent interdit ou limité dans le reste du monde. Toutefois les effets de la pornographie sur les les adultes ne devrait pas être négligée. Pour autant, soit parce qu'ils y sont confrontés pendant l'adolescence, soit parce qu'elle contribue encore à donner une vision déformée la sexualité. Enfin, les adultes ont naturellement une responsabilité dans leur propre usage de la pornographie et dans les conseils qu'ils doivent apporter aux mineurs on évoque là le sujet de l'éducation. En conclusion, convaincu de la nécessité d'agir plus efficacement pour lutter contre les dérives de cette industrie, les membres du du RDSE voteront pour l'adoption de cette proposition de résolution.

Madame la Ministre, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui la proposition de résolution de nos collègues Annick Billon, que je salue, Alexandra Borchio-Fontimp, Laurence Cohen et Laurence le signale que je sais lui aussi toutes les quatre, appelant à faire de la lutte contre les violences pornographique une priorité de politique publique que nous sommes nombreux à avoir cosigné. La pornographie est partout et accessible d'un seul clic-t-elle un produit de consommation courante. Le marché est si peu régulé, qu'il suffit de répondre à une question simplissime, avez-vous plus 18 ans pour accéder à des contenus sensibles que l'on soit mineur ou majeur. Une réponse positive permet d'entrer dans l'univers sordide des vidéos porno tournés avec des actrices parfois vulnérable qui n'aurait jamais consenti à l'acte sexuel si elles avaient été informés des conditions de tournage et des pratiques que ce milieu ignorant de la dignité humaine leur impose. Qu'importe le respect dû à la femme et à son intégrité physique, devenu de la Chair à canon pour des pornocrate, des pornocrate sans scrupule. Elle doit contribuer à leur fortune personnelle et à leur gloire. Certains fatalistes banaliser la pornographie en affirmant qu'elle n'est finalement qu'une version modernisée de la sexualité. Et c'est là que le bât blesse car la pornographie aussi répondu soit-elle, ne peut être assimilée à la sexualité qui est un découverte partager mettant en scène une intimité complice. Plusieurs chercheurs auditionnés par notre délégation nous ont confirmé que ces vidéos ont une influence certaine sur les pratiques des adolescents à travers leurs normes corporelles et les diktats qu'elle impose pire et véhicule la culture du viol dans un contexte où l'éducation à la sexualité dans le cadre scolaire est quasi inexistante. Dans certains cas la consommation de contenus pornographiques peut conduire à des traumatismes psychologiques et psychiques et physiques graves auxquelles concourent également les réseaux sociaux numériques comme Instagram ou je n'Snapchat. Snapchat ou l'image des corps dénudés et banalisé et le Revenge porn, une pratique courante. De mon point de vue la réponse à ce phénomène est double. Éduquer pour mieux protéger et réprimer pour mieux réguler. Protéger nos jeunes contre les contenus inappropriés par la prévention et l'éducation est en effet la première réponse à apporter à ce fléau de la pornographie en libre accès. Le rôle des parents et décisif. Je pense en particulier à la mise en oeuvre du contrôle parental pour les plus jeunes qui possèdent souvent un smartphone dès l'âge de 10 ans. Celui de la communauté éducative et des associations est également très important non seulement pour encadrer les bonnes pratiques informatiques mais également pour délivrer à nos adolescents une information Perpignan pertinentes sur la sexualité et c'est pratique. Si les enjeux de prévention sont majeurs, ils ne sont cependant pas traité avec suffisamment de détermination et de moyens humains aujourd'hui dans notre pays. La seconde réponse peut être apportée à travers la mise en oeuvre d'une politique coercitive beaucoup plus forte à l'égard des éditeurs de contenus. Agir sur le terrain juridique et renforcer les outils techniques sont certainement le meilleur moyen de réguler l'accès à la pornographie. La loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales a constitué une étape importante en matière de lutte contre les contenus portant pornographique. Je tiens ici à saluer l'engagement ferme et constante de notre collègue Marie Mercier sur ce sujet essentiel de la protection de l'enfance. C'est à l'Arcom qu'incombe désormais la responsabilité de faire respecter l'interdiction de l'accès des mineurs aux sites pornographiques. Et si récemment employé en mettant en demeure plusieurs plateformes de rendent leur contenu inaccessible puis en saisissant le président du tribunal judiciaire de Paris pour obtenir le blocage de l'accès au site et leur déférence ment. Les éditeurs concernés se sont lancés depuis dans une bataille juridique acharnée afin de protéger leur activité et le revenu l'indécence n'a décidément pas de limites. Il faudra sans aucun doute, comme le propose la délégation aux droits des femmes, renforcer les pouvoirs de l'Arcom. Par exemple on insère montant ces agents afin de leur permet de constater eux-mêmes les infractions des éditeurs de contenu sensible la possibilité de prononcer elle rencontre des sanctions administratives avec des montants dissuasif est aussi parfaitement envisageable. Dans ce contexte, je me réjouis de l'annonce récente par le gouvernement du test prochain d'un dispositif technique reposant sur le principe du double anonymat destiné à vérifier l'âge des internautes. Une telle solution plus performantes que celles actuellement proposées par les éditeurs de contenus serait de nature à répondre aux recommandations de notre délégation. Enfin, nous devons avoir conscience du rôle pivot de l'éducation nationale et de la nécessité d'aborder dans le cas de séances d'éducation à la vie sexuelle et affective des sujets relatifs à la marchandisation des corps et à la pornographie. De même, ça aurait été judicieux de recruter plus de professionnels formés en matière d'éducation à la santé dans les établissements scolaires. C'est à ces conditions que nous pourrons faire échec aux violences pornographique et permettront à nos enfants et adolescents de vivre sereinement le passage progressif vers l'âge adulte. Compte tenu de l'importance des enjeux de la nécessité d'agir sans délai contre ces violences. Je voterai en faveur de la proposition de résolution qui nous est soumise. Je vous remercie. Merci cher collègue. Là. La parole est maintenant monsieur Pierre vielle pour le groupe les indépendants pour cinq minutes. Monsieur le Président Madame la Ministre, mes chers collègues. Quel parent ne s'est jamais interrogé sur le type de contenu auquel son enfant a versé sur Internet. Parmi les contenus qui inquiète. Il y a évidemment ceux à caractère pornographique. Ils s'inquiètent car la plupart des parents veulent protéger leurs enfants de ce type de vidéos. Tout en sachant que l'accès à ces contenus volontaire au monde relève justement bien trop souvent d'une simplicité enfantine. Ce qui interroge en revanche beaucoup moins ce sont les conditions de tournage de ces vidéos. Pourtant parfois excessivement violentes notamment envers les actrices. Quiconque consulter le rapport d'information du Sénat pour l'enfer du décor n'a pu être que bouleversé perturbé à la lecture de certains témoignages de victimes. Certains font clairement état d'un système organisé, d'abus de faiblesse, de viols et d'actes de torture et de barbarie. Je souhaite ainsi salué le travail des rapporteurs qui a permis de mettre en lumière les dessous très tabou de milieu qui l'est tout autant. La pornographie constitue déjà en elle même, un genre de cinéma très particulier dans lequel les actes les plus intimes ne sont ni simuler ni fin mai reproduit. Et lorsque ces actes incluent des pratiques très violentes, voire déshumanisante. Non consentie. On ne peut plus du tout parler de cinéma. Le sujet que nous abordons aujourd'hui n'est pas celui d'être pour ou contre la la pornographie mais celui de condamner totalement et formellement toute forme de violences commises à l'encontre des acteurs et des actrices de cette industrie. Ces dernières années le secteur amateur s'est considérablement développée. Notamment en raison du développement des réseaux sociaux des messageries privées. Et des plateformes gratuites. Entièrement dédié à ce type de compte-tenu. Pratiques sexuelles imposées rapports forcés nombre de partenaires excessif les tournages se font parfois dans des conditions inhumaines. Si certains producteurs tentent de mettre en place des pratiques différentes respectueuse des actrices et des acteurs de leur dignité. De leur consentement et de leurs conditions de travail. Ces pratiques restent malheureusement encore très minoritaires. Nous souhaitons également affirmé notre volonté de renforcer la protection des mineurs. Face à ce type de contenu car. Si le code pénal interdit leur accès aux mineurs. Il serait illusoire de prétendre que telle n'est pas le cas en pratique. Une simple déclaration de majorité suffit pour accéder aux sites pour adultes. 62% des adolescents ont déjà vu des images pornographiques avant 15 ans et 31% avant 12 ans. Plus inquiétant encore, un enfant de primaire sur deux il y a déjà été exposé. Au-delà d'une simple déclaration un véritable contrôle de âge devrait être assuré avant l'accès à tout, compte tenu pornographique. C'est là un point crucial. Comment s'assurer de l'âge de l'internaute. Tout en respectant la confidence. Confidentialité pardon des données à caractère personnel. La piste principale proposée par le pérenne et la CNIL pour les sites pornographiques, mais aussi plus largement à tous soumis à une obligation n'vu vérification. Vise à ce qu'il ne réalise pas eux-mêmes cette vérification. Elle devra s'appuyer sur des tiers de confiance banque fournisseur d'énergie. Dont la validité aura été vérifié de manière indépendante. Aucun système cependant ne sera parfait et aucun ne sera elle détourna bleu. Il s'agira de trouver la la moins mauvaise des solutions pour protéger les mineurs. Et cette solution devra nécessairement s'inscrire dans le cadre d'un débat démocratique. Enfin. Et parce que l'actualité nous y renvoie. Il faut renforcer les moyens permettant de lutter contre la pédopornographie. Comment est-il possible que de tels contenus sont encore disponible aujourd'hui. En 2021, la plateforme Pharos empêcher plus de 3 millions de consultations. Dont 90% concernaient du contenu à caractère pornographique. Mais combien de compte tenu de ce type sont encore librement accessibles. Nous appelons. À un renforcement de l'arsenal pénal des effectifs et des moyens permettant de lutter contre toute forme de violence pornographique et de diffusion de contenus illicites. Nous espérons que cette proposition de résolution. Donnera lieu à des mesures concrètes. Et le groupe les indépendants votera bien sûr en faveur de cette proposition de résolution. Merci cher collègue. La parole est maintenant à madame Monique de Marco pour le groupe écologiste pour cinq minutes. Monsieur le Président Madame la Ministre, mes chers collègues. À quoi bon éduquer. Les enfants à la notion du consentement si des contenus pornographiques mettant en scène des adultes. Qui en sont privés, leur sert de lieu d'apprentissage de la sexualité par défaut, selon les termes de cette résolution. Contrairement aux fantasmes véhiculés par ces contenus. Les faits judiciaires à l'origine de cette initiative sont bien réelles. Dès 2020, plusieurs tests de viol. d'être plainte traite d'être humains et actes de torture liés à des actes commis sur des plateaux et hors des plateaux de tournage ont été déposées. Ces plaintes sont toujours en cours d'instruction. Le Sénat s'est saisi de la question, donnant lieu à la publication d'un rapport d'information en septembre dernier et je tiens à saluer l'initiative ne mes quatre collègues. Au moment de sa publication déjà certains représentants du secteur y'du travailleurs du sexe ont mis en avant la possibilité d'une régulation alternative et la nécessité de distinguer la pornographie, de la violence. Bien que de jeunes production offre des contenus destinés à un public plus large est désormais féminin moins marquée par des rapports de domination. La marginalisation du secteur ne permet pas de garantir une protection satisfaisante pour les personnes engagées de part ses productions. Il est donc urgent de s'assurer que de droit existant soit correctement appliquée au regard surtout du hein. C'est c'est continue sur les mineurs. Il est vrai que les images véhiculant les rapports de domination ne relève de. Pas des seuls contenus pornographiques. Mais ce secteur doit comme les autres prendre ça, pas de responsabilité alors que de qui a des enfants de moins de 15 ans, il y a un tiers des enfants de moins de 12 ans ont déjà eu accès à de tels contenus. On observe en outre un Net retour des perceptions sexy. Les jeunes générations. Selon le rapport du Haut Conseil à l'égalité, 23% des jeunes de 25 à 35 ans, estime qu'il faut parfois être violent pour être respecté en tant qu'homme. Et l'image des femmes véhiculée par la pornographie est jugée problématique par seulement la moitié d'entre eux. Par ailleurs les travaux de la mission de. Ont permis de mettre, de faire le constat des faibles moyens d'action de l'Arcom. Lors d'une audition à la commission culture en septembre dernier j'avais interrogé le président de l'Arcom sur ses capacités de mettre en place un écran noir en l'absence de vérification de la majorité de l'utilisation du site et de disposer d'agents assermentés pour constater les infractions. Question restée sans réponse. Le président de l'Arcom, a mis en avant des campagnes de communication et signalétique. Celle-ci me paraissent totalement insuffisante. C'est pourquoi, avec d'autres de mes collègues du groupe écologiste. J'ai signé cette proposition de résolution. Il s'agit également de poursuivre la réflexion législative qui s'est ouverte depuis plusieurs années sur l'existence de violences sexuelles et sexistes structurelle ce M. dans notre société et les moyens de mettre en place pour les empêcher. Une répétition générationnel. Sans verser dans le prohibitifs me 3 pistes devraient être examiné en priorité. Premièrement, il importe de s'assurer que les contenus soient produits dans des conditions légales et respectueuse du droit du travail et des personnes et de la dignité humaine et que les manquements donne lieu à des sanctions adaptées. Il y a un accompagnement des victimes. Une réflexion pourrait sourire également sur le soutien aux productions plus respectueuse des droits des personnes dans l'esprit des travaux législatifs conduit sur la prostitution. Deuxièmement, il aime pas de garantir que les contenus pour adultes soient réservés aux adultes. Autrefois le filtre était assuré par un contrôle physique des distributeurs de films à l'entrée des salles de cinéma par exemple et dans les vidéos clubs. L'époque a changé. La digitalisation nécessite. D'adapter les outils de régulation dans le respect bien sûr de la protection des données personnelles. J'espère que le gouvernement parviendra rapidement un dispositif efficace. En s'inspirant par exemple du modèle de la Louisiane. Troisièmement, il faut impérativement renforcer l'éducation à la sexualité qui nécessite d'importants moyens humains et matériels et ça c'est le rôle de l'éducation nationale. Il me semble. Important de rappeler que la consommation de pornographie n'est qu'un aspect de la liberté sexuelle quand des moyens de vivre, ses fantasmes et qu'il existe des sexualités heureuse sans y avoir recours. Dans Totem et Tabou Freud écrivez que le besoin sexuel loin d'unir les hommes les divise. J'espère que nous pourrons parvenir à dépasser ses divisions pour parvenir à une régulation de toute la pornographie respectueuse de toutes sexualité et de toutes les dignités. Je vous remercie. Merci cher collègue. Là. La parole est maintenant Madame Samantha Cazebonne pour le groupe RDPI pour six minutes. Monsieur le Président Madame la Ministre, mes chers collègues, le rapport annuel 2023 sur l'état des lieux du sexisme en France et marquant 48% des hommes entre 15 et 34 ans, considère que l'image des femmes véhiculée par les contenus pornographiques est problématique, ce chiffre monte à 79% des hommes âgés de 65 ans et plus, soit 30 points d'écart. Ce constat est alarmant surtout quand on le regarde à l'aune d'un autre chiffre 90 pour des scènes pornographiques comporte de la violence. Comment se fait-il que des images de violence choc moi les jeunes. Comment agir contre le sexisme en France dans toutes les sphères où ce dernier existe. Comment protéger mieux les femmes aujourd'hui. Dans ce contexte, la délégation aux droits des femmes a réalisé un rapport d'information sur les pratiques de l'industrie pornographique. C'est la première fois qu'un tel travail réalisé et nous ne pouvons que nous en féliciter, car pour endiguer un phénomène de violence pour protéger les femmes qui en sont victimes, pour encadrer une industrie qui représente 25% du trafic web de vidéos dans le monde. Il faut en comprendre les acteurs les enjeux les limites et les risques ce travail parlementaire nous permet aujourd'hui d'avoir une vision plus claire des mesures à prendre pour avancer vers une meilleure protection des femmes et des mineurs face aux violences pornographique existantes. C'est tout l'objet de la proposition de résolution qui nous est aujourd'hui soumis et que j'ai souhaité cosigné avec plusieurs de mes collègues. Dans une ou les vidéos se diffuse en quelques secondes aux 4 coins du monde les régulation d'accès sont rendues difficiles par les contenus disponibles en quelques clics. Les mesures protectrices sont recherchés par nombre d'entre nous. C'est ainsi que l'année dernière. La loi proposée par notre collègue député Bruno Schröder visant à conforter à renforcer le contrôle parental sur les moyens d'accès à Internet a été promulguée, elle rend obligatoire la pré-installation d'un dispositif de contrôle parental sur les appareils connectés vendus en France l'activation de ce dispositif devrait être proposé gratuitement à l'utilisateur lors de la première mise en service de l'équipement. Le gouvernement s'est également engagé sur le sujet avec notamment l'objectif de mieux protéger les mineurs. Face à ces contenus. C'est ainsi qu'une campagne gouvernementale sur le site je protège mon enfant et les dispositifs de contrôles parentaux a été lancé il y a quelques semaines. Cette plateforme d'information, de prévention et de protection des mineurs contre l'Exposition aux contenus pornographiques en ligne propose des outils, des conseils et des ressources pratiques pour mieux informer les parents afin qu'ils protègent leurs enfants. De plus, le rapport commandé par le gouvernement concernant l'éducation à la sexualité a été publié en 2021 et permet d'avoir un état des lieux dans la mise en oeuvre de cette politique publique. Il préconise notamment d'inscrire des notions d'éducation à la sexualité dans les programmes de certaines disciplines appartenant au domaine des sciences humaines, économiques et sociales et lié à l'éducation de la sexualité. Enfin un travail commun est actuellement menée par Jean-Noël Barrot et Charlotte Caubel pardon sur la vérification d'âge par le biais de l'attestation numérique Il a été annoncé le lancement en mars d'une expérimentation visant à trouver une solution de vérification de l'âge des internautes en double anonymat. Cette annonce fait suite à un avis de la CNIL sur ce sujet il s'agira donc de s'assurer de la mise en oeuvre d'un outil protecteur des mineurs mais également de la vie privée et des données personnelles de chacun. Comme tout travail sur ces enjeux centraux. Il faut donc parvenir à l'équilibre. Il me semble que c'est l'objet de la proposition de résolution protégé avec justesse. Cette dernière prévoit donc tout d'abord de demander une prise de conscience collective de la réalité des pratiques de l'industrie pornographique et de leurs conséquences. C'est un objectif essentiel, le texte vise également à faire de la lutte contre les violences que cette industrie génère et véhicule une priorité de politique publique et pénales à mieux informer accueillir et protéger les victimes de violences commises dans un contexte de pornographie en particulier en formant les forces de l'ordre et les intervenants du numéro national 39 19. A recommandé la création d'une catégorie violences sexuelles sur la plateforme. Pharos que vous connaissez, afin de faciliter et de mieux comptabiliser les signalements. À protéger la jeunesse en bloquant tous sites ou réseaux proposant des contenus pornographiques sans exiger une preuve de majorité des utilisateurs à plaider pour une généralisation des dispositifs de contrôle parental et de navigation sécurisée qui pourrait être activé par défaut. Dès lors qu'un abonnement téléphonique est souscrit pour l'usage d'un mineur et enfin alerter sur la nécessité d'appliquer les 3 séances annuelles d'éducation à la vie affective et sexuelle et la nécessité d'aborder lors de ces séances, les sujets relatifs à la marchandisation des corps et de la pornographie. Cette proposition de résolution vise ainsi à aller au-delà d'un mot connue de tous, la pornographie, ce dernier utilisait d'ailleurs trop souvent par les mineurs qui ont parfois accès à ces contenus, avant même d'en apprendre davantage sur les notions de consentement de sexualité et les problématiques liées à ces dernières. Le texte, en s'attachant à trouver une réponse exhaustive temps sur l'information, le contrôle, la formation et la protection des plus fragiles, nous apparaît d'importance c'est pour ces raisons que le groupe RDPI votera en faveur de cette proposition de résolution merci. Merci monsieur le président, madame la ministre, madame la présidente de la délégation aux droits des femmes, mesdames les rapporteurs, mes chers collègues perversion partout respect nulle part l'industrie pornographique organise un monde parallèle où le spectacle de violence de sévices et de viol est la norme. La pornographie s'est infiltré partout dans notre société et installe dans les esprits une vision sordide de la sexualité, c'est une activité économique extrêmement lucrative. Autrement dit, une machine à cash générant dans le monde des milliards d'euros chaque année. Ce qui est plus qu'alarmant. Ce sont les taux d'Exposition des mineurs à des images pornographiques ces massif est proprement hallucinant avant 13 ans, bien plus que le tiers des garçons et plus du quart des filles avant 18 ans les chiffres nous donne le vertige. La quasi-totalité des garçons 95% et une très large majorité des filles 86% rappelons-le, la loi interdit l'accès des mineurs au contenu pornographique pour le coup, nous sommes très très loin du compte. S'agissant du respect de la loi. Les effets dévastateurs sur les comportements des enfants sont d'ores et déjà constater multiplication des attouchement et harcèlement sexuel dans les collèges et les lycées visionnage subit parce qu'imposer de vidéos pornographiques. Les filles constituant bien sûr la majorité des victimes et ceci se passe dans l'ignorance quasi totale des parents si un témoignage ou une affaire est révélée ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. N'oublions pas que quasiment tous les enfants ont vu des vidéos pornographiques avant 18 ans. Les effets du porno sont absolument toxiques sur les esprits, à fortiori sur les plus jeunes, chez les adolescents. La rencontre avec la brutalité du porno précède la construction de l'imaginaire sexuel, l'enfant peut être profondément choqué et dans l'incapacité d'analyser ce qui l'a vu, c'est tous les possibles des rapports amoureux qui peuvent être balayés. Attirance séduction c'est et je le dis avec force parce que c'est grave. Une violence psychique qui constitue une blessure à vie infligées aux enfants en ne les protège protégeant pas dès qu'on ait les conséquences sont délétères, notamment de nombreux troubles et traumatismes et surtout comme un apprentissage au non-consentement s'ajoute à cela que les contenus sont de plus en plus violents. Il ne semble pas y avoir de limites apologie du viol de l'inceste et tout un panel de déviance sexuelle. Un nombre non négligeable de consommateurs vont développer une addiction entraînant une accoutumance à des contenus de plus en plus violents érigeant la domination masculine en modèle dans une escalade sans fin 90% des scènes pornographiques sont violentes, voire ultraviolente. Elles peuvent être qualifiées d'actes de torture et de barbarie et de traite d'être s'humains. Beaucoup de femmes recrutées sont trompés abusés et vont être filmé, alors qu'elles sont violentées blessées violées. La réalité c'est qu'elles ont été piégées n'ayant aucune idée de la violence inouïe des actes sexuels qu'elles allaient subir la rapide évolution de l'industrie pornographique tirée par le développement d'Internet à créer des opportunités pour des acteurs sans scrupules bâtissons des fortunes alors que les pouvoirs publics sont restés aveugles et sourds des hein des empires se sont créés insaisissable et d'une certaine manière par l'absence de réglementation de cadres du surveillance résultat une réalité parallèle où prospèrent l'esclavage sexuel dont la valeur marchande constitue une forme de barbarie contemporaine ce monde semble échapper à toute poursuite à toute sanction. Quant aux femmes victimes, elle se trouve dans la quasi-. Impossibilité de demander justice pour ce qu'elles ont subi. Si quelques affaires ont été. Dévoilant l'ampleur du phénomène. Nous sommes pourtant devant le constat effrayant des chiffres, 19 millions de visiteurs par mois en France dont 17 millions d'adultes et 2 millions d'adolescents. Un marché colossal, provoquant un appel d'air à l'arrivée de nouvelles vidéos sur les plats fort sur les plateformes pour répondre à la demande, marché qui de plus connaît une dérive sans précédent en créant une passerelle avec une forme de proxénétisme très particulier, celui du viol sur commande une femme pensant elle participer au bout. Tournage d'une vidéo pornographique. La lutte est vraiment inégale devant l'accélération du phénomène. Quelle société résultera demain de notre inaction et du manque de protection des enfants. Le constat du rapport est sans appel, il faut agir sans tarder avec volontarisme et efficacité notamment élargir les prérogatives de l'Arcom pour sanctionner les sites qui ne respectent pas, ben tout simplement la loi, soit l'interdiction d'accès aux mineurs et d'autre part généraliser. La plateforme Pharos aux violences sexuelles. Pour cela il faut émettre des moyens humains conséquents. La lutte contre la marché marchandisation du corps des femmes doit être une priorité absolue de politique publique. Alors que les violences exercées par les hommes sur les femmes ne baisse pas dans notre pays, on peut légitimement se questionner, voire même s'inquiéter du rôle que joue la consommation massive de pornographie merci très sincèrement à la délégation aux droits des femmes de ce travail ô combien nécessaire et courageux sur ce que vous avez très justement appelé l'enfer du décor. Le groupe socialiste, écologiste et républicain votera cette proposition de résolution.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues. Aujourd'hui, nous examinons une résolution importante qui appelle à faire de la lutte contre les violences pornographique une priorité de politique publique. Un principe de réalité s'impose à nous, mes chers collègues, nous vivons dans une société où la pornographie est omniprésente et où les violences sexuelles. Ils sont malheureusement aussi très présente. Car oui la pornographie contribue à la culture du viol et à la normalisation de la violence sexuelle. Les images violentes et dégradantes qui sont représentés, on donne impact réel sur la façon dont les hommes et les femmes se perçoivent eux-mêmes c'est pourquoi nous devons nous opposer fermement à une industrie opaque et mondialisée qui exploite et objective, le corps des femmes et des minorités de genre, nous devons comprendre que le porno est un produit culturel qui se nourrit des discriminations de genre dans notre société, pour générer des milliards d'euros de profits en effet l'excellent rapport de nos collègues mettent en relief dans que dans la pornographie, les femmes et les minorités de genre ils sont souvent relégués à des rôles stéréotypés et dégradants tandis que le mythe de la performance masculine. Il est sur-représenté. Il est grand temps de dénoncer cette représentation des sexes biaisé qui renforce les inégalités existantes et nourrit la culture de la violence sexuelle. En outre, nous ne manquerons pas de pointer du doigt une industrie sans aucun scrupule, dans laquelle les actrices pornographiques sont victimes d'exploitation de harcèlement et de violences sexuelles de plus. Par cette résolution nous souhaitons dénoncer une industrie du porno qui a des répercussions néfastes sur la santé physique et mentale des acteurs et des spectateurs. D'une part les actrices pornographiques sont exposés à des infections sexuellement transmissibles à des troubles de stress post-traumatique à des troupes de l'alimentation et à d'autres problèmes de santé mentale. les spectateurs de porno peuvent développer des addictions, des troubles de la sexualité et des problèmes de santé mentale. Mes chers collègues. Il est impératif que nous prenions des mesures pour contrer les effets nocifs de la pornographie actuelle sur notre société, en particulier, comme l'a évoqué, ma collègue Laurence Cohen nous devons fournir des ressources pour éduquer le public sur les dangers de la pornographie et sur les moyens de résister à ses effets néfastes. Cela peut inclure des des campagnes de sensibilisation ou encore des programmes éducatifs pour promouvoir une éducation sexuelle qui met en avant la diversité des identités de genre et des orientations sexuelles qui respecte la dignité et l'autonomie de chacune et qui lutte contre les stéréotypes sexistes et homophobes.

De plus, nous plaidons en faveur de mesures pour lutter contre l'exploitation des actrices dans l'industrie pornographique. Il est grand temps de travailler à créer des espaces sur égalitaire afin de protéger leur dignité et leur intégrité physique et mentale. Les violences systémique qu'elles subissent doivent cesser en nous devons renforcer les lois et les politiques qui protège les victimes de la violence sexuelle et de l'exploitation dans l'industrie pornographique. En France, la justice commence à ouvrir les yeux avec l'affaire French banking. C'était la première fois en France que des acteurs sont poursuivis pour viol dans des investigations visant l'industrie pornographique et nous n'y voyons nous vers la reconnaissance du fait que les actrices pornographiques ne sont pas des citoyennes de seconde zone leur plainte à la police doivent être prises au sérieux une meilleure formation des policiers et nécessaire au recueil de telles dénonciations en outre le droit à l'oubli ne doit pas être à 2 vitesses, pour les actrices du porno. Faut-il donc rappeler que certaines ont dû débourser entre 3 et 5000 euros pour faire retirer des vider l'eau des vidéos en ligne dans lesquelles elles apparaissait en faisant valoir leur droit à l'oubli. Cela n'est pas acceptable. Nous ne pouvons demeurer les bras quoi croisés et à ce propos Madame la Ministre j'ai envie de vous demander. Que comptez-vous faire des recommandations de ce rapport qui méritent à l'évidence que nous agissions, mes chers collègues, la violence sexuelle dans la pornographie est un problème de société qui nécessitent des réponses collectives en adoptant cette résolution. Nous nous engageons en faveur de la lutte contre les violences pornographique. Nous attendons qu'elle soit érigé en priorité de politique publique afin de mieux éduquer face à ces dangers et protéger les actrices pornographiques très souvent victimes de violences sexuelles. C'est une responsabilité que nous devons tous partager et un engagement que nous devons prendre. C'est pourquoi le groupe CRCE dans l'ensemble des membres et signataire votera bien évidemment cette proposition de résolution. Merci cher collègue. La parole est maintenant à monsieur Loïc Hervé, pour le groupe Union centriste pour 4 minutes. Monsieur le Président Madame la Ministre, mes chers collègues. Avant toute chose et comme tous les collègues qui se succèdent à cette tribune cet après-midi je tiens à saluer le travail exceptionnel qui a été effectué par notre délégation aux droits des femmes, en particulier par nos collègues la présente Annick Billon. Et nos collègues Alexandra Borchio-Fontimp Laurence Cohen et Laurence Rossignol, auteur du rapport d'information porno l'enfer du décor dont Ayman la présente proposition de résolution. Il s'agit d'un travail véritablement Pionnier, aussi incroyable que cela soit alors que la pornographie est à l'évidence devenue un problème social majeur. Le Parlement ne l'avait jamais véritablement investi. Avec ce rapport d'formation et cette proposition de résolution, la représentation nationale ouvre enfin les yeux. Il était temps, contre les préjugés, les plus communément répandue, c'est évidemment tout à l'honneur de notre haute assemblée d'avoir porté cette prise de conscience. Je tiens donc à affirmer sans ambiguïté que je soutiens sans réserve chacun des considérants de cette proposition de résolution dont je suis moi-même qu'on se cosignataires. La question qui est devant nous est importante. Madame la ministre, après la publication du rapport l'adoption ou je l'imagine tout à l'heure de cette résolution. Tout cela nous entraînera Madame la Ministre sans doute vers un texte de loi. Et posera nécessairement la question de l'adoption de mesures pragmatiques pour être efficace. L'interdiction pure et simple de la pornographie est un chemin que certains de nos collègues nous proposerons peut être d'emprunter. 100 préempter sur ce débat. Je crois pouvoir affirmer que la prohibition pourrait générer immédiatement la bascule de la pornographie dans la contrebande et la mafia. Qu'ils ont des mots encore pire que ce que nous connaissons déjà aujourd'hui et qui ont été longuement évoqués. Existe-t-il une pornographie éthique. Existe-t-il une pornographie moral est-ce notre rôle. D'y répondre dans les débats à venir. Je serai de ceux qui défendront un encadrement strict. C'est un chemin de crête qui demande de la conviction, mais qui à mes yeux et le seul qui soit en mesure de produire de réels effets sur la réalité vécue dans notre pays. Or pour encadrer la pornographie. Nous avons tout à faire. Et c'est bien ce travail que nous invite à mes yeux, encore une fois. Cette présente résolution. La seule pornographie qui puisse exister, se doit de respecter la loi mais avant tout la personne humaine et bien évidemment les femmes. C'est une pornographie Tulle de Côte d'adultes consentants et qui ne s'adresse qu'à eux. Aucune tolérance pour les viols. Ce sont des crimes aucune tolérance pour les abus de faiblesse ni la prostitution et encore moins le proxénétisme. C'est d'ailleurs ce que considère la Cour de cassation qui dans sa décision du 18 mai 2022. A. Refusé d'étendre la définition jurisprudentielle de la notion de prostitution à l'activité dite de Camille constituera proposé moyennant rémunération une diffusion d'images ou de vidéos à contenu sexuel. Pour séparer le bon grain de l'ivraie. Un cadre transversale doit être créée de toutes pièces car schématiquement on peut classer les problèmes causés par la pornographie en 2 grandes familles. Ceux liés aux personnes qui la font et ceux liés aux personnes qui ont accès. La protection des premières c'est-à-dire principalement des actrices. Pose la question des conditions de travail, ça a été évoqué par plusieurs collègues et des, des conditions de tournage dans la production de tous ces contenus pornographiques. C'est la seule solution pour prévenir les crimes tels que ceux qui ont récemment défrayé la chronique et qui sont d'ailleurs devant des juridictions de notre pays, ce sont même ces crimes qui sont à l'origine de notre prise de conscience collective. Quant à la l'énorme problème de l'accès de nos enfants et de nos adolescents. Il soulève l'impérieuse nécessité des plats que les plateformes soit. Contrainte à vérifier l'âge. La CNIL a fait des propositions et il y a un monsieur le président. Je suis un peu long mais il y a eu un élément qui est très important et j'en j'en terminerai par là et qui a à nos yeux doit être un élément de réflexion, c'est la régulation également des messageries instantanées qui sont un Champ extrêmement important. Vous l'aurez compris dans mes propos. Le groupe de l'Union centriste votera cette proposition de résolution sans aucune réserve. Merci cher collègue. La parole est maintenant Madame Esther Benbassa pour les non inscrits pour 3 minutes. Monsieur le président, mesdames les rapporteurs, madame la Ministre, mes chers collègues. Le ministre en charge du numérique, Jean-Noël Barrot, déclarait récemment, je le cite, en 2023 c'est la fin de l'accès aux sites pornographiques pour nos enfants. À seulement 12 ans près d'un enfant sur 3 a été exposés à du contenu pornographique en ligne. L'interdiction d'accès aux sites pornos mineurs manque sa cible quand il est juste demander à l'internaute de répondent en cliquant oui à la question de confiance sur sa majorité. Conscient de cette faille. Le gouvernement prévoit une phase test à compter. À partir de ce mois pour bloquer toute consultation de sites pornos aux mineurs. De fait, la jeunesse est trop souvent confrontés ici à une représentation déformée et inégalitaire des rapports hommes-femmes ces contenus accessibles facilement toujours plus violents font la promotion de l'acte sexuel forcé. Or, selon une étude de la BBC. Plus d'un tiers des femmes subissent des violences lors de l'acte sexuel ces pratiques ne sont-elles pas encourageait par la consommation d'un certain type de pornographie. Il est urgent d'agir. Mais comment. La corrélation de violences sexuelles et pornographie s'observe déjà au niveau des conditions de travail imposé aux actrices, lequel relève pourtant du code du travail, censé les protéger notre législation a clairement échoué jusqu'ici à dissiper les flou juridique entourant les métiers de la pornographie. Comment protéger les actrices sans les empêcher d'exercer leur métier. Il ne s'agit pas d'aggraver leur précarité en espérant abolir le porno, mais de se doter d'un arsenal législatif capable à la fois de garantir efficacement le consentement et la dignité des actrices et de sanctionner efficacement les producteurs encourageant les actes de violence lors des tournages. La pornographie relève du débat public. Cette résolution pourrait servir de point de départ à l'écriture d'un projet de loi. Sans oublier que le problème posé n'est pas un problème français mais international et que l'Europe devrait collectivement s'en saisir et sans oublier non plus qu'encadrer et punir ne suffit pas et que la clé est aussi comme le suggère AMIA Srinivasan professeur à Oxford, une éducation rappelant le jaune que le sexe peut restait ce que les anciennes générations en ont fait, mais qu'il peut aussi si eux-mêmes le choisissent, je cite, devenir quelque chose de plus joyeux de plus égalitaire de plus libre. Merci. Merci. Si cher collègue, la parole est maintenant Madame Valérie Boyer pour le groupe Les Républicains pour cinq minutes. Monsieur le Président Madame la Ministre, mes chers collègues. Pendant plus de 6 mois. La délégation du droit des femmes à mener des travaux sur l'industrie de la pornographie et ses travaux ont abouti à un rapport porno l'enfer du décor. Je veux remercier la présidente de la délégation du droit des femmes. Annick Billon d'avoir permis ce travail de fond aux côtés de nos rapporteurs Alexandria. Borchio-Fontimp. Laurence Cohen, Laurence Rossignol pour le formidable travail qui a été fait. Je voudrais vous féliciter parce que votre travail fait avancer à la fois les mentalités mais je l'espère aussi notre droit. Plus de 250 sénateurs dont 7 présidents de groupe on souhaite être associés à cette résolution. Le Sénat a pleinement conscience de d'urgence et de l'important de ce sujet et même si des mesures iront dans le sens de la protection des mineurs face à l'Exposition de la pornographie ne passons pas à côté d'un autre enjeu dont je voudrais vous parler, tout en soulignant quand même que cette industrie porno galère graphique réalise un hold-up sur l'intimité et le développement de nos plus jeunes en 2018, j'avais auditionné à l'Assemblée nationale, le journaliste Robin d'Angelo qui venait de publier le livre du jeudi. Lola Sofia et moi pendant un an il s'était infiltré dans le milieu du porno soi-disant amateur incarné en France par la puissante entreprise Jacky et Michel aussi. Alors que nous sommes interrogés à juste titre pendant des années sur l'Exposition et l'accès des jeunes à la pornographie nous avions occulter tout un pan de ce sujet si grave, il avait expliqué ce que personne n'osait dire à l'époque l'absence récurrente de consentement. Le non respect du droit du travail et des pratiques contraires à la dignité humaine dignité humaine. N'ayons pas peur des mots, il parle d'une forme de normalisation de la violence assez marquante est assez forte, je le cite, qui conduit forcément à des abus. Ce sont des abus. Ce ne sont pas des films, ce sont des scènes de violence et dès 2020, ses actes éclatèrent au grand jour avec l'ouverture d'une information judiciaire pour traite d'êtres humains. Viol aggravé en réunion ou proxénétisme aggravé contre la plateforme de vidéos pornographiques fraîche Bichkek. De graves atteintes au consentement pour des scènes dégradantes et très violentes sont mentionnés par les plaignantes et le réquisitoire du parquet feraient état de viols répétés de mensonges, d'intimidation et de l'utilisation de drogues quelques fois à leur insu de tests VIH falsifiés et de rackets pour retirer les vidéos pédo-porn pornographique pardon qui empoisonne leur vie. De même, l'ouverture d'une 2ème information judiciaire dans le cadre d'une procédure distincte à l'compte notamment des sociétés Jacquie et Michel, un des sites pornographiques français les plus consultés pour complicité de viol et traite d'être s'humains en bonne organisée a été réalisé ces procédures témoigne de la volonté des enquêteurs et la justice de porter une plus grande attention aux violences sexistes et sexuelles commises dans le milieu dit du porno français sans compter toutes les victimes qui n'ont jamais osé parler c'est près de 220.000 vidéos vues chaque minute sur la principale plateforme où se cachent parfois des réseaux criminels proxénètes et de traite d'être s'humains à grande échelle. C'est une industrie prospère. Une recherche sur huit sur un ordi concernent une vidéo porno ayant le courage de dire que les méthodes de l'industrie pornographique sont trop souvent identiques à celles des réseaux de traite d'être humains. C'est de la traite d'être s'humains d'ailleurs. Rabattage mise en confiance soumission par le viol exploitation mise sous terreur inversion de la culpabilité et chantage. Les tournages des actes. Sexuel sous contrainte économique et moral des agressions sexuelles et des viols, voire des actes de torture et de barbarie doivent être lourdement condamné. C'est pourquoi, mes chers collègues, nous ne pouvons pas voter dans cet hémicycle des lois pour protéger les victimes de violences sexuelles et fermer les yeux ou même toléré ce qui se passe bien trop souvent dans ces entreprises du porno et c'est pourquoi je crois que le Sénat peut être fier de proposer notamment de faire des violences sexuelles commises en 2. Contexte de pornographie un délit d'incitation à une infraction pénale de favoriser l'émergence de plaintes des victimes de violences commises dans un contexte de pornographie en améliorant leurs conditions d'accueil en formant des forces de l'ordre au recueil des plaintes de ses victimes spécifiques en instaurant le suivi de leur dossier par un contact unique de traduire dans les effectifs et les moyens matériels des services d'enquête et des magistrats, la priorité donnée à la lutte contre les violences collègues dans un contexte de pornographie ou en s'attaquant directement aux plateformes de diffusion car ces femmes et parfois ces hommes nous ne vont pas les oublier doivent à la fois se reconstruire mais supporter la diffusion non contrôlée de leurs vidéos dont elles sont victimes. Alors, mes chers collègues, je sais qu'aujourd'hui il est de notre responsabilité de porter le message de ses victimes et de ses victimes, qui sont aussi bien les personnes qui les regardent que celles qui sont exposées dans ses films ces disant acteur qui subissent ces violences voter cette résolution sites liés dire à toutes ces victimes. Nous sommes avec avec vous. Soyons fier. En votant ses propositions pour protéger. Ces hommes et ces femmes exploitées nous les défendons la liberté mais surtout la fraternité parce que la solidarité que nous leur devons est très importante et je crois que aujourd'hui les votants ce texte et cette. Sicilienne protégeant la dignité humaine vous remercie, merci pour votre travail. La parole est à monsieur Serge Riou pour le groupe socialiste, écologiste et républicain pour 4 minutes. Madame la présidente, madame la Ministre, Mesdames, Mesdames, et messieurs, chers collègues. Dans l'enfer des films porno. Le nom n'existe pas. Le oui est la norme. Malheureusement la réalité des dépasse parfois la fiction qu'ce rapport au consentement ou plutôt au non-consentement s'invite sur les tournages et s'immisce dans le cerveau des consommateurs. Le porno c'est avant tout la mise en avant d'une vision très singulière misogyne de la sexualité. Une une sexualité majoritairement filmées par des hommes pour des hommes le porno c'est une vision violente, brutale, dans laquelle les femmes sont souvent réduites à l'état d'objet dont on peut disposer, sans limite. Les insultes, les propos dégradants se substitue aux sentiments les coups aux caresse. L'écrit à la passion des gros pains les gros plan à la tendresse, la réalité est bien différente. Pourtant c'est à cette conception toute particulière de la sexualité, à laquelle nos enfants sont exposés. On a déjà dit, mais en effet 2 tiers des enfants de moins de 15 ans et un tiers des enfants de moins de 12 ans ont déjà eu accès à des contenus pornographiques. C'est le triste constat que tirent les autrice de 7 PPR. Smartphones Tablettes ordinateurs avec le numérique, chaque enfant, chaque adolescent détenteur d'un de ses appareils peut se rendre sur des sites pornos. Et être exposés à de la pornographie ah plupart du temps l'accès n'est conditionné qu'à un clic sur un bouton. J'ai plus de 18 hein. Un rap un rempart un carton facilement franchissable par quiconque sachant se servir d'une souris. Ce clique des pourtant pas sans conséquence pour un cerveau en plein développement. Pour un jeune en pleine construction. L'Exposition à la pornographie et pour certains une première approche de la sexualité. Une découverte qui parfois débute par le visionnage d'un vol à réunion d'un viol en réunion d'une vidéo hardcore. En effet, des contenus violents des gradins 100 souvent mise en avant sur les sites. L'impact sur les enfants dans la représentation qu'ils se font des femmes et des hommes de la sexualité des différentes orientations sexuelles est indéniable et destructeur traumatisme trouble du sommeil de l'alimentation vision déformée et violente de la sexualité. Des effets sont graves. Cette vision rétrograde violente est basée sur les rapports de domination entre les individus. Cette vision instaurée par le porno véhicule également des clichés des préjugés racistes Lesbos forme. Homophobes et transphobes qui nous revient de combattre. Lutter contre cette Exposition à des mineurs des mineurs à la pornographie n'est pas chose simple beaucoup des parents pensent contrôler les pratiques web de leur enfant. Malheureusement la pornographie est partout. Twitter, Facebook, Snapchat telegram redites qu'il s'agisse de continue Publié directement sur ces plateformes ou de Liens. Par message privé nos jeunes sont exposés de toute part, mes chers collègues. Il nous faut protéger nos enfants. Et en ce sens. Je remercie les autrice de ce PPR qui font des propositions pertinentes mieux contrôler l'accès aux plateformes est impératif et doivent respecter la loi. L'exposition de mineurs à des contenus pornographiques est un délit durcissant les conditions de vérification de l'âge, enfin il est essentiel d'accélérer des initiatives de prévention et de sensibilisation à destination des parents et des enfants, ces derniers doivent avoir davantage d'informations relatives à la sexualité à leur disposition pour que leur seul modèle ne soit pas la pornographie. En ce sens l'école et l'État doivent jouer un rôle. Mes chers collègues, cette position de 33 disposant de bon sens et bien sûr le groupe socialiste, écologiste et républicain de la votera. La parole est à Madame, Catherine Morin-, Desailly pour le groupe Union centriste pour 4 minutes. Madame la présidente Madame la Ministre, mes chers collègues. Avec cette proposition de résolution contre les violences pornographique. Que nous examinons aujourd'hui c'est effectivement une priorité publique avec le développement d'Internet les contenus pornographiques sont devenus quasiment libre d'accès via un ordinateur ou un téléphone. Or, comme le démontre le remarquable travail de nos collègues de la délégation aux droits des femmes. Ces contenus diffusent des images souvent dégradante reposant sur des maltraitances des viols ou du proxénétisme, y compris de mineurs et on assiste à une banalisation de la diffusion de ce type de contenus, pour le plus grand bénéfice d'une industrie qui elle prospère. C'est pourquoi, comme l'a dit notre collègue Loïc Hervé Le groupe de l'Union centriste votera cette proposition de résolution visant à susciter une prise de conscience dans notre pays. Pour améliorer le soutien aux victimes. Renforcer la réponse pénale contre ces violences. Empêcher la diffusion de ces contenus illicites et protéger notre jeunesse côté réponse pénale. Nous disposons déjà d'un outil exemplaire et unique en Europe la plateforme Pharos regroupant, policiers et gendarmes. Cette plateforme effectue une veille d'Internet et disposent des moyens juridiques et techniques pour retirer les contenus illicites ou en bloquer l'accès sur la base de signalements tout ceci sous le contrôle d'une personnalité qualifiée Laurence pécho Rivolier membre de l'art comme j'ai pu échanger avec eux leurs témoignages sont attirants. À la limite du supportable lorsqu'il s'agit d'enfants ou même de nourrissons. Leur travail est exemplaire. La création d'une catégorie violences sexuelles serait effectivement bienvenue mais les moyens de Pharos doit être aligné sur cette ambition en particulier la personnalité qualifiée dont le travail est très éprouvant et qui mériteraient d'être remplacée par une structure collégiale maintenant la régulation sur Internet dépend aussi et principalement de la législation européenne le 18 ou vous le savez ces actes récemment voté prévoit que les autorités des États membres peuvent demander aux fournisseurs d'agir contre les contenus illicites. Je regrette toutefois et je l'ai maintes fois dit que la responsabilité des fournisseurs de services d'hébergement dont on connaît le modèle économique particulièrement toxique demeure limité dans la diffusion de ce type de contenu. N'oublions pas qu'ici même, Francis. La lanceurs d'alerte nous avertissait que Facebook privilégiera toujours le profit à la sécurité des enfants ainsi dans la proposition de résolution européenne sur la lutte contre les abus sexuels sur les enfants en ligne qui a été adopté par notre commission des affaires européennes. Le 15 février dernier avec mes collègues Ludovic et et André rachat nous avons redit cela et nous avons proposé aussi que la Commission européenne puisse indiquer au public quel fournisseur ne respectent pas leurs obligations. Tout cela dans une logique de. Afin que le risque réputationnel les incite à respecter scrupuleusement la réglementation ensuite merci aux auteurs de la proposition pour leurs mesures visant à mieux protéger notre jeunesse notamment la mise en place de dispositifs de contrôle parental a activé par défaut sur les appareils où l'écran noir qui serait imposée aussi ne vérifie pas l'âge de leurs utilisateurs. Ces recommandations conforte celle que nous avons fait avec mes co-rapporteur pour mieux lutter contre la pédopornographie. Cette nuit-là nécessite des efforts plus que redoubler au niveau national comme au niveau européen car elle constitue une délinquance de masse multiforme qui prolifèrent. Ainsi en 2021, l'agence policière européenne Europol que j'ai pu visiter il y a une quinzaine de jours démanteler le réseau Boys Town, qui comptait 400.000 utilisateurs sur le dark web on peut aussi rappeler l'enquête ouverte contre TikTok l'an dernier pour son nom signalements de contenus pédo-pornographiques. L'Union européenne détient hélas un triste record. Mes chers collègues, celui du 1er hébergeur de contenus à caractère pédo-pornographique dans le monde et en France, selon Madame Picoury voliez sur 150.000 contenu litigieux examinés par elle. En 2021, environ 70% étaient des contenus à caractère pédo-pornographique

Madame la présidente, madame la ministre, madame la présidente de la délégation droits des femmes. Mes chers collègues corapporteur que je félicite pour leur excellent travail, mes chers collègues, en quelques clics sur leur téléphone. Les petits Marceau. Noé peuvent aujourd'hui très facilement visionner des contenus pornographiques disponible gratuitement en ligne, même lorsqu'ils mettent en scène des pratiques violentes douloureuse, humiliante, voire des viols. Est-ce acceptable. Les conséquences sur nos enfants sur leur développement affectif, psychologique et sexuel sont alarmantes. Nous l'avons vu donc nos mineurs peuvent accéder à des contenus gratuits mais pas à des sites pornographiques, payants. N'est-ce pas curieux. En 2020, le Sénat était saisi d'une PPL visant à protéger les victimes de violences conjugales, présenté par des députés de la majorité, rapporteur de ce texte qui inclut l'accès des mineurs aux sites pornographiques. J'ai donc procéder à des auditions complémentaires afin de pouvoir proposer au Sénat un dispositif à la hauteur des enjeux m'inspirant une mesure en vigueur depuis 10 ans pour les jeux en ligne. J'ai proposé un amendement visant à instituer une nouvelle Prost il dure destiné à obliger les éditeurs des sites pornographiques à mettre en place un contrôle de l'âge de leur clients ni chers collègues, vous avez voté mon amendement à l'unanimité le 10 juin 2020. Je vous en remercie. Il donne des prérogatives à l'comme que je ne vais pas détailler. Quel bilan depuis le vote de cette loi visant à protéger les victimes de violences conjugales du 31 juillet 2020. Pourquoi faut-il déployer tant d'énergie pour être entendu alors qu'il s'agit bien là d'une priorité publique d'une loi votée de la protection de l'enfance, rappel des faits. Le décret d'application de mon amendement n'a été pris en compte que le 7 octobre 2021 soit 14 mois plus tard pourquoi 5 sites pornographiques parmi les plus regardées sont alors sommé de se plier à cette loi ni mise en demeure sont restées sans effet. Malgré des constats d'huissier. Plus de 500. Le président du tribunal judiciaire de Paris est saisie en septembre 2022, la justice française examine la demande de blocage de ces sites et en juin finalement l'Arcom de rencontrer un médiateur. Vous avez bien entendu un médiateur, c'est du jamais vu. De leur côté les sites dépose une QPC, la Cour de cassation refuse heureusement leur argument, le 5 janvier 2023. C'est une petite victoire pour nos enfants l'Arcom confronté à des sites pornographiques, usant de manoeuvres dilatoires pour éviter un blocage par la justice a récemment mis fin à ce processus de médiation inutile incompréhensible et choquant. Le ministre Barrot a annoncé testé fin mars à système de vérification d'agent double anonymat qui ne laisse perplexe testé mais jusqu'à quand. Cette solution devrait avoir fait ses preuves avant de pouvoir être étendue quand sera-t-elle mise en place définitivement en attendant que va faire la justice reporter ces décisions et pendant combien de temps. Et pendant ce temps là nous petit Jules Gabin Daphné peuvent continuer de voir de la pornographie gratuite. Enfin et pour moi c'est le plus important ce système déresponsabilise les sites pornographiques gratuits mon amendement leur impose pourtant de vérifier l'âge de leurs visiteurs. Comme d'autres sites savent le faire les outils législatifs sont en place, il faut seulement se préoccuper de faire appliquer la loi avec une vraie volonté politique et des moyens. Après une intervention, mes chers collègues. Les pompiers employes une très jolie formule, ils évaluent le sauver. Depuis l'adoption de cette loi. Peut-on évaluer le nombre d'enfants protégés de ces contenus qui ne sont pas faits pour eux. Quel est le sauver. C'est facile à évaluer. Je vais vous le dire, la loi n'est pas appliquée. Madame la Ministre le sauver c'est zéro. Je vous laisse juge. Merci beaucoup. La parole est à madame Isabelle Rome, ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes de la diversité et de l'égalité des chances. Madame la présidente. Madame la présidente de la délégation aux droits des femmes cher Annick mesdames les sénatrices messieurs les sénateurs. En préambule, je tiens à souligner mesdames les sénatrices Bion. Borchio-Fontimp Cohen et Rossignol. La qualité du rapport que vous avez produit en octobre dernier. Vos travaux jette la lumière sur des faits de société trop souvent passé sous silence mais qui portent en eux une violence inouïe, à l'égard des femmes. Vos travaux contribuent à faire évoluer les mentalités et permettent au Parlement pour la première fois de mettre ce sujet à l'ordre du jour. Je sais aussi que vous avez fait preuve d'une grande force en recevant les victimes et en écoutant l'effroyable récit des sévices qu'elles ont subi. Aujourd'hui parmi les termes les plus recherchés sur les plateformes pornographique on trouve sexe brutal ados amateurs Mohamed sonne ou encore ado vierge. Ces termes ne sont pas des fantasmes. Ils sont des appels à la violence au crime. Il peut s'agir osant nommer les choses de viol avec torture et actes de barbarie punissable de la réclusion criminelle à perpétuité. Je tiens donc à remercier les sénatrices qui ont conduit ce travail d'avoir fait la lumière sur ce tabou. Chaque seconde que sont tu les violences pour nos graphique est une seconde de souffrance pour des milliers de victimes. Des milliers de femmes abusées. À force de pressions financières et psychologiques, ces femmes se sont par exemple toutes celles qui sont condamnés à vivre avec un cauchemar qui se répète chaque fois qu'un une qu'un utilisateur appuie sur play et qui attendent le jugement de leur agresseur. C'est aussi pour elle que nous devons agir. C'est en pensant à chacune d'elle que je parle devant vous aujourd'hui, elles sont les victimes de la violence de l'industrie pornographique, j'utilise le thème industrie à dessein car ces violences répondre à la demande des consommateurs. Pour y mettre fin. Sur le long terme la réponse pénale ne suffit pas. Nous devons protéger et sensibiliser les plus jeunes aux dérives de la pornographie. Vous l'avez rappelé, sur les 19 millions de personnes qui en France visite chaque jour un site pornographique. Il y a un million d'adolescents qui ont entre 15 et 18 ans et 1,2 millions d'enfants âgés de moins de 15 ans. La violence des sites pornographiques et souvent pour eux le premier aperçu de ce qu'est la sexualité et cela se traduit chez nombre de jeunes par une vision déformée et violente des rapports sexuels qui peut aussi entraîner des difficultés à construire et entretenir des relations affectives. En tant que magistrate je peux l'affirmer. Il y a là un terreau très favorable à des comportements violents envers les femmes. Une des clés réside dans l'éducation. L'école de la République doit être un lieu de savoir d'émancipation et d'éducation à la citoyenneté depuis 2001. La loi prévoit que l'éducation à la sexualité doit être dispensés dans les écoles, les collèges et les lycées, à raison de 3 séances annuelles. Des séances d'éducation à la sexualité fondée sur un apprentissage du respect de l'autre sur Novak valeur cardinale du respect de soi et de l'autre, d'égalité et sur l'apprentissage du consentement. Dès notre arrivée au gouvernement avec mon collègue Pap Ndiaye. Nous avons fait de l'application de cette loi, l'une de nos priorités. Nous devons porter un message pédagogique fort à destination de notre jeunesse. Nous avons pris le problème à bras le corps. Le ministre de l'Éducation nationale a publié le rapport produit en juillet 2021 par l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Il a publié également sur son site un vade-mecum de l'éducation à la sexualité afin d'en exposer le contenu et les gens je et. Depuis février. depuis quelques semaines, un groupe de travail interministériel a été mis en place pour élaborer ou. Renouveler actualiser les contenus. J'ai les ressources pédagogiques et renforcer les formations des personnels pédagogiques. L'autre message éducatif doit être assez puissant pour mettre à mal l'idéologie patriarcale et méprisante pour les femmes que diffuse trop souvent les plateformes quelle qu'elle soit. Car il serait erroné de penser que l'on ne peut trouver la violence pornographique que sur les sites dédiés le rapport l'illustrent parfaitement les plateformes telles que Twitter Meta Tik Tok ou Snapchat héberge aussi ces contenus d'une grande violence. Par cette proposition de résolution nous devons exprimer une position claire sur un sujet que la société doit enfin regarder en face. À mon initiative des discussions interministérielles sont actuellement en cours pour prendre des mesures fortes à l'encontre des diffuseurs qui ne pourront plus se cacher derrière un prétendu pseudo vide juridique. Votre travail mesdames les sénatrices a porté ses fruits. D'abord avec cette proposition de résolution que vous examinez aujourd'hui et puis ensuite par le travail qui est en cours pour imposer aux plateformes qu'un travail qu'un pardon qu'un contrôle efficace de l'âge de l'internaute soit enfin mise en place et ce. Grâce à l'engagement de mes collègues. Éric Dupond-Moretti Jean-Noël Barrot et Charlotte Caubel. Le décret. Prévoyant le contrôle parental sur tous les terminaux sera promulguée prochainement. Je tiens par ailleurs à rappeler la campagne gouvernementale ambitieuse lancée à l'occasion du Internet Safer. Grâce au site je protège mon enfant Point gouv Point FR nous offrons enfin aux parents les outils dont ils ont besoin pour préserver leurs enfants des contenus violents ce qu'est la pornographie. Nous voulons aller plus loin, un travail est en cours également sur les prérogatives de l'Arcom et je suis aussi particulièrement attaché à améliorer les possibilités de retrait des images intimes divulgué à l'insu des personnes. Et parce que c'est problématique dépasse nos frontières la collaboration internationale est essentielle pour réellement porter un coup d'arrêt assez de violence. J'étais en Suède hier pour échanger avec mon homologue sur les bonnes pratiques mises en place dans nos pays respectifs. Nous allons approfondir notre coopération sur le sujet. Mesdames les sénatrices en votant cette proposition de résolution vous soutiendrez la politique ambitieuse. Que mène votre gouvernement face à ce fléau et messieurs les sénateurs. Je j'ai dit Madame le sénatrice triste que c'était les, c'était les rédactrices de ce rapport. En votant cette proposition de résolution vous aiderez les victimes à ne plus se sentir seul face à cette industrie violente. Que ces femmes nous entende cet après-midi. Ensemble, nous devons faire face à cette responsabilité qui est la nôtre. Je vous remercie. Merci madame la ministre. Alors nous allons procéder au vote sur la proposition de résolution, la conférence des présidents, a décidé que les interventions des orateurs Vali explications de vote. Alors je mets aux voix, la proposition de résolution qui et pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Donc adopté. À l'unanimité. Je vais demander à chacun de rejoindre sa place, je ne vais pas suspendre la séance on va démarrer de suite. Alors

l'ordre du jour appelle les explications de vote et le vote sur la proposition de loi visant à renforcer la voix des élus locaux au sein du service public de l'assainissement francilien présenté par Madame. Marta de Cidrac et plusieurs de ses collègues. je vais donner de suite la parole à Madame Catherine Bell Rithy rapporteur de la commission des lois pour sept minutes, chers collègues.

Madame la présidente Madame la Ministre, mes chers collègues. La proposition de loi de Marta de Cidrac et de nos collègues entend répondre à un réel problème dans le fonctionnement du Syndicat interdépartemental pour la liste hennissement de l'agglomération parisienne. Le Siaap et ses relations avec les élus des communes disposant d'une station d'épuration sur leur territoire ou situé à proximité et exploité par ce syndicat. Cette lacune est apparu de manière particulièrement criante lors des différents incidents survenus au sein de l'usine Seine Aval et récemment encore lors de la fuite de 4 tonnes de biogaz en octobre 2022. Les élus des communes des Yvelines et du Val-d Oise pointe à juste titre un déficit sérieux de communication sur ces accidents leur ampleur leurs conséquences et leurs solutions pour y remédier, vous le savez en matière d'assainissement, la région parisienne et doté d'une organisation spécifique avec un syndicat dont les membres statutaires sont les départements de Paris et de la petite couronne. Actuellement seul le dispositif qui associe officiellement les élus locaux à la gouvernance du Siaap et la conférence d'information annuelle de l'assainissement de l'agglomération parisienne prévue par les statuts du sien. Or cet outil n'est pas suffisant pour répondre aux attentes légitimes en matière d'information des élus locaux. Puisqu'elle ne se réunit qu'annuellement et ne traite pas spécifiquement de la gestion des sites qui peuvent être sensibles comme les stations d'épuration. Cette situation doit donc évoluer rapidement, car nous savons bien, les élus locaux sont toujours en première ligne auprès de leurs concitoyens lorsque de graves incidents surviennent dans leur commune. Il est donc pas acceptable que ces derniers soient laissées sans information. Bien que par la voix de son président le Siaap et reconnu que des défauts d'information ont eu lieu par le passé. Et mais indiqué mener des actions pour y remédier. Celle-ci ne saurait suffire. C'est pourquoi l'intention qui anime la proposition de loi de Marta de Cidrac a emporté la complète adhésion de la commission. Qui a néanmoins souhaité améliorer le caractère opérationnel du dispositif du texte au bénéfice des élus locaux. En 1er lieu, la Commission a décidé de renforcer l'effectivité juridique de la proposition de loi en précisant son Champ d'application. En effet, les communes situées sur le territoire des départements de l'Essonne. De la Seine-et-Marne du Val-d Oise et des Yvelines ne bénéficient pas des prérogatives dont disposent les départements membre du CIAT Paris, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis. Puisque ces communes ou leurs intercommunalités de rattachement ne sont pas liées. Au CIAP que par des conventions et non à ce titre, pas d'accès aux organes de gouvernance du sien. En second lieu. La commission a choisi de préserver l'équilibre de la gouvernance du sien. Le Siaap rempli sa mission de manière satisfaisante pour nos concitoyens francilien. La proposition de loi prévoyait l'octroi d'une voix délibérative aux communes siégeant au sein du conseil d'administration et du bureau du sien. La commission a estimé qu'apporter des bouleversements conséquent dans sa gouvernance. Qui plus est, dans le contexte du déploiement du plan baignade en vue des Jeux olympiques de 2024, ne semblait pas opportun. La commission a préféré attribuer une simple voix consultative aux communes. Cette solution apportera une réponse immédiate et adéquates aux attentes exprimées par les élus locaux. Tout en maintenant les équilibres existants. En 3ème lieu. Le texte retenu par la commission renforce l'opérationnalité du dispositif en améliorant l'information de tous les conseillers municipaux des communes concernées via à 2 mécanismes distincts. D'une part en rendant tous les conseillers municipaux des communes représentées au conseil d'administration du CIAT destinataire de la convocation adressée. Avant chaque réunion des documents afférents et de la liste des délibérations qui ont été examinés.

faisant l'objet d'une délibération ayant une incidence directe ou indirecte sur la gestion des installations de traitement des eaux usées situées sur leur territoire. Pour conclure mon propos. Je tiens à souligner que j'ai travaillé en parfaite coopération avec notre collègue Marta de Cidrac. Je la remercie chaleureusement de la qualité de nos échanges et donc de notre collaboration pour formuler des pistes de solutions équilibrées et sans et consensuel pardon dans l'intérêt des élus locaux des communes de la grande couronne parisienne. Je vous remercie pour votre attention. Merci cher collègue. Là. Parole et maintenant madame Madame Dominique Faure au Ministre délégué chargé des collectivités territoriales et de la ruralité. Merci ruralité. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, madame. La sénatrice. Cidrac. Sûr, monsieur le président de la commission et madame. La rapporteure. Nous sommes aujourd'hui réunis pour étudier une proposition de loi de la sénatrice Marta de Cidrac visant à renforcer la voix des élus locaux au sein du service public de l'assainissement francilien le Siaap. Proposition de loi qui a été adopté en commission des lois après un avis de sagesse du gouvernement. Le Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne. Le Siaap, qui a été créé en 1970 est en effet chargé du transport et du traitement des eaux usées produites par l'agglomération parisienne, à savoir 287 communes rassemblant plus de 9 millions d'habitants. Le Siaap est un établissement public administratif ayant historiquement pour membres les départements de Paris, des Hauts-de-Seine de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Le conseil d'administration du sien est ainsi constitué de 33 représentant de ces quatres départements 12 représentants de Paris 7 représentants des Hauts-de-Seine, 7 de la Seine-Saint-Denis et cette du Val-de-Marne par ses missions le ciel travaille toutefois une échelle territoriale plus large et en particulier dans les départements de la grande couronne parisienne. C'est la volonté d'être associés au fonctionnement du Siaap qui vous a conduit mesdames et messieurs les sénateurs à présenter la présente, proposition de loi qui vise à prévoir la présence au conseil d'administration avec voix consultative de représentants des conseils municipaux des que des communes accueillant une installation géré par le sien. Ce souhait d'association large des collectivités au fonctionnement de cette structure de coopération interdépartementale me semble parfaitement légitime, notamment pour assurer la bonne information des élus quand surviennent comme cela a pu être le cas sur certains sites du Siaap des accidents d'exploitation. S'agissant du simple État s'est montré particulièrement attentifs au cours des dernières années a renforcé cette structure et les modalités d'associations, des élus du territoire assez décision à la suite d'une mission conduite par le préfet Gaudin pour le compte du préfet de la région Île-de-France. Une conférence de l'assainissement a ainsi été mis en place avec pour objectif d'assurer l'information et l'association des élus des territoires d'implantation du Siaap par ailleurs les commissions de suivi de site mises en place ont aussi des lieux d'information et d'échange qui associent largement les collectivités les élus accueillant des stations d'épuration gérée par le Siaap. La proposition de loi dans sa forme initiale comportait un certain nombre de fragilités juridiques qui ont été corrigés par un amendement de Madame la rapporteure prévoyant que seules les communes présentant la double condition d'être situé dans un département non membre du Siaap et d'avoir sur leur territoire, une station de traitement des eaux usées exploité par ce syndicat intègre le conseil d'administration avec une voix consultative cette évolution de l'écriture et de nature à limiter les fragilités juridiques de votre proposition. Même si le gouvernement estime qu'une révision des statuts du Siaap pourrait avoir le même effet, sans nécessiter de recours à un support législatif mais pour toutes ces raisons conforme à ma position lors de l'examen de ce texte en commission, je m'en remettrai à votre sagesse, je vous remercie. Merci madame la ministre. La parole est à madame Marta de Cidrac pour le groupe Les Républicains pour cinq minutes. Madame Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois. Madame la rapporteure les chers collègues. La proposition de loi que nous allons voter vise à renforcer la voix des élus locaux au sein du Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne, communément appelé le sien. Et qui exerce de manière dérogatoire au droit commun la compétence assainissement pour 4 départements de la petite couronne parisienne. Ces départements qui était à l'origine de la création du sien pour 1970 sont Paris Les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis et regroupe près de 9 millions d'habitants. Depuis sa création en 1970 son Champ d'action s'est étendu via des conventions à 187 communes des départements du reste d'France toutefois ces communes ne participe pas à la gouvernance du Siaap, pas plus que les départements dans lesquels elle se situe. Vous comprendrez chers collègues que cette situation incompréhensible est devenue un inacceptable pour les élus locaux concernés car elle ne leur permet pas d'exercer pleinement leur mandat d'élu local et d'être le relais pertinent auprès de auprès de leurs habitants et de les rassurer. Lorsque des incidents majeurs se produisent comme ce fut le cas à l'usine Seine Aval. Ces dernières années. Alors je tiens à remercier les cosignataires de ma proposition de loi présentée aujourd'hui au vote du Sénat car il permettra, j'en suis certaine Madame la Ministre de rassurer les élus de ces territoires et de faire évoluer les relations entre le Siaap et les territoires d'implantation. Je tiens également à remercier le président de la commission des lois et ma collègue Catherine Belghiti dont je salue le travail et l'écoute. La rédaction qui est proposée aujourd'hui permet de trouver une première réponse aux demandes des élus locaux des départements de la grande couronne parisienne qui ne sont pas ou ou trop peu informés des décisions du sien. De la même manière qu'ils sont trop peu, trop peu informés des événements importants qui concernent les installations situées sur leur territoire. Le texte qui est soumis à votre, à votre votre cher collègue renforcent leurs droits. L'information et leur assure une voix consultative au sein du conseil d'administration du sien. Ainsi, les élus locaux pourront participer aux réunions du syndicat et seront en mesure de faire valoir directement leurs difficultés tout en obtenant davantage d'informations sur le fonctionnement des installations situées sur le commune. Rien de plus normal. Toutefois, j'ai quand même un regret, on en a toujours. Je regrette que le sous-amendement proposé par notre collègue Jacqueline Eustache-Brinio n'ait pas été adoptée à l'occasion de l'examen du texte et cela malgré l'avis favorable de la rapporteure. Il aurait permis aux aux communes ne disposant pas d'une station d'épuration sur leur territoire de bénéficier des de et des nouveaux droits créée par la proposition de loi en se fondant sur un critère lié aux risques plutôt qu'à un critère géographique. Toutefois, comme je l'ai déjà dit et je le rappelle, le texte que nous allons voter permet d'ores et déjà, de trouver une première réponse aux demandes des élus locaux des départements de la grande couronne parisienne et en tant qu'auteur de ce texte la rédaction équilibrée ainsi trouver me satisfait pleinement car elle tient compte des observations des remarques et des réserves qui ont pu s'exprimer tout au long de nos débats. Pour toutes ces raisons, le groupe Les Républicains votera l'adoption de ce texte et je ne serai pas plus long et je remercie l'ensemble des collègues qui ont prêté attention à mes propos. Merci cher collègue. La parole est à monsieur Franck Menonville pour le groupe les indépendants pour cinq minutes. Madame la présidente, madame la ministre madame la rapporteure. Monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues. Depuis 1970, le Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne. Sia transporte et dépollue pour quelque 9 millions d'usagers. Les eaux usées, les eaux pluviales et industriel de l'agglomération francilienne. Nous le savons, les stations d'épuration sont des sites particulièrement sensibles. Les risques que que peuvent présenter les accidents pour la santé publique pour l'environnement et et les populations avoisinantes ne sont. Évidemment pas négligeable. Malheureusement, en juillet 2019 et ça a été. Rappelé un important incendie s'est déclaré au sein de la station d'épuration d'Achères du Siaap.

sur la surface du fleuve. Cet incident grave s'ajoute à une liste d'accidents survenus récemment n'ayant pas toujours d'ailleurs fait l'objet d'une communication en spontanée. Ainsi, en octobre dernier, les élus ont dû attendre plusieurs jours avant d'apprendre la fuite dans une usine des Yvelines, laissant échapper plus de plus de 4 tonnes de méthane dans l'atmosphère. Cette fuite a été qualifié d'incident majeur par la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'aménagement et des transports. Il est aujourd'hui donc nécessaire de rétablir la confiance, la confiance des élus mais aussi la confiance de nos concitoyens. Cette proposition de loi vise à apporter donc des réponses. Au manque de dialogue entre le syndicat et les élus en favorisant des échanges plus transparents et plus systématique. Actuellement les élus se réunissent seulement lors des conférences annuelles de l'assainissement et c'est insuffisant. Je salue donc l'initiative de notre collègue Marta de Cidrac qui était parfaitement nécessaire et légitime. Elle permettra de faciliter la transmission des informations et d'impliquer davantage les élus concernés en renforçant leur voix le travail donc menée par Madame la rapporteure Catherine Bell Arletty a permis de renforcer le contour juridique du texte et d'assurer la représentation équilibrée au sein du syndicat. Je pense notamment à l'octroi aux élus d'un simple d'une simple voix consultative cette mesure donc répond aux attentes qu'ils ont exprimé. Elle permet d'associer davantage les élus locaux tout en garantissant l'équilibre institutionnel. Donc cette solution. Va dans l'intérêt des communes concernées. Elle conserve ainsi l'esprit d'initia initial donc de la proposition de loi la rapporteure aussi permis de renforcer l'information des conseils municipaux bien via la communication en amont des documents nécessaires aux délibérations. Par ailleurs ce texte garantit donc le droit à l'information des conseils municipaux concernés par une délibération au sein du Siaap ayant une incidence directe ou indirecte sur leur territoire. Au nom du groupe les uns des correspondants donc j'accueille donc favorablement cette proposition de loi qui. Qui renforce et associe davantage et mieux les élus. C'est dans l'ADN du Sénat et c'est dans la veine de notre groupe. Merci. Merci, cher collègue, la parole est à Monsieur Daniel Breuiller pour le groupe. Ah. Écologiste solidarité et territoires excusez-moi chers collègues. Et madame la présidente. Madame la présidente. Madame la rapporteure de la commission des lois. Madame la ministre, chers collègues. Le texte qui est soumis au débat aujourd'hui vise à renforcer la voix des élus locaux au sein du syndicat public de l'assainissement francilien le Siaap cette demande fait notamment suite à plusieurs incidents survenus sur la station d'épuration dite Seine le dernier une fuite de 4 tonnes de biogaz qui vient d'être révoqué de l'usine d'épuration d'Achères est particulièrement grave et montre un dysfonctionnement avéré de la gestion de crise du Siaap la sécurité des stations est un sujet important et l'on ne peut que déplorer l'absence d'un circuit efficace d'information à l'égard des élus locaux tels que vous le formulez cher collègue madame de Cidrac Rome à remédier à ces difficultés en associant à la gouvernance du Siaap les élus à proximité des stations d'épuration. Bien que la réponse apportée soit discutable en termes de gouvernance des syndicats. La proposition nous semble légitime au regard de la situation réelle. Les propositions de la rapporteure Catherine Bell. Sur le critère lié aux risques plutôt que géographique et sur deux le maintien des équilibres de gouvernance nous paraissait nécessaire. Le groupe geste sera favorable est favorable à plus de représentativité des collectivités locales et notamment des communes directement impacté par les installations d'un d'assainissement. Il est normal que les élus en première ligne auprès des populations concernées par les dommages et les nuisances de ces stations est une voix délibérative toutefois s'en tenir au seul sujet de gouvernance sur cette question me laisserai dire comme Cyrano, c'est un peu court, on pouvait dire bien des choses en somme la gestion du risque et le coeur en fête du sujet plus que la gouvernance le Siaap a été sommé de faire des modifications dans ses process de sécurité et de formation du personnel, suite à l'incendie de 2019, mais qui porte réellement la responsabilité de tous les risques dus à la présence de la plus grande station d'épuration d'Europe qui traite les eaux usées de 9 millions d'habitants. Cette usine classée Seveso en seuil aux impôts, à la fois cela lui impose à la fois des normes drastiques de sécurité et des contrôles réguliers de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'Aménagement et des Transports, le sujet d'actualité, la semaine dernière une barge d'un des fournisseurs du Siaap qui naviguaient sur la Seine a heurté la pile d'un pont de Triel-sur-Seine des essence échapper 70 à 80 m3 de nitrate de calcium dans la Seine, la communication s'est améliorée, les élus ont été informés dans la presse locale, le maire s'est voulu rassurant, les habitants n'ont pas à s'inquiéter. Évidemment ce n'est pas bon pour les poissons évidemment et je le confirme, c'est même très mauvais pour l'ensemble de l'environnement et pour la biodiversité. En 2019, l'incendie de l'usine avait provoqué la mort de 3 tonnes de poissons un bras entiers de la scène montrer ce spectacle de désolation aspect le plus visible de la catastrophe et les odeur était pestilentielle. Depuis le fonctionnement de la station en mode dégradé là s'évacuer toujours dans la scène des eaux non traitées en cas de fortes pluies et je veux parler aussi de l'épandage des boues sur les Terres agricoles du parc naturel du Vexin qui permet de recycler les boues résiduaires de la station d'épuration d'Achères et qui sont impropres à la culture. Dans un compte rendu d'un comité de suivi du 8 mai 2021. Le sous-préfet indiquait que la France n'avait pas la culture du risque, en effet la conclusion des documents d'analyse de santé publique France révèle des concentrations de plomb allant de 138 à 176 milligrammes par kilogramme de terre alors que le seuil qui définit une pollution due à l'activité humaine est fixé à 53 milligrammes. La présence de plomb ne peut pas. Rend impossible d'exclure un effet sanitaire en lien avec cette présence de plomb dans les sols pour les enfants de 0 à 6 ans la France n'a donc pas la culture de la gestion du risque, mais elle a une culture du silence sur ces sujets. Alors qui est responsable. L'ARS à qui nous demandons de lancer un dépistage de saturnisme pour les enfants de moins de 7 ans dans les plaines des Yvelines et du Val-d Oise. L'État qui glane Madame la Ministre des informations dans tous les comités de suivi avec le Siaap mais sans réelle garantie de résultat à ce jour, ni d'exigence peut être suffisante. Le Siaap lui-même qui doit mieux assumer les conséquences directes et indirectes de ces activités très utiles aux populations mais conséquences parfois dramatiques sur le vivant et la biodiversité. Il doit mieux informés et donc intégrer les représentants des collectivités dans sa gouvernance aura nous l'espérons, cet effet de peut-être mieux protégés et d'anticiper des retombées dans les territoires concernés. Des élus impactés doivent avoir droit au chapitre pour toutes ces raisons, malgré des interrogations profondes le geste votera pour cette proposition de loi. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur le président, Alain Richard pour le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants pour cinq minutes. Merci madame la présidente. Madame la Ministre, mes chers collègues. Je voudrais ajouter un petit point d'histoire pour expliquer pourquoi ce syndicat a été créé en 1970 et ce point d'histoire est plutôt satisfaisant. Quand on regarde le passé profond parce que la Ville de Paris avait les ressources et avait le le savoir- faire pour développer un système de d'assainissement, je parle là des du début du XXe siècle et du fait que son statut jusqu'à la réforme de 75 ne lui permettait pas d'entrer dans un syndicat de communes. La ville de Paris d'une certaine tendance politique à l'époque et les petites communes de banlieue qui se développait en général d'une autre tendance politique ont eu la sagesse de se mettre d'accord en considérant que ce serait le département de la Seine qui serait le rookie commun pour le transport et l'assainissement des eaux et il faut préciser que ce projet date des années 1920, le 1er projet de l'usine d'Achères 22.929 et que j'ai pu être directement témoin de ce que l'agglomération centrale de Paris la a traité correctement ses eaux usées sans les rejeter dans la Seine qu'au cours des années 90. Jusqu'à présent nous étions. Franchement. Défectueux et je veux rendre hommage au travail qui a été fait sur cette longue durée par le Siaap et par ses ingénieurs en particulier. Mais bien sûr par les élus qui en avait la responsabilité car à travers. De sérieuses difficultés et de des financements tout à fait considérable. le CEA a développé une technologie. Qualité de gestion de ces installations de d'épuration qui je crois lui permettent de. Bien remplir sa mission et dans des conditions de sécurité. Mais comme l'a dit le collègue en effet ça ne fait pas. Ça n'empêche pas qu'il y ait des incidents ou des difficultés de voisinage. Alors il y a. Un point que je trouve convaincant dans la proposition de loi telle qu'elle sort de la commission. C'est la liste des. Prérogatives des droits reconnus ou représentants des communes directement intéressés, c'est-à-dire les documents qui doivent recevoir la participation qu'il peut avoir au débat. Ou aux travaux du syndicat. En revanche, il y a me semble-t-il de manque ou de défauts significatifs. Le premier alors qu'il s'agit d'un syndicat de collectivités territoriales c'est de donner le droit de participer. Dans une assemblée d'élus responsables. À des élus qui ne font pas partie de la structure, c'est-à-dire de autant d'avoir une 2ème assemblée consultative. Bénéficiant de ses droits d'information serait parfaitement cohérent. Autant de faire siéger dans la même assemblée. Et à ce Et à ce moment-là je me mets à la place du président de l'Assemblée, ça ne sera pas très facile de répartir les interventions entre les élus responsables et les élus qui sont des témoins. Donc c'est à mon avis une première faiblesses du système et puis la deuxième tout de même et en écoutant le collègue à l'instant qui parlait des conséquences sur l'environnement, sur les voisins, les voisins, c'est que la liste des bénéficiaires de cette participation et ses droits à l'information elle est trop réduite, elle ne porte que sur les communes directement support de des des usines cette c'est-à-dire. De communes à ma connaissance, dans les Yvelines. Alors que il y a évidemment un nombre de communes directement intéressés qui est beaucoup plus important. Donc si j'avais une suggestion à faire pour la suite du travail, ce serait tout simplement de se servir de l'accord qui a été conclu il y a quelques années en créant un comité. Certes annuel donc insuffisant d'informations information mais dont le tour de table. La liste le communes participant est beaucoup plus logique et à ma connaissance en tant que voisin. La liste des communes associées à ce que ce comité d'information n'a plus été discuté. Donc il me semble que dans la suite des travaux. Il faudra élargir mais en effet puisque c'est une disposition légale, il faut que la liste des communes qui dure dans la disposition législative, mais il faut élargir la liste des des communes d'une part et d'autre part, prévoir une une instance voisine et et éventuellement concomitante du comité syndical du du conseil d'administration. Mais en revanche il n'est pas logique et sauf erreur, personne ici n'a jamais vu ni n'a jamais proposé de faire siéger dans la même assemblée des représentants consultatif et les représentants responsable, donc c'est la raison pour laquelle, répondant à l'appel de la ministre l'utiliserait le peu de sagesse dont je dispose pour m'abstenir. Merci, cher collègue, la parole est à madame Marie-. Pierre de La Gontrie pour le groupe socialiste, écologiste et républicain pour cinq minutes également. Madame la présidente. Madame la la ministre. Monsieur le président de la commission, madame la rapporteure. Je voudrais tout d'abord remercier les collègues non franciliens de d'assister à nos débats. Qui ne sont pas très poétique. Mais. Qui sont néanmoins très important dans notre région, puisque cela a été rappelé. Ce syndicat interdépartemental concerne 9 millions d'habitants. Un budget qui n'a pas été évoqué mais d'un milliard trois. Et concerne 187 communes d'Île-de-France. Donc évidemment cela. Est nécessairement intéressant et et et indispensable pour les élus que nous sommes. Au-delà, le texte qui nous est proposé aujourd'hui et finalement. Il pourrait reprendre une formule facile. Une mauvaise réponse à une vraie question. En tout cas une réponse qui n'est pas totalement satisfaisante à une question qui semble totalement pertinente. Quelle est la question. Il semble que les élus. Et ça n'est pas contestée, soit insuffisamment informés lorsqu'il se passe ce qu'on appelle pudiquement un incident. Dans l'unique installation à ce jour, qui se trouve donc dans les Yvelines et qui couvre semble-t-il. 3 communes distinctes, mais voilà. Et qu'effectivement on peut comprendre que ces stations classées Seveso lorsqu'il se passe quelque chose d'inhabituel. Puisse évidemment inquiétés de manière totalement les gitans légitime les habitants et. Évidemment au 1er chef les élus. Il se trouve que à cette époque. La gestion du Siaap la gouvernance du Siaap que sais-je n'ait pas cru devoir associer de manière suffisamment. et que donc. Les élus de ce département, mais aussi du département voisin du Val-d'Oise et manifesté depuis lors. Ce qu'on peut appeler une mauvaise humeur caractérisée. En indiquant que la meilleure solution était sans doute de rentrer au conseil d'administration. Lorsque je dis mauvaise réponse c'est pas du tout pour être péjorative avec la proposition notre collègue Marta de Cidrac mais on voit bien que la proposition initiale qui consistait à faire entrer dans le conseil d'administration. Les communes non pas sur lequel se situent les stations, la station mais toutes les communes potentiellement concernés sans d'ailleurs on sache très exactement définir la liste. Aurait transformé le conseil d'administration du Siaap qui se réunit tous les mois. En une assemblée d'une ampleur qui n'aurait pas rendu la possibilité d'un d'un travail sérieux. Atteignable. Donc ce qui a été. Proposé. Par amendement et qui a été adopté par la commission c'est effectivement de restreindre le Champ de ces communes, puisque seules les communes sièges une station dont 3 communes. Nous sommes en train de légiférer pour trois communes. Puissent être conviés au conseil d'administration avec un statut de voix consultative. Alors on voit bien le le le côté Alain Richard là dit totalement hybride de cette formation puisque nous allons être dans un syndicat. Interdépartemental qui va associer des communes qui n'auront pas de statut délibératif mais qui pourront tout de même assisté et pour lequel ça peut ne pas répondre au souci d'information parce que il y a Dieu merci rarement des incidents. Mais même si le conseil administration se réunit tous les mois. Il ne se réunit pas nécessairement le lendemain de l'incident. Donc la question est vraiment de l'amélioration de la gouvernance du Siaap. Avait été proposé à la Richard l'rappelé par le préfet Gaudin l'instauration d'une conférence qu'on peut appelle parfois conférence des territoires qui a ensuite un autre nom, en l'occurrence conférence. D'assainissement. Je crois qu'rassembler l'ensemble des communes concernées. C'était nous semble-t-il la meilleure chose alors elle ne se réunissait qu'une fois par an, insuffisant bien sûr mais pour notre part pour mon groupe nous avions proposé que cette conférence soit instituée par la loi. Et qu'elle se réunissent. À une fréquence beaucoup plus importante et cela nous semble toujours la voie la plus intéressante pour l'ensemble des élus, puisque je le rappelais, il y a 187 communes. Alors, le texte a été modifiée en législation en commission les voix délibérative sont devenus consultative. Le nombre de communes concernées a été restreint et de ce fait, même si nous légiférons donc aujourd'hui pour faire entrer 3 communes avec voix consultative au conseil d'administration du Siaap je ferais au nom de mon groupe comme Alain Richard, preuve d'une sagesse extrême et nous nous abstiendrons. Merci, cher collègue, la parole est à madame Laurence Cohen pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. Pour cinq minutes. Madame la présidence de Madame la Ministre, mes chers collègues, la proposition de loi de notre collègue Marta de Cidrac pose une vraie question et entend répondre à un problème légitime. On se souvient toutes et tous, ici, du manque d'information des élus locaux, notamment face aux différents incidents qui ont touché les stations d'épuration du syndicat d'assainissement de l'agglomération parisienne le Siaap notamment la fuite de plusieurs tonnes tonnes de biogaz. Il est tout à fait légitime que l'information notamment lors d'incidents graves puissent être directement transmise aux élus afin qu'il puisse gérer la crise comme il se doit et communiquer. De leur côté si nécessaire. Mais est-il pour cela nécessaire de modifier la gouvernance de ce syndicat. Peut être qu'améliorer le circuit de l'information serait déjà suffisant. Le Siaap propose une conférence d'information annuelle de l'assainissement de l'agglomération parisienne, qui regroupe 100 compétence délibérative l'ensemble des élus des communes. EPCI ou syndicats des territoires raccordé au par voie statutaire ou conventionnelle là aussi des améliorations pourraient être apportées en prévoyant notamment des conférences plus nombreuses à raison d'une par trimestre par exemple. De plus cette PPL créerait une sorte de rupture d'égalité entre les différents élus alors que ce sont des conseillères et conseillers départementaux de la petite couronne qui siège au conseil d'administration, là on va faire entrer des conseillers municipaux et encore triés sur le volet puisque ce serait uniquement celles et ceux de grande couronne, à savoir du département des Yvelines. Les départements de l'Essonne, de la Seine-et-Marne et du Val d'Oise ne possédant pas de station de traitement des eaux usées. Nous considérons que cet élargissement entraînerait un déséquilibre au niveau de la gouvernance et de la composition du Siaap ce qui ne nous semble pas opportun. Le fait que la rapporteure et modifier le texte en permettant uniquement une voix consultative et non délibérative nous paraît plus cohérent et encore une fois plus respectueux des équilibres actuels de gouvernance. Mais cela ne suffit pas convaincu de l'importance de mieux associer les communes ils nous sommes tout aussi important de le faire de manière responsable pour que chacune et chacun puisse s'y retrouver les élus municipaux qui sont élus de la strate de collectivité la plus décentralisée méritent de savoir en effet ce qui se passe sur leur territoire mais aussi de comprendre et d'anticiper les décisions du Siaap autant en petite qu'en grande couronne. Il y a sans nul doute des améliorations apportées à la gouvernance du Siaap. Mais. Le syndicat d'assainissement de l'agglomération parisienne a décidé l'augmentation de la partie assainissement de la facture d'eau pour certaines villes du département de l'Essonne, ceux par exemple sans consultation. Aucune des villes de grande couronne concernés non représentés dans son conseil d'administration. Donc on voit bien qu'il y a besoin effectivement de réfléchir à tous ces manquements, mais franchement, est-ce que la réponse. Va résider dans le fait de faire entrer quelques élus supplémentaires au conseil d'administration. J'en doute énormément. Cette proposition de loi en l'état ne semble pas du tout satisfaisantes, elle servira l'intérêt de quelques-uns sans prendre en compte globalement la réalité de chaque commune francilienne. Mais évidemment comme beaucoup de de mes collègues, je vais exercer un pouvoir de sagesse, ainsi que l'ensemble des membres de mon groupe et nous avons décidé de nous abstenir ce cette sur cette proposition. tout en rappelant que la dépollution des eaux usées d'environ 9 millions de Franciliens et Franciliennes des eaux pluviales et des eaux industrielles de 400 entité est un véritable enjeu politique et que cette PPL ne répond ni aux anges ni aux ambitions qu'on pourrait. Avoir je vous remercie. Merci cher collègue. La parole est à monsieur le président Laurent Lafon pour le groupe Union centriste a pour cinq minutes. Madame la présidente. Madame la Ministre, Monsieur le président de la commission des lois, chers collègues. Le Siaap est une vieille machine comme toutes les vieilles machines. Sa mécanique est solide et bien rôdé son ne outillage robuste et opérationnel l'obsolescence programmée, ne le concerne pas. Mais comme toutes les vieilles machines. Il arrive qu'il faille en huiler les rouages, faute de quoi il s'encrasse et perdent de leur fiabilité. Nous avons tous à l'esprit et nombre de nos collègues le rappeler. Les incidents fâcheux causé par la l'activité récente du Siaap dans la nuit du 9 au 10 octobre 2022, notamment plus de 4 tonnes de biogaz ont été accidentellement relâché dans l'atmosphère des Yvelines par l'usine Seine Aval qui est la plus importante station d'épuration d'Europe. Sans que la préfecture les élus ou la population locale n'en soit immédiatement alerté. À plusieurs autres reprises. Le syndicat a tardé à informer les communes de ce qui se passait sur leur territoire. Ce défaut de communication répétées et sans compter hein. Sans conteste un raté de la machine CIAT. Je remercie à ce titre, notre collègue Marta de Cidrac auteur de la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui d'avoir soulevé la question importante des défaillances du Siaap à travers cette proposition de loi. Je salue également le travail de notre rapporteure Catherine Belghiti sur ce texte, ainsi que les éléments apportés au débat, par l'ensemble des commissaires. Aux lois du Sénat avec mes collègues de l'Union centriste. Nous ne pensons pas que la solution aux problèmes constatés réside dans un changement de machine car c'est bien de cela qu'il s'agit la présente, proposition de loi prévoit de créer un objet juridique non identifié combinant, départements et communes au risque de créer un précédent hasardeux qui viendraient encombrer l'activité de nos assemblées. notamment d'intégrer les représentants des conseils municipaux des communes concernées par l'activité des stations d'épuration au conseil d'administration du Siaap avec voix consultative. Mais si l'objectif est de renforcer le partage d'informations entre les élus locaux et le syndicat de fluidifier la communication de crise. À quoi bon les convoquer à une réunion mensuelle qui arrivera systématiquement soit trop tôt, soit trop tard. Face à l'urgence au problème. la situation la la plus problématique et celle de l'usine Seine Aval dans les Yvelines. Les incidents successifs y étant survenue. Ont légitimement indignés les élus de ce territoire qui n'ont pas été suffisamment Il n'est pas normal en effet que les représentants du conseil départemental des Yvelines ne siège pas au conseil d'administration du CIAT l'adhésion de ce département, syndicats et donc nécessaire mais il s'agit d'une décision pouvant être prises par simple délibération du Siaap nul besoin d'une loi de nous trompons pas de véhicule Peillon en outre à ce que la réponse apportée aux défaillances du Siaap soient bien dimensionnées aucune station de traitement des eaux usées n'est implantée à ce jour en Essonne en Seine-et-Marne ou dans le Val d'Oise la présente, proposition de loi mentionne pourtant ces départements qui n'ont pas vocation, me semble-t-il à rejoindre le Siaap à court terme. pour rassurer les élus et les habitants des territoires concernés par l'activité du syndicat. Nous avons besoin d'une meilleure communication de crise et d'un élargissement ciblé du Siaap au département des Yvelines. Ni l'une ni l'autre de ces solutions n'est retenu par le texte que nous examinons aujourd'hui aussi avec la majorité de mes collègues du groupe de l'Union sont centriste, nous nous abstiendrons par rapport à dans. Cette proposition de loi. Je reconnais toutefois à à nos débats et à cette proposition de loi la vertu de mettre en lumière les dysfonctionnements réels du système d'assainissement des eaux en région parisienne dont pâtissent de nos concitoyens. Ces échanges auront je l'espère, l'effet d'un électrochoc pour les responsables du siège du Siaap même si la vieille machine se doit de disposer. Au XXIe siècle, des canaux de communication moderne et efficace. J'espère que cet électrochoc de. Mise en oeuvre à travers cette PPL aura. Pour résultat de leur faire prendre conscience de la nécessité de s'ouvrir davantage. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Jean-Yves Roux pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen pour cinq minutes. Madame la présidente, madame la Ministre, madame la rapporteure. Monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues. Notre groupe a l'habitude de défendre les causes de la ruralité, laquelle ouvrent trop souvent d'une forme de décrochage d'inadaptation institutionnels à l'heure de la métropolisation. Mais je constate sans m'en réjouir que même les territoires les plus urbaine, notre pays connaissent des difficultés, notamment lorsqu'il est question de concertation dans la prise de décision. En toute transparence. J'ai découvert à l'occasion de cette proposition de loi, l'importance des difficultés rencontrées par le service public de l'assainissement francilien. Les incidents recensés en 2019 et en 2022 dans la station d'épuration d'Achères en. De quoi provoquer de l'inquiétude, voire de la colère de la population locale et aussi chez les élus qui peuvent légitimement souhaitez participer davantage à la gestion du Syndicat interdépartemental d'autant plus que ces incidents sont d'une importance majeure et interviennent dans une des plus grandes usines d'Europe. Cela a déjà été souligné mais nous parlons tout de même d'une fuite de plusieurs tonnes de biogaz, laquelle avait pu conduire en 2019 pour parler de manière très concrète à ce que de nombreux poissons soient retrouvés morts dans la Seine et sur les rives du fleuve dans les Yvelines où le Val-d Oise. Nous conviendront que ce genre d'images n'aident pas à rassurer nos concitoyens. Quand bien même on expliquerait que les produits hein. Fuite ne représenterait pas de danger pour les habitats aussi au regard des circonstances, il est effectivement inquiétant que les élus locaux n'ait pas été informé comme il le faudrait de ces incidents, ou l'été avec du retard. Je rejoins donc la remarque de notre collègue Marta de Cidrac l'absence de circuit efficace d'information à l'égard des élus locaux qui est nécessaire aux mains de l'inquiétude parmi les habitants des communes concernées. Par principe, notre groupe est favorable à toute disposition qui participeraient à mieux associer à informer les élus des communes et dans ce cas précis à toute disposition et qu'qui participerait à mieux associer les communes accueillant des stations d'épuration des eaux usées, gérée par le sien. L'actuel gouverneur du syndicat a été critiqué à juste titre plus spécifiquement, il a été admis de manière assez consensuelle et qu'elle n'avait pas permis que cette bonne information des élus des départements non maman du cap sur le territoire desquelles des incidents graves s'était produit. Nous saluons donc l'initiative de notre collègue qui répond aux souhaits des élus de pouvoir prendre part à la gouvernance de cet établissement public. Nous saluons également les travaux menés par notre rapporteur et qui a cherché à améliorer la proposition à la rendant davantage opérationnel. Le texte initial proposé que des représentants des conseils municipaux des communes sur lesquelles sont implantées les stations d'épuration des eaux exploité par le Siaap ou des communes situées à proximité de ces stations siègent avec voix délibérative au conseil d'administration et au bureau du conseil administration du syndicat. Cela permettrait effectivement de rhésus dans le déséquilibre observé au sein de la gouvernance et de limiter également certaines difficultés à en matière de communication des informations. J'entends toutefois les craintes qui ont résulté de cette modification statuaire du syndicat. Personne ne peut prévoir les incidents dans le futur de ce changement. Le nombre de sièges, a ajouté le caractère délibérative des voix des nouveaux représentants restaurer une source d'imprévision, voire d'instabilité. La commission des lois et apporter un ajustement Arenc trains autour des seules communes situées le territoire de département non du et ayant leur territoire, une station de traitement des eaux usées exploité par ce syndicat. Je soutiens ce dispositif qui adoucit nettement l'effet de la modification tout en permettant. Tendre d'atteindre le but initialement visés. De la même manière, je soutiens l'ajout de mécanismes améliorant l'information des conseils municipaux des communes ainsi concernés par le traitement des eaux usées par le sien. C'est un apport essentiel à la transparence de la vie publique et administrative. Vous voulez dire, vous l'aurez donc compris mes chers collègues, le groupe RDSE votera en faveur de la proposition de loi. Merci cher collègue. Alors je vais mettre aux voix, la proposition de loi visant à renforcer la voix des élus locaux au sein du service public de l'assainissement francilien. J'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe Les Républicains. Alors il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

Plus personne ne demande à voter. Le scrutin clos. Alors résultat du scrutin. Nombre de votants, 343. 184 pour, 184 contre 0 la proposition est adoptée. Mes chers collègues. La conférence des présidents, avaient prévu de siéger éventuellement le dimanche 5 mars pour l'examen du projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale pour 2023. Au vu du nombre d'amendements déposés sur ce texte et en accord avec la commission des affaires sociales. Je vous confirme que nous siégeons effectivement ce dimanche à 9h 30 à 14h 30 et le soir. Par lettre en date de ce jour, le gouvernement demande l'inscription à l'ordre du jour du mardi 21 mars après-midi sous réserve de leur dépôt de la lecture des conclusions des commissions mixtes. Paritaires sur la proposition de loi visant à ouvrir le tiers-financement à l'état à ces établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique et sur la proposition de loi tendant à renforcer l'équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs. Ils demandent également l'inscription à l'ordre du jour du mercredi 22 mars après-midi et éventuellement le soir de la suite éventuelle de la proposition de loi portant fusion des filières à responsabilité élargie des producteurs d'emballages ménagers et des producteurs de papier et amplification des encarts publicitaires destinée à informer le public sur la transition écologique. Acte et donner de ces demandes le délai limite pour les inscriptions de parole sur les conclusions de ces commissions mixtes paritaires serait fixée au lundi 20 mars à 15h. Y a-t-il des observations. Je n'en vois pas. Il en est ainsi décidé. Je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 21h 40 pour le débat sur la mixité sociale à l'école, la séance est suspendue.